Madame la première ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je vous prie d'excuser le président du Sénat, en déplacement à Colombey les 2 églises. Je vous rappelle que la séance est retransmis en Direct sur Public Sénat et sur notre site Internet, au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun de vous, mes chers collègues ah observé au cours de nos échanges, l'une des valeurs essentielles du Sénat le respect qu'il s'agisse du respect des uns et des autres ou de celui du temps de parole. La parole est à madame Christine Lavarde. Pour le groupe républicain. Madame la première ministre, cette question vous étiez adresser car elle concerne plusieurs membres de votre gouvernement et je vois qu'il a été choisi pour me répondre, quelqu'un qui n'a pas assisté au débat dont il va être question, un de nos illustres prédécesseurs sur ces bancs Asie que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, alors ma question va être en 2 temps : tout d'abord la forme, comment pouvez-vous oser redéposer par l'intermédiaire d'un 49 3, une disposition qui a été rejetée par les 2 assemblées, une première fois à l'Assemblée nationale, une deuxième fois au Sénat et cette disposition d'ailleurs a été déposé en catimini, car elle ne figurait pas dans les amendements retenus dans la première version du texte si on l'a vu arriver dans le texte consolidé envoyée le jeudi matin aux assemblées, je parle là des contrats de confiance au contrat de Cahors et donc j'en arrive maintenant à ma question sur le fond, madame la première ministre, cette disposition va-t-elle être remise une fois que le Sénat leur a supprimé lors de l'étude de la du PLF pour 2023 dont le 49 3 qui sera de nouveau déposé à l'Assemblée nationale.

Monsieur le monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice là-bas de quoi s'agit-il, je pense que vous faites référence à l'article 23. Et à un processus législatif que je souhaite reprendre quelques instants. Au moment de du début de ce quinquennat la première ministre a souhaité que la nature des relations que nous puissions engager avec les associations d'élus changent de nature, ça a donné lieu à une rédaction initiale, celle effectivement d'un dispositif qui tournait le dos, contrat de Cahors qui supposait des engagements individuels ont préfecture avec des trajectoires assorti de sanctions qui était très automatisées pour arriver un schéma pas saluée par toutes les associations d'élus mais par certaines d'entre elles comme étant une évolution du dispositif de dialogue, je pense en particulier intercommunalité de France et la défaite et l'ADF, pardon, qui repose sur l'idée d'arrêter un objectif global de dépenses publiques dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques et qu'à l'issue des comptes administratifs 2023 par strates, on regarde où on en est et qu'on puisse ensuite seulement s'il y a des dépassements regarder à l'intérieur de la strate les collectivités qui dépasse le problème, c'est que ce dispositif dont on a besoin pour crédibiliser la trajectoire des finances publiques de la France, a été écartée, dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques, il a été décidé dans le cadre du PLF 2 réintroduire les articles dont nous avions besoin pour crédibiliser cette trajectoire des finances publiques et très concrètement, c'est une façon aussi de re provoquer le dialogue. On ne peut pas écarter d'un revers de main. J'ose espérer. J'ose espérer. Que ça n'est pas la nature de la relation vous aurez quand on va entrer dans le détail de ces articles, le gouvernement est prêt sur ce sujet à discuter mais il considère que la voie d'un compromis à la fois sur les finances des collectivités sur les finances de l'État nécessite précisément un travail de co-construction et le balayer d'un revers de main ne peut pas être une attitude responsable. Alors juste je voudrais revenir sur cette histoire de crédibiliser la trajectoire des finances publiques pour vous dire que les APUL, c'est 9 % de la dette publique, les APUL sont en excédent les APUL sur la période 2018, 2021, on fait des économies de 11 milliards par rapport aux tendanciel alors même que les contrats de corps avait été ajourné, alors je suis désolé mais cette crédibilité quand je cite le ministre Atal qui nous dit : si on veut contenir l'évolution de la dépense publique des collectivités territoriales, qu'il faut prévoir un mécanisme d'encadrement, c'est une question de crédibilité, mais alors pourquoi appelez-vous ça contrat de confiance et Monsieur le Ministre, Béchu, je suis désolé, mais je vais vous citer au mois de juin sur Public Sénat, vous indiquiez il est certain qu'on ne repartira pas sur les bases d'un contrat de corps qui consisterait à dire qu'il y a un pourcentage d'inflation à ne pas dépasser, vous avez récidivé début juillet au moment de l'inauguration de Landru, vous avez dit il va de soi que l'idée de penser que l'on va faire dans ce quinquennat la même chose que ce que l'on a fait dans le quinquennat précédent avec un contrat de Cahors, des objectifs n'existe pas, excusez-moi mais là c'est exactement la même chose qu'on nous propose et c'était même pire dans la version initiale puisque vous disant quadrillé le fonctionnement et vous veniez reprendre des dotations de l'État pour l'investissement des collectivités donc vous Betty et même à le financement de la transition. Président

monsieur le président, Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre du Travail. La COP27 s'est ouverte dimanche dernier à Charm el-Cheikh il s'agit d'un rendez vous déterminants pour l'avenir de la planète, nous ne pouvons que saluer les engagements pris par l'Europe et la France pour parvenir à la neutralité carbone en 2050 atteindre cet objectif va nécessiter des compétences, telle est l'objectif de ma question, celle des ressources humaines et de la transition, si nous ne prenons pas assez au sérieux, l'enjeu de la formation, la transition écologique pourrait demain se heurter à une pénurie de savoir-faire dans notre pays en ce moment même des soudeurs américain répare les défaut de corrosion sous contrainte de notre parc nucléaire, car nous n'avons pas assez de ressources humaines pour y parvenir seuls dans des délais resserrés actuel parmi les problématiques les plus parlante au sujet de la pénurie de compétences, on sait que le secteur des transports et l'un des gros émetteurs de gaz à effet de serre le ferroviaire va avoir un rôle clé dans le verdissement de ces secteurs, or une étude prospective menée par l'Observatoire des métiers de la métallurgie a récemment démontré que, d'ici à 2030 le le besoin en ingénieur ferroviaire serait de près de 14000 ingénieurs nécessitant plus de 7900 nouveaux recrutements en tenant compte des départs à la retraite, ce qui signifie que devrait sortir des formations supérieures spécialisés dans le ferroviaire, environ 790 ingénieurs par an, alors il n'en sort aujourd'hui que 250 la question est, en l'occurrence quantitative, mais elle est aussi qualitative, il faut former à la décarbonation, c'est particulièrement vrai dans le domaine des énergies renouvelables du nucléaire ou encore de l'agriculture telle était d'ailleurs le message de l'appel des étudiants de l'Agro ParisTech il déplorait, ne pas être formé à l'agro-écologie, monsieur le Ministre, à l'heure de la COP27 notre système de formation initiale et continue, a-t-il bien pris en compte l'enjeu de la transition et environnemental si oui comment merci. d'abord merci de rappeler par votre question, l'importance des transitions, l'importance des travaux menés lors de la COP27, mais pour vous répondre en 2 points : un 1er point simplement pour dire : vous avez 1000 fois raison sur ce pour ce qui concerne la formation initiale et la nécessité qu'elle soit orientée vers l'accompagnement des transitions et en particulier la transition écologique mon collègue ministre de l'Éducation nationale avec madame la ministre déléguée en charge de la formation professionnelle pourrait vous dire tout ce qui est fait en matière de réorientation de la formation de réorientation et de réforme de la voie professionnelle, justement pour avoir des formations qualifiantes qui permettent d'aborder l'avenir c'est vrai pour les études secondaires, c'est vrai pour les études supérieures à madame la ministre de l'enseignement supérieur, il veille aussi faire en sorte que notre appareil de formation initiale, hein, tellement les besoins de formation que vous avez évoquées mais au-delà de la formation initiale, nous devons aussi penser l'accompagnement des transitions pour l'ensemble des entreprises et l'ensemble des salariés, c'est la raison pour laquelle nous sommes aussi extrêmement attentif à ce que les entreprises puissent accompagner la transition en leur sein, vous avez évoqué le secteur du nucléaire, vous avez évoqué l'agriculture, vous avez évoqué le secteur de l'hydrogène et des transports, le secteur de l'automobile aussi est particulièrement concernés et nous devons faire en sorte, par la formation continue transition que des transitions collectives par les dispositifs de formation des salariés d'accompagner cette transition pour que celles et ceux qui ont été formés sur des techniques qui étaient des techniques d'excellence, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, puisse être à nouveau montée en pouvoir monter en qualification et à accompagner ces transitions dans le cadre de la loi de finances pour 2023, vous aurez l'occasion de le constater dans les prochains jours, plus de 350 millions d'euros ont été prévus pour réabonder le le Front national pour l'emploi, sur son volet formation le FN fait pour financer aussi les dispositifs de transition collectives et permettre, dans le cas du dialogue social, que les branches professionnelles se saisisse de ce besoin de reclassement, de formation et d'apport de nouvelles qualifications de nouvelles compétences à leurs salariés et ainsi répondre aux enjeux de transition que vous avez rappelé. Merci, monsieur le Ministre, la parole est maintenant à notre collègue Gérard Lahellec pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Merci monsieur le président, ma question s'adresse à monsieur le ministre des transports. Dans le contexte où se réunit la COP27 il est bon de rappeler que les transports représentent un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre. Mais pas en raison des politiques publiques, mais plutôt en raison de ce que ne font par nos politiques publiques, tout le monde s'accorde pour reconnaître que pour changer de cap, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et doubler la part des du ferroviaire d'ici 2030, ce n'est pas de mesurettes, dont nous avons besoin, mais au contraire d'une grande ambition publique il nous faut tout à la fois, développer le fret ferroviaire, assurer la remise à niveau de notre réseau par un tout autre contrat de performance ou encore, pourquoi pas développer les trains de nuit, donc la marge de progression est gigantesque, comme l'a rappelé et lourd rappelle constamment les mouvements des usagers, la désertion de nos territoires, il les difficultés de recrutement et précisément s'il est un thème sur lequel on peut agir, c'est bien sur le thème des transports, une majorité politique existe pour dégager des moyens supplémentaires à la fois au Sénat, comme en attestent les divers rapports adoptés ici mais aussi à l'Assemblée nationale ou un amendement au budget proposant 3 milliards d'euros supplémentaires pour le ferroviaire, a été adopté, disons-le avec des voix de gauche et les voix de droite, le gouvernement est-il prêt à s'emparer de cette situation inédite d'une majorité politique possible pour dégager des moyens afin de donner un nouvel élan au transport ferroviaire, merci.

vous avez raison d'insister sur cette priorité. Je crois, vous l'avez exprimé dans le ton, même de votre question, elle est largement partagée, il y a un consensus à la fois pour rappeler les chiffres que vous avez indiqué les c'est le transport, pardon, c'est 30 % des émissions de gaz à effet de serre et notre consommation énergétique, et donc nous devons lui donner une priorité très forte, notamment dans le transport ferroviaire et dans le report d'autres modes de transport vers le ferroviaire, le budget qui sera soumis à votre débat dans quelques jours, porte un effort extrêmement important en faveur des transports, notamment les transports publics, je tiens à le redire parce que c'est parfois un peu oublié notre débat, quand nous avons plus de la moitié de l'effort de l'État, au total 12 milliards d'euros, 6,6 pour le transport ferroviaire qui est consacré précisément aux trains et aux transports publics, je ne crois je crois que ce ne sont pas exactement ni des mesurettes, ni des cacahuètes budgétaire quand nous avons plus de 85 % du programme budgétaire des transports qui sont consacrés, pour la première fois au transport ferroviaire, je crois que nous sommes aussi dans une action importante, vous avez évoqué un certain nombre de domaines, plus précis, je pense au fret, nous avons un plan d'un milliard d'euros sur 6 ans qui est consacré au fret, qui vous sont chers et qui sont si importantes, c'est pour la première fois le 1er ministre Jean Castex avait initié d'ailleurs ce mouvement, ce sont les protocoles pour près à le 6 milliards d'euros qui sont aujourd'hui signés avec les régions pour investir sur plusieurs milliers de kilomètres de lignes, près de 6000 d'ores et déjà, devons-nous prolonger, amplifier cet effort ensemble, c'est exactement la démarche transpartisane que vous avez décrite, qui, à l'occasion de se déployer dans le cadre du comité du Conseil par une orientation des infrastructures à laquelle participent plusieurs membres du Sénat, comme plusieurs membres de l'Assemblée nationale, toutes sensibilités confondues, nous aurons ces travaux d'ici la fin de l'année et sur cette base, nous pourrons aussi définir une programmation des moyens et des priorités très claires pour le ferroviaire, en particulier, j'insiste sur un point, j'insiste sur un point qui est essentiel, c'est que le réseau ferroviaire doit être absolument prioritaire dans le choix budgétaires et c'est en plus la responsabilité de l'état du niveau national que d'investir encore davantage dans ce réseau, je veux dire que nous avons quasiment doublé les crédits qui sont consacrés ces 5 dernières années, donc nous avons engagé cette démarche, nous irons plus loin et nous le ferons ensemble. Merci, monsieur le Ministre Monsieur Lahellec. vous avez la chance de disposer de dispositions parlementaire saisissons je pense, l'occasion pour avancer. Merci, cher collègue, la parole au président Alain Richard pour le groupe Rassemblement des démocrates progressistes. C'est indépendant. Monsieur le ministre de l'économie, les entreprises industrielles de quelques secteurs fortement utilisateurs d'énergie, concentre une part importante des émissions de gaz à effet de serre celles qui opèrent en France ne font pas exception, mais nous savons tous ce que les décennies passées ont vu certaines industries disparaître et ce n'est évidemment pas de ce côté-là qui la solution pour l'avenir, la réduction efficace de nos émissions ne peut pas se traduire par une nouvelle désindustrialisation et par un gonflement de nos importations, les responsables de ces entreprises ont pour beaucoup d'entre eux progressé dans leur transformation et commencer à obtenir des résultats, le rythme de baisse des émissions des industriels français se comparent honorablement celui de leurs concurrents de l'Union européenne et des grands pays développés. Mais il faut aller plus vite, le président de la République a organisé une réflexion partagée avec ses dirigeants pour définir ensemble le meilleur programme d'action, le thème était : comment répondre à l'urgence climatique et soutenir les industries moderniser créative et compétitive pour produire de la richesse et développer de l'emploi qualifié en France Monsieur le Ministre, quels sont les grands engagements que le gouvernement veut obtenir de nos partenaires industriels et quels sont les grands axes du programme de soutien que vous pourrez présenter prochainement pour relever ce défi. Merci, cher collègue. Que le ministre Bruno Lemaire, ministre de l'économie. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, Alain Richard, je vais vous raconter une histoire. Pas une histoire à dormir debout. Voilà. Une histoire à rêver debout, c'est celle du site de Solvay, que nous avons visité ce matin avec le Ministre de l'Industrie, Roland Lescure, site qui a un siècle d'histoire industrielle derrière lui, un site qui produit des produits chimiques du carbonate de soude, du bicarbonate de soude, avec comme énergie du charbon importé de Russie incite donc émet beaucoup de CO2, qui a des problèmes de compétitivité et qui aujourd'hui ne répond plus aux standards les plus innovants et à nos exigences environnementales, ce site est en train d'opérer une révolution climatiques et industriels, il va transformer son énergie charbon en utilisant les déchets recyclables de tout le bassin tout le bassin géographique pour réduire son empreinte carbone améliorer sa compétitivité et ouvrir un nouveau Shia que d'histoire industrielle pour le site de Solvay, hé bien je veux rendre hommage aux ouvriers, aux ingénieurs, aux techniciens, aux entrepreneurs à Solvay qui opère cette révolution industrielle et environnementale cette décarbonation cette histoire à rêver debout, elle doit être l'histoire de tous les grands sites industriels français et notamment des 50 sites industriels que le président de la République a choisi auquel nous allons apporter 5 milliards d'euros d'aide immédiatement et 5 milliards d'euros d'aide complémentaire si jamais nous suivent dans cet objectif de décarbonation pour que nous ayons demain l'industrie mondiale la plus décarbonés de de la planète, voilà une grande ambition pour la France, et voilà l'objectif que nous nous sommes fixés avec le président de la République et pour tenir cet objectif, non seulement nous allons accompagner chacun de ces 58 mais nous allons compléter de de décision la première c'est évidemment accompagné toutes ces entreprises dans les mois qui viennent pour faire face à l'explosion leur facture d'énergie et pour qu'elle puisse accomplir cette transition en ayant le soutien de l'État à l'accompagnement de l'État et la 2ème décision c'est accélérer la mise en place d'une taxe carbone aux frontières, parce que la décarbonation de notre industrie, qui construira l'avenir industriel français doit se faire aussi sur la base d'une équité de concurrence en évitant d'importer des produits qui eux continuent à polluer et qui viennent du dehors des frontières de l'Europe. bien. Je vais passer maintenant la parole à notre collègue Émilienne Myrhol pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Santé et de la prévention, soins déprogrammé faute de lits, transfert hors région de certains patients enfants hospitalisés dans des services adultes, les services de pédiatrie sont saturés douleur cri de détresse, il y a quelques jours, et la situation tendue en pédiatrie n'est que l'arbre qui cache la forêt car c'est tout l'hôpital public qui est en voie d'effondrement, le vrai problème est structurel, les conditions de travail amène les personnels a quitter l'hôpital et des services, y compris aux urgences doivent être fermés face à cette situation, vous avez annoncé un plan pour soutenir les services obtention de l'hôpital de 150 millions d'euros, puis de 400 millions d'euros et enfin hier au détour du débat sur le PLFSS de 556 millions d'euros au total, et ce sans aucune nouvelle recette ces enveloppes successives, bien que Bienvenue sont l'illustration de votre pilotage à la petite semaine, malgré votre communication lambda, mais 2 fois inférieur à l'inflation et de fait, le gouvernement réduit les moyens du système de soins et l'hôpital public année la première victime, alors Monsieur le Ministre, à quand une réponse pérenne et d'envergure pour l'hôpital public. Merci, cher collègue, la parole à monsieur le ministre de la. Santé de la prévention Monsieur François Braun. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Miral, vous imaginez bien, et vous le savez, je suis de très près la situation des services de pédiatrie, plus généralement, la situation également de de notre hôpital public et de ses difficultés. Je peux vous assurer que l'ensemble des moyens disponibles sont mobilisés pour faire face à cette nouvelle nouvelle crise et à cette épidémie de bronchiolite Santé publique France d'ailleurs, ce matin, nous indiquait que c'est une épidémie qui dépasse les pics épidémiques que nous avons connu depuis plus de 10 ans. D'ailleurs, pour accompagner cette cette information, j'ai décidé ce matin, en complément de tout ce qui étaient déjà mobilisés de déclencher le plan or 100 spécifique à cette épidémie pour renforcer encore les moyens des des ARS et permettre que l'ensemble de l'hôpital puisse se concentrer sur ce problème particulièrement aigu aujourd'hui. Des mesures d'urgence ont été prises et le gouvernement et je remercie le Sénat a amené effectivement des moyens financiers supplémentaires pour faire face à ces difficultés, je vous rejoins lorsque vous dites que le problème est plus structurelle au sein de notre hôpital public et de notre système de santé et le ministère de la Santé, de la prévention ne doit pas et ne sera pas uniquement un ministère de crise mais un ministère chargé de refonder notre système de santé dans son ensemble, c'est d'ailleurs tout l'enjeu du Conseil national de la refondation en santé, qui a voulu le président de la République. J'ai commencé à rencontrer depuis une semaine, l'ensemble des professionnels bien sûr de la pédiatrie, mais l'ensemble des professionnels de l'hôpital, également en ce qui concerne plus spécifiquement la pédiatrie nous travaillons aux assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant, puisque tout le Champ de la santé de l'enfant mérite d'être réformé, nous aboutirons au printemps avec une feuille de route pour les années à venir, sur un de la santé de l'enfant dans les mêmes dates, nous aurons les résultats des différents CNR territoriaux et nationaux sur la santé pour la refondation de notre système de santé pour qu'il soit basée non plus sur l'offre de soins, mais bien sur la réponse aux besoins de santé de la population française, je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre, chers collègues, allez-y. Monsieur le Ministre, ne veut pas se cacher derrière l'épidémie de bronchiolite pour parler des problèmes actuels, vous avez fait des choix et ces choix, il faut maintenant les assumer, vous avez décidé de faire porter les 17,7 milliards d'euros de la dette Covid sur la sécurité sociale, créant 7 emmener son déficit, vous avez décidé d'exonération de cotisations qui sont passés en 5 ans de 39 à 71 milliards mais vous refusez, dans le même temps, toutes les propositions que nous avons pu vous faire pour trouver de nouvelles recettes, c'est donc que vous faites le choix délibéré du déficit pour la sécurité sociale et ce peut être ou sans doute au profit du système privé à but lucratif, alors Monsieur le Ministre, nous sommes à croisée des chemins : soit vous décidez d'abord nous d'hôpital public soit vous engagez enfin cette réforme structurelle, le groupe socialiste, écologiste et républicain, de son côté est claire et réclame une réforme urgente et pérenne, tenant compte du ratio patients personnel soignant sur tous les territoires. Et maintenant, la parole est de notre collègue Guilaine Pantel pour le groupe du Rassemblement démocratique et Social Europe. Monsieur le président, madame la première ministre, mesdames et messieurs les Ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre délégué chargé des collectivités territoriales. Vous êtes interpellé à intervalles réguliers dans cet hémicycle sur les ressources dont disposent les collectivités territoriales pour alimenter leur budget et assurer le bon fonctionnement des services publics locaux. Après la suppression progressive de la taxe d'habitation au cours du 1er mandat d'Emmanuel Macron l'année 2023 doit être marquée par une nouvelle étape de la transformation de la fiscalité locale, avec la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises la CVAE doit donc être supprimée après avoir vu son taux divisé par 2 en 2021 naturellement des mécanismes de compensation voient systématiquement le jour avec plus ou moins de réactivité, comme le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes, ainsi que l'ajout d'un coefficient correcteur dans les cas où le transfert ne suffit pas, or plusieurs or plusieurs arguments viennent se percuter avec ce système de suppression compensation si l'intention de ce gouvernement et d'enclencher une vraie décentralisation la disparition de taxe doit pas avoir pour effet de restreindre les ressources fiscales des collectivités territoriales, au point d'entraver leur libre administration et leur développement. Le contexte inflationniste nous prouve que les dotations de l'État, qui par définition ne sont pas dynamique de peuvent seul : satisfaire les besoins en fonctionnement et investissement des collectivités. Un exemple : la commune de Mumbai, la Lozère, perçoit une DGF de 25000 euros alors que le fonctionnement de l'école lui coûte 20000 euros par un C. Costa sont faits depuis bien longtemps, il est maintenant nécessaire de réinventer, à la fois les concours financiers de l'État et la fiscalité locale pour que les communes et collectivités rurales puissent se développer, accueillir de nouvelles populations et faciliter la création d'entreprise, en somme, le gouvernement a-t-il l'intention d'impulser une réflexion globale pour un système plus équilibré de ressources pour les collectivités, et notamment les plus rurales, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à madame Caroline Cayeux, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Pentel vous m'interrogez sur l'évolution des ressources des collectivités locales face aux suppressions des impôts locaux et au montant de la DGF des petites communes, tout d'abord faire un rappel, à savoir que les suppressions d'impôts sont une bonne chose pour le pouvoir d'achat des Français car elles Servent à leur augmenter et, d'autre part, elles permettent d'améliorer la compétitivité des entreprises, du côté des collectivités locales pour la taxe d'habitation, comme pour la CVAE il y a des compensations à l'euro près qui sont prévues, elles seront dynamique en clair pour revenir sur la CVAE à la demande des associations d'élus, nous leur avons consacré une part de TVA notamment, vous le voyez, la volonté du gouvernement, c'est bien de préserver l'autonomie des collectivités et j'y suis moi- même personnellement attaché en ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement après la forte baisse sous le mandat de François Hollande, la DGF a été stabilisé à partir de 2018. Avec le PLF 2023, ce sont 320 millions d'euros qui sont rajoutés pour la première fois depuis 13 ans dont 200 millions d'euros de hausse pour la dotation de solidarité rurale dont bénéficieront les communes de Lozère c'est un changement important demandé par de nombreux élus locaux et de parlementaires depuis de depuis de nombreuses années, alors faut-il aller encore plus loin, je sais que la Cour des comptes a proposé une au Sénat une réflexion très ambitieuse et pour ce sujet, comme pour tout ce qui concerne nos collectivités je reste évidemment à l'écoute de la chambre des territoires et de vos propositions, avant de conclure, je voudrais rappeler néanmoins que, au-delà des concours financiers de l'État, le gouvernement a mis en place une politique ambitieuse pour accompagner

Merci. Mais le respect du temps de parole fait partie de notre règle du jeu commune la parole à notre collègue Monique de Marco, pour le groupe Écologie Solidarité territoires. Monsieur le Président, Madame la Ministre parlons festival j'avoue être un peu perdus, je ne sais plus si je dois m'adresser au ministre de l'Intérieur, ou à vous, Madame la Ministre de la culture, pourquoi le 25 octobre le ministre de l'Intérieur, monsieur Darmanin a présenté le dispositif de sécurité des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 près de 45000 policiers et gendarmes seraient mobilisés de juillet à septembre face à l'ampleur de ce dispositif, il a évoqué je cite la possible annulation ou le report de tous les événements en France qui demandent des unités de forces mobiles à l'heure des programmations des organisateurs de festival, les syndicats, les centaines de milliers de travailleurs du secteur et les millions de spectateurs s'inquiète faute de services de sécurité suffisant les faciles valent seront-ils sacrifiés pour les Jeux olympiques. Les festivals sont l'image de la France et de son exception culturelle ils garantissent une offre culturelle diversifiée dans l'ensemble du territoire en attirant des millions de de personnes leurs retombées financières sont également conséquentes, par exemple, les FrancoFolies de La Rochelle, génère 11 millions d'euros, le festival d'Avignon 50 millions d'euros et les fêtes de Bayonne attire chaque année un 1000000 de personnes si l'activité financière festivalière est annulée, qui assurera les conséquences financières l'annulation ou le report serait catastrophique pour un secteur qui peine à se remettre de la pandémie, la culture ne doit pas être une nouvelle fois la variable d'ajustement de décisions nationales, vous avez tenu une réunion avec les acteurs de la filière, le 2 novembre qui n'a pas permis de répondre à leurs inquiétudes, vous n'avez apporté ni solution ni réponse, il ne suffit pas, Madame la Ministre, de dire que vous êtes conscient des enjeux, nous voulons savoir qui sera concerné, quand, comment et dans quelle mesure, comme tous les acteurs du spectacle vivant et de la musique, nous attendons des réponses claires et des engagements, je vous remercie. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice de Marco, vous avez raison de dire que la France est une terre de festivals, que c'est une partie importante de l'ADN culturel de la France, notamment l'été, et vous avez raison de mentionner toutes les retombées économiques pour les territoires qui sont majeurs, mais nous savons aussi que l'organisation des Jeux olympiques, c'est un moment exceptionnel hors norme, c'est une fois par siècle, ça va être un grand moment festif et populaire qui nécessite une organisation hors norme et évidemment une sécurisation particulièrement renforcées, or les festivals aussi ont besoin d'être sécurisés, les festivals mobilise pour les très très grands festivals qui mobilise des dizaines de milliers de personnes, des unités de forces mobiles, donc le travail que nous sommes en train de faire avec Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra c'est ce travail enfin au cas par cas des situations les plus impactés pour chercher les solutions pour voir comment concilier le mieux possible, cette vitalité culturelle des festivals et les nécessités de sécurisation pour eux comme pour les Jeux olympiques, mais il a aussi l'enjeu des moyens techniques des personnels, des tensions sur les bénévoles sur les transports des spectateurs, c'est un ensemble de paramètres en réalité qui impacte les festivals et qui nécessite un travail au cas par cas, phase par phase avec les professionnels, vous l'avez dit, je les ai reçus assez longuement, je poursuis le travail en bilatéral, si je puis dire, avec chacun d'entre eux et avec leur syndicat leurs organisation professionnelle, nous sommes en train dans les semaines qui viennent, nous verrons se dessiner, certaines solutions et et je pourrais vous en faire part, nous sommes pleinement conscients de cette nécessité de concilier la force des Jeux olympiques et la force des festivals. Je vous remercie. Merci madame la ministre, la parole est maintenant à monsieur Pierre Jean Verzeaux laine pour le groupe, les indépendants. Monsieur le Ministre des transport, que se passe-t-il à la SNCF, que va faire la SNCF nous savons bien que vous vous êtes pas de président de cette entreprise publique, mais enfin, l'État en est l'actionnaire unique. En général, 5 pour 100 des trains annulés, c'est ce qu'on appelle un trafic normal à la SNCF mais nous quand nous constatons tous que depuis quelques semaines et de quelques mois, la situation se dégrade, je vais prendre l'exemple d'une région que je connais bien, celle des Hauts-de-France, en plus des retards depuis le mois d'avril, c'est près d'un train sur 10 en moyenne et chaque jour qui est annulé, ce qui crée un climat de tension et d'anxiété pour les usagers et, évidemment, et notamment ceux qui travaillent, la raison principale qui est invoqué, c'est le manque de personnel, on peut aussi et notre collègue là fait pointer le sous-investissement chronique dans le réseau secondaire depuis 30 ans, ce manque d'anticipation de la part de dirigeants d'un grand groupe public paraît aberrant comment en sommes-nous arrivés là et comment la situation va se rétablir. Grave. Monsieur le Ministre, la SNCF prend de plein fouet la hausse des prix de l'électricité, quid du bouclier tarifaire pour protéger les voyageurs de la hausse du prix des billets déjà que nous savons que le train n'est pas forcément plus attractif que la voiture ou l'avion au moment où la France prend des engagements à la COP27 on ne peut pas se satisfaire que le moyen de transport le plus économe en CO2 soit financièrement le moins intéressant, j'ajoute que les régions en charge des TER sont censés, je dis bien censé avoir un dialogue quotidien avec la SNCF, elles sont confrontées à un manque de transparence de la part de l'entreprise et aussi de ce qu'on peut appeler le triangle des Bermudes de la SNCF, c'est-à-dire une organisation enfin où il y a tellement d'interlocuteurs, on ne sait plus qui fait quoi, on ne sait plus qui vous répond et personne ne sait vous dire oui ou non, monsieur le Ministre, comment retrouver cette relation de confiance entre les régions et la SNCF : comment rétablir l'offre de trains et comment la SNCF va répercuter ou pas, la hausse du coût de l'énergie sur le prix des billets merci. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre, Clément Beaune. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Vert de vous avez raison, je n'ai pas l'habitude de fuir mes rêves. On s'habiliter nous parlons d'un grand service public qui doit être prise entièrement public et donc cela ne peut pas rester sans réponse ou faire face à un quelconque désintérêt de la part de l'État, c'est la raison pour laquelle je l'ai dit la situation Les France est inacceptable et nous avons eu un entretien puisque les TER sont effectivement la charge des régions avec le président, Xavier Bertrand, je me suis rendu à Lille dès lundi, et je me suis sûr entretenu hier avec le président Farandou, une nouvelle fois il y a un effort exceptionnel de formation qui est fait pour compenser ce que vous avez décrit, c'est-à-dire une pénurie de conducteurs qui, malheureusement, parce que cela fait partie des métiers en tension ne concerne pas que la région Les Hauts-de-France mais concerne très fortement très douloureusement les usagers du France, aujourd'hui qui a été tout à fait exceptionnel qui a été mis en place ces derniers mois, qui prévoit en 2022 2023 le recrutement inédit de 440 collaborateurs TER en haut de France mais j'ai demandé au président Farandou face à la gravité de la situation, un plan exceptionnel d'urgence et d'accélération de ces recrutements par tous les moyens possibles, qui sera présenté par l'entreprise dans les prochains jours, en lien avec la région, car cette situation ne peut rester sans réponse, je l'ai dit, très honnêtement, une situation de cette nature ne se règle pas en quelques jours, elle ne se résout pas totalement quelques semaines mais nous devons montrer des améliorations visibles sérieuse dans les toutes prochaines semaines pour les usagers, vous avez parlé aussi de la question tarifaire cela doit mérite mérite pardon quelques précisions : d'abord les tarifs qui sont justement ceux du TER et de beaucoup de trains, des quotidiens ne relève pas de l'État, les tarifs en revanche qui sont ceux des trains à grande vitesse ou des trains d'équilibre du territoire sont de niveau national est du ressort national c'est dans ce contexte que j'ai demandé pour ces trains à la SNCF de mettre en place un bouclier tarifaire qu'est-ce que cela signifie concrètement, cela signifie que nous devons d'abord agir pour réduire les charges de la SNCF, c'est ce que fait l'État par les mesures que nous prenons sur la maîtrise des coûts de l'énergie qui a permis de réduire très fortement le montant qu'évoqué devant le Sénat, le président Farandou près de 2 milliards d'euros, nous ne sommes plus du tout dans cette sorte de grandeur ensuite d'avoir des hausses qui soit, en tout état de cause, inférieure à l'inflation et 3ème point de préserver ceux qui ont le plus besoin du train, les ménages modestes, les utilisateurs réguliers, notamment pour le travail, c'est pourquoi je demande un effort tout particulier sur les abonnements et sur les bigots, ce plan sera présenté là aussi dans quelques jours par la SNCF, je vous remercie. la parole est maintenant à notre collègue Philippe Dominati pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, mes chers collègues, la France est à sec à sec d'argent à sec d'eau sec d'électricité à sec de gaz à sec de nucléaire à sec, de médecins et maintenant à sec de certains médicaments. Spasfon et Gaviscon nous cherchons amoxicilline et paracétamol aussi rare que le pétrole en cette épidémie de bronchiolite c'est dramatique ce sont pourtant des médicaments matures peu onéreux et essentiel, tout au long de l'année, alors ma question, monsieur le ministre de la Santé est aussi simple qu'elle inquiète les professionnels de santé et les patients. Quelle est votre stratégie pour que la France puisse retrouver sa souveraineté sur les produits de santé.

Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le, le sénateur Bruno Belin, le président de la République a fixé un cap lors du Conseil stratégique des industries de santé de 2021 réindustrialiser garantir notre capacité d'approvisionnement et notre souveraineté tout en maintenant un taux de croissance de l'industrie du médicament supérieure à 2 %. Nous avons 2 enjeux favoriser d'une novation sous soutenir l'accès aux médicaments innovants, mais aussi maintenir l'accès à des médicaments plus anciens mais particulièrement utile, vous parliez du paracétamol, c'est bien sûr un enjeu majeur de santé publique des obligations ont été renforcées pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeure des obligations au niveau du volume des stocks des obligations également au niveau des moyens et des dispositifs d'alerte en cas de craintes de rupture toutefois et et je vous rejoins nous connaissons en ce moment des tensions liées à la reprise covid sur certains médicaments, plus que sur certains médicaments sur certaines formes de médicaments par les de l'Amoxicilline, en particulier le sirop Amoxicilline et difficile d'accès, alors que les autres formes d'amoxicilline sont facilement accessibles, vous évoquez la bronchiolite, j'en profite et je suis obligé dans cette semaine de l'antibiorésistance de bien préciser que la bronchiolite est une maladie virale sur lequel il ne faut pas donner d'antibiotiques, au risque de développer l'antibiorésistance. Je suis bien sûr ces situations en temps réel avec l'Agence nationale de sécurité du du médicament situations qui sont complexes et j'ai demandé toute la transparence aux industriels, il est difficile de faire la part des choses entre

je vous rappelle que dans le cas de du plan France 2000 37 5 milliards d'euros ont été mis dans cette filière, à titre d'exemple et vous parliez du paracétamol, l'année prochaine, ouvre en Isère, une usine qui va produire 10000 tonnes de paracétamol par an pour en couvrir largement le marché français, je vous remercie. Monsieur Bala. Je prends acte de votre réponse Monsieur le Ministre, et je pense que vous-même et votre collègue Agnès Firmin Le Bodo aide de bonne volonté. Mais, mais le sirop typhon c'est fini à vouloir asphyxier le médicament et surtout son prix Bercy depuis des années, a tué une industrie nationale stratégique, le coup de la panne du Doliprane et révélateur d'une France exsangue, la réalité c'est Sanofi, incapable de faire un vaccin, la réalité c'est des médicaments contingentées, tous les matins, la réalité c'est un accès plus compliqué à la santé, c'est une récession indiscutable de la puissance santé de la France, la mascarade des masques à illustrer de façon insoutenable cette impuissance cette faiblesse. Il faut réindustrialiser la France car aujourd'hui ce sont des médicaments qui manquent. Le combat pour la santé et donc celui pour la vie passe par là, je vous remercie, monsieur le président. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à notre collègue Rémi Cardon pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci monsieur le président, madame la première ministre les savoirs techniques et sont essentiels à notre quotidien et à la réussite collective de notre pays et pourtant. Lors de sa présentation sur la réforme de la voie professionnelle, en septembre dernier, le président de la République a fait savoir qu'il entendait réduire le nombre d'heure dédié aux savoirs fondamentaux dans les lycées professionnels, cela n'est pas sérieux et pour preuve en 10 ans presque 1400 heures d'enseignement ont été supprimés, il reste aujourd'hui moins de 2 heures de français par semaine pour les bacs pro. Les heures d'enseignement fonde en réalité comme neige au soleil et on pousse de plus en plus tôt les jeunes dans les bras du marché du travail, au détriment de leur ouverture culturelle et de leur émancipation. Le manutentionnaire n'aurait pas besoin de trop d'éloquence pour la basse besogne, peu importe si cela le met en difficulté pour défendre ses droits ou changer sa carrière un ouvrier n'est pas fait pour devenir poète ou ou encore professeur et puis c'est bien connu, s'il veut s'insurger, il aura la grève ou l'abstention madame la première ministre les inégalités commencent dès la naissance, et avec cette réforme, vous les accentuer et même pire, vous renoncez à déjouer les pronostics, ce qui est pourtant au coeur du pacte républicain, alors on ne choisit pas toujours d'où l'on vient ni le métier que l'on exerce, mais une chose est sûre. L'école est faite pour donner à tous ses élèves une formation suffisamment qualifiante pour avoir le choix de partir et de pouvoir rebondir finalement cette réforme suit la même logique que votre réforme de l'assurance chômage, à savoir le travailleur de se soumettre au marché du travail, et son émancipation ça sera pour plus tard, ma question est assez simple : que comptez-vous faire pour sécuriser le parcours de vie de notre jeunesse en lycée professionnel, je vous remercie. Merci, cher collègue, et la parole et et maintenant à madame. Carole Granjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement de la formation professionnelle. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, cardons au fond, je crois que c'est la première fois qu'un président de la République porte aussi fort les valeurs de la voie professionnelle et le lycée professionnel au coeur de son engagement de campagne et de politique publique, au fond, tout doit être fait pour faire réussir la jeunesse et effectivement à l'heure qu'un tiers des lycéens passent par la voie professionnelle, nous devons accompagner l'évolution de la voie professionnelle pour qu'elle mette en réussite, l'ensemble de ces jeunes, vous l'avez dit, monsieur le sénateur, nous avons un défi, celui aussi de mettre en place partout sur tous nos territoires dans tous les lycées professionnels, le pacte républicain, celui de la promesse que nous devons leur faire qui est celui de les accompagner, bien sûr, en tant que citoyen pour qu'il puisse grandir par faire effectivement leur éducation et être demain, des citoyens éclairés qui s'engageront dans une voie professionnelle et qui doit les préparer aussi à une insertion professionnelle réussie, c'est tout le défi finalement de cette réforme professionnel, d'accompagner les savoirs fondamentaux que vous avez évoquées et monsieur le président de la République ainsi que madame la première ministre l'ont réaffirmé à plusieurs reprises, nous souhaitons préserver les savoirs fondamentaux, nous souhaitons accompagner ces élèves souvent plus fragiles sur ces savoirs fondamentaux qui sont essentiels à la citoyenneté, mais nous souhaitons également leur donner toutes les cartes pour qu'ils puissent s'insérer professionnellement et réussir l'insertion professionnelle qui aujourd'hui, je tiens à le rappeler, ne concerne qu'un élève sur 2 diplômé, 2 ans après l'obtention de leur diplôme et or poursuite d'études cette ce constat-là, il n'est évidemment pas le fait des enseignants qui sont évidemment pris dans un système, c'est de notre responsabilité collective que d'accompagner ce changement de système pour que nous donnions toutes les cartes aux enseignants pour qu'ils puissent accompagner les élèves et les mettre en situation de réussite effective. Madame la Ministre, bah, écoutez, je ne suis pas surpris de votre réponse, vous conforter même ce que je suis en train de dire en tout cas, tout ce que je vois c'est que ce gouvernement est un spécialiste des slogans notre école faisant la ensemble notre lycée professionnel faisons lancent ensemble, chiche, Madame la Ministre, il y a les chez moi en tout cas, il y a les faisait il les disent les Français vous demande tout simplement d'être les et de construire une vraie concertation pour sauver le lycée professionnel et pas l'inverse. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à notre collègue Philippe Dominati pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, il y a 4 ans. Avec Peugeot et Renault, la France disposait de 2 constructeurs automobiles de dimension mondiale ayant commun un actionnaire, l'État français qui était un actionnaire d'influence. Depuis la à trouver la voie de la croissance en acceptant d'être diluées dans le groupe Fiat, Chrysler groupe italo-américain et l'autre est passé de la première place mondiale à celle de plus petits constructeurs automobiles européens. Hier, le directeur général de Renault, a annoncé le 3ème volet de son plan pour cette entreprise, ce plan qui consiste à scinder en 2 cette entreprise et notamment avec de nouveaux partenaires l'un chinois, l'autre saoudien. Dans le même temps, le directeur général de Nissan en début de semaine dans la presse économique revendiqué la nécessité de rééquilibrer l'alliance avec Comme beaucoup de Français, je m'interroge et je m'étonne de ce qui semble être la passivité du gouvernement français vis-à-vis de ses partenaires dans la mesure où on ne comprend pas pourquoi 4 ans après la crise suscitée par l'incarcération de l'ancien directeur général de Renault d'ailleurs sans preuves probante jusqu'à ce jour, le gouvernement accepte éventuellement cette remise en cause, je voudrais savoir si il s'agit d'un rééquilibrage volontaire, ou si vous allez accepter le démantèlement de cette alliance.

Je pense que vous avez mis le doigt sur la réalité de l'industrie automobile actuel juste quelques chiffres pour commencer, capitalisation boursière de Renault 6 milliards d'euros. Capitalisation boursière de Stellantis 44 milliards d'euros Ford 53 milliards d'euros. Tesla 610 milliards d'euros. 2ème chiffre que je tiens à rappeler, Renault fait 60 % de ses ventes, c'est la grande différence par rapport à à Stellantis en Europe, l'Europe a décidé d'abandonner les véhicules thermiques, c'est pour ça que nous pensons que la stratégie de Luca de Méo est la bonne stratégie pour Renault, la bonne stratégie pour cette entreprise, c'est d'abord une stratégie qui lui permettent de retrouver de l'espace financier, c'est pour cela qu'elle sait pas les activités thermique des activités électriques et qu'elle a besoin d'un partenaire je partenaires le chinois Geely, qui je le rappelle, est déjà actionnaire majoritaire de Volvo, actionnaire de Lotus et actionnaire de Daimler en Allemagne, c'est donc un partenaire qui nous paraît un bon partenaire sur les activités électriques hein, Renault va pouvoir donc dégager des moyens financiers plus importants pour investir dans le moteur électrique, investir dans le véhicule électrique avec un projet de 1 1000000 de véhicules électriques, réalisée dans le nord de la France, Renault va donc être un des fers de lance de la réindustrialisation automobile de notre pays, il va développer également des batteries électriques pour que nous ayons l'indépendance totale sur la chaîne, il va développer pour la première fois un véhicule utilitaire léger électrique qui va répondre à toutes les questions que vous souvent posée sur les artisans, les commerçants, les BTP, les très petites entreprises qui ont besoin de véhicules utilitaires électriques légers, ils seront produits à Sandouville en France par Renault nous chou tout donc sa stratégie qui doit permettre la réindustrialisation automobile sur la base du véhicule électrique qui a été lancée par Luca de Méo et Renault s'agissant de l'Alliance nous continuons à penser que cette alliance entre Nissan et Renault et pertinente, nous soutenons donc les propositions qui sont aujourd'hui sur la table entre Renault et Nissan car de potentiel de synergies possibles qui renforceront encore Renaud. Merci monsieur le ministre, monsieur Dominati. Monsieur le Ministre, je suis pas très convaincu de votre réponse, parce que vous êtes de coeur et de Nissan, ce qu'il y a 2 gênant c'est con mais je tout sur l'électrique, d'un côté, le président de la République nous dit économiser mettais le chauffage à 19 degrés, éteignez la tour Eiffel, fait un certain nombre de choses à peine allocution présidentielle terminée, on offre 7000 euros pour acheter une voiture par exemple Nissan électrique dont on ne sait pas véritablement comment avec nos impôts, on pourra finalement continuer ce développement avec cette politique dans les jeux olympiques à Paris, dans ma ville, ou ceux de l'an 2024 il y aura que des voitures étrangères pour accueillir. Nos autres merci. La parole est désormais à notre collègue Jean-Michel Arnaud pour le groupe Union centriste. Monsieur le président, Mesdames et messieurs, le Ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse au Ministre de l'Économie et des Finances, l'explosion du coût de l'énergie, touche de plein fouet les particuliers, les entreprises mais également les collectivités territoriales, garant des services publics du quotidien, les communes en particulier ont subi nos stratosphériques des prix lors du renouvellement de leur contrat de fourniture d'énergie, il en est le même pour toutes les infrastructures publiques qui leur sont liés, à commencer par les remontées mécaniques, par exemple, pour mon département, les Hautes-Alpes pour leur venir en aide, ont été mis en place ou promis une succession de dispositif budgétaire et financier tout d'abord cet été dans le cas du projet de loi de finances rectificative a été instauré à notre initiative, le Sénat, un filet de sécurité en faveur des collectivités filet qui devait originalement concerné 22000 communes que nenni, seule une infime partie des collectivités en seront finalement bénéficiaire, par exemple, dans mon département, 5 communes sur 162 ensuite, nous avons eu l'introduction d'un bouclier énergétique dans le projet de loi de finances pour 2023 que nous allons bientôt examiner ici au Sénat, enfin madame Borne Première ministre a récemment annoncé la mise en place d'un amortisseur électricité nous attendons, là encore, la parution d'un décret pour savoir qui en bénéficiera, précisément et selon quelles conditions Monsieur le Ministre, tout ceci commence à ressembler à un véritable maquis nous avons du mal à nous y retrouver, alors imaginez également les maires des petites communes, comment vont s'articuler ces différents dispositifs toutes les collectivités seront-elles concernées par ces mesures de soutien et quand toucherons tels les premières Z, c'est essentiel pour le maintien des services équipements publics du quotidien qu'elles assument. Merci. Cher collègue, la parole à monsieur le Ministre. Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, vous me permettrez de répondre, puisque la partie collectivités territoriales a été plus intense dans votre question, que la partie économique qui s'adressait à Bruno Lemaire, d'abord pour articuler très rapidement hier et aujourd'hui, il y a la situation de l'année 2022, et il y a la situation de l'année 2023 sur 2022, les choses sont assez simples avec le bouclier, qui a été mis en place, qui concerne toutes les collectivités de moins de 10 salariés de moins de 2 millions d'euros de budget et pour celle-là. La règle 2022 sera la règle 2023 toutes les entités de moins de 10 salariés, c'est le bouclier, le sujet c'est au-dessus pour l'année en cours et le Sénat, il a pris toute sa part, le filet de sécurité qui a été votée cet été, permettaient de compenser le fait que, au delà d'un certain niveau de dépense énergétique, il n'y avait pas de dispositif spécifique pour les collectivités, à l'heure où nous parlons, vous savez que les collectivités peut faire la demande d'une avance et l'estimation sur le nombre de communes par département qui pourraient bénéficier du dispositif, vous avez l'air de le connaître, chez vous, je ne connais pas France entière pour 2023 bouclier pour les moins 10 amortisseurs pour celles qui sont à plus de 10 salariés pour faire très simple : quand vous additionnez la moitié de la facture qui est couverte par la reine et la part qui est libre, au delà de 180 euros. Du kW/h du mégawattheure nous nous retrouvons dans un dispositif de soutien qui prend la forme de 50 pour 100 du niveau de facture jusqu'à un plafond qui est située à 420 euros, ça c'est le dispositif. Daniel. Le caractère pas immédiatement accessible du calcul, explique que le décret étant encore à la minute où nous parlons, en cours de rédaction et vous mesdames et messieurs les sénateurs, vous allez dans quelques jours. Pouvoir prendre le filet de sécurité qui arrive de l'Assemblée, avec un aval. Qui a été donné par le gouvernement pour un dispositif qui est beaucoup plus puissant que celui qui a été validé pour l'année 2022 puisque c'est un milliard et demi d'euros. Que nous envisageons de consacrer au soutien des factures énergétiques de toutes les collectivités locales qui se retrouvent avec une diminution de leur capacité d'autofinancement trop importante pour qu'elle puisse supporter seuls la facture que le ministre, monsieur, il y a les marges d'amélioration et ne doutons pas que le dialogue permettra de simplifier le dispositif.

lorsque vous regardez le dispositif d'amortisseur électricité lorsque, par exemple, les stations de sports d'hiver des Hautes-Alpes se retrouvent à utiliser ce dispositif, elle se retrouve avec une capacité à assumer les charges énergétiques à hauteur de 20 % de leur chiffre d'affaires et donc ça signifie qu'elles sont en situation de risque vital à l'issue de la saison, elles sont en situation de faillite, de faillite, donc je crois qu'il est nécessaire dans le dialogue parlementaire de trouver des solutions, mais il faut trouver des solutions opérationnelles et des 1er décembre ce Monsieur le Ministre, je vous en conjure. Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la première ministre en août dernier lors du vote de la loi de finances rectificative pour 2022 le groupe Les Républicains a fait adopter un amendement il visait à mettre en place les premiers crédits permettant de lancer dès l'Automne suivant le chantier de la mise en oeuvre d'une carte Vitale biométrique permettant de s'assurer s'assurer de l'identité de son détenteur, l'avis du gouvernement était à l'époque un avis de sagesse et vous vous étiez engagé à prévoir d'autres crédits, crédits dans le PLFSS pff pardon 2023, l'enjeu est important. Un rapport conjoint de lier l'IGF et de l'IGAS a estimé que le nombre de titulaires d'une carte vitale excédé de plus de 7 millions le nombre de personnes résidant en France un rapport sénatorial quant à lui l'évaluait, en 2019 entre deux et plus de 5 millions et la directrice de la sécurité sociale en 2020, reconnaissait lors d'une audition au Parlement un surnombre de de 16 6 millions de cartes vitales quant au montant de la fraude sociale il entre 14 et 45 milliards d'euros par an, la fraude à la carte vitale ayant toute sa part dans cette dérive madame ce sujet de la fraude sociale mériterait que le gouvernement s'en saisisse vraiment or, que constate-t-on non seulement le gouvernement n'a rien fait pour aller dans ce sens mais, pire encore, aucun crédit n'est inscrit pour cette action au PLFSS 2023. Décidément, votre gouvernement a bien du mal à écouter le Parlement à prendre le chemin de la réforme et à se donner les moyens et d'économiser l'argent public. J'aurais donc 3 questions, ne pensez-vous pas madame la première ministre que la lutte contre la fraude sociale devrait être une priorité et que tous les moyens pour y contribuer, de votre être mise en oeuvre, pourquoi avez-vous refusé d'inscrire pour 2023 des crédits, donc d'engager enfin le programme de création des cartes vitales Pio biométrique et pour finir au-delà de votre réticence à agir se poser une question plus large ne pensez-vous pas que dans une démocratie, les décisions du départ du du Parlement, pardon, c'est-à-dire ce que prévoit la loi doit être respectée par le gouvernement. et. Ah Madame Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Monsieur le Président, Madame et messieurs les mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Claudine Thomas, vous l'avez dit, la lutte contre la fraude est un sujet essentiel à la fois pour des raisons éthiques et de soutenabilité de notre modèle de protection sociale, c'est bien parce que c'est un sujet essentiel que, dans ce PLFSS 2023, que nous avons commencé examiné au Sénat, mon collègue Gabriel Attal et moi-même portons des mesures fortes et ambitieuses à la fois pour prévenir, détecter et sanctionner les fraudes, conformément aux engagements qui ont été pris, lors du vote au Parlement en juillet dernier une mission IGAS IGF a été lancé en vue d'évaluer l'intérêt et les conditions de mise en oeuvre d'une carte Vitale biométrique cette mission permettra de recenser des travaux déjà conduits pour évaluer la fraude liée à l'usage des cartes et notamment son impact financier elle analysera ensuite les différentes solutions techniques et leur faisabilité et, le cas échéant, leur condition de mise en oeuvre dans le même temps, le gouvernement a lancé le chantier d'une carte vitale dématérialisée qui correspond davantage aux nouveaux usages, ainsi qu'aux attentes des professionnels de santé eux-mêmes une phase expérimentation a été entamée en 2019 auprès d'assurés et des professionnels de santé, la carte vitale dématérialisée est en cours dans 8 départements jusqu'à l'année jusqu'à la fin de l'année auprès des assurés volontaires en parallèle de cette étude sur la carte Vitale biométrique, le gouvernement entend aller au terme de cette expérimentation, qui d'ailleurs pour sécuriser l'identification de la personne contient de la biométrie cette carte vitale dématérialisée pourrait être généralisé à partir de 2023 en fonction de résultats de l'évaluation et des exigences de simplification auxquelles nous sommes très attachés, je vous remercie. merci madame la Ministre, la parole est maintenant à notre collègue Marie-Arlette Carlotti, pour le groupe socialiste. écologiste et républicain. Monsieur le président, Mesdames, messieurs les Ministres, chers collègues depuis 54 jours le sang coule en Iran, et c'est d'abord le sang des femmes en février 79, avant même l'instauration de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Khomeiny déjà que la liberté de la femme était un principal obstacle à son projet politique et depuis l'élection de l'ultraconservateur a ici, la situation s'est encore dégradée depuis 54 jours depuis la mort de Mahsa Amini, les manifestations se multiplient et la répression et de plus en plus brutal au fur et à mesure que le pouvoir se sent en danger une répression sans précédent samba sur le peuple iranien la politique ou la police ouvrent le feu sur les manifestants, il y a plus de 300 morts, 14000 arrestations, comme ces 2 journalistes qui sont aujourd'hui en prison, parce qu'elles ont dénoncé le Crime commis par la police des moeurs toutes celles qui brûlent leur voile qui arrachent leur carcan qui se coupe les cheveux risque aujourd'hui la peine de mort l'Iran balaie l'intégralité des droits humains et pourtant et pourtant depuis mai 2021, la République islamique d'Iran et membre de la commission de la condition des femmes des Nations-Unies, c'est surréaliste, en niant le droit des femmes et en menant une répression féroce contre son peuple, l'Iran, vous en conviendrez, à démontrer qu'il n'avait pas sa place au sein d'une commission qui promeut le droit des femmes et l'égalité des sexes, les premiers à réagir ont été les Canadiens, puis ce furent les États-Unis qui lance désormais une initiative pour provoquer le départ de l'Iran de cette instance, que dit la France, que dit la France Monsieur le Ministre, vous allez allez vous exigé l'exclusion de l'Iran de la commission des droits des femmes de l'ONU, le régime des mollahs n'a rien à y faire. Merci, cher collègue. Est à monsieur Olivier Becht Ministre. Délégué chargé du commerce extérieur. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Carlotti d'abord je voudrais excuser l'absence de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Catherine Colonna, oui, le mouvement de protestation des Iraniennes et des Iraniens se poursuit alors que le 26 octobre à marquer le 40ème jour suivant le décès de Mahsa Amini, ceux du ceux du cycle de deuil musulman chiite plusieurs cérémonies de deuil pour d'autres protestataires, décédé au début du mouvement, ont été organisées ces derniers jours c'est très nombreux et triste anniversaire suscite des rassemblements qui continue de faire résonner qui a le cri femme vie liberté face aux revendications légitimes de la jeunesse iranienne, les autorités maintiennent leur répression violente hé oui le bilan aujourd'hui et de plus de 300 morts comme vous le savez, nous avons réagi fermement à cette brutalité, notamment à travers un 1er paquet de sanctions européennes adoptée le 17 octobre visant les responsables de la répression, nous travaillons actuellement avec nos partenaires européens à un second paquet de sanctions visant d'autres responsables, il ne doit y avoir et il n'y aura aucune impunité à aucun niveau en fin de semaine dernière, nous avons également échanger avec nos partenaires du G7 au sein de l'évolution de la situation en Iran, nous partageons les mêmes préoccupations très fortes quant à la réponse brutale des autorités iraniennes aux aspirations légitimes de sa population, nous sommes donc tout ce clair si la répression se poursuit, c'est aussi les sanctions qui se poursuivront et la France agira à tous les niveaux, y compris au niveau de l'Organisation des Nations unies si nécessaire. Madame Carlotti. Merci, Monsieur le Ministre, je regrette, cette réponse timide, certes nous il y a certes des sanctions ont été prises par la France et par l'Union européenne, mais elles sont bien timides aujourd'hui et pendant ce temps là le régime continuent à tuer aujourd'hui la situation s'est aggravée, il y a urgence et c'est plus le moment de la simple compassion ça ne suffit pas, nous attendons de la France, qu'elle soit plus audible pour dénoncer la répression et pour défendre ceux qui se battent pour leur liberté, alors faisons les sortir de la commission. merci, cher collègue, la parole est maintenant à notre collègue Jérôme Bascher pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur Bruno Lemaire viser l'économie Monsieur le Ministre, nous nous connaissons depuis longtemps et nous partagions à une époque, la conviction commune qu'il fallait lutter contre les déficits, or depuis 5 ans et demi que vous être mise de l'économie, vous serez le ministre du record historique du déficit public du déficit budgétaire mais aussi, et voilà l'exploit du déficit commercial aujourd'hui, mes chers collègues, nous pouvons penser que. En fin d'année, nous serons à 200 milliards de déficit commercial 150 milliards sur 3 trimestres et il s'aggrave de trimestre en trimestre alors Monsieur le Ministre, comment analysez-vous votre échec et quelle à partir de cette bonne analyse quelles pistes avez-vous pour redresser la barre. Monsieur Bruno Lemaire. Je le sénateur Bachere si c'est un échec, c'est un échec collectif, puisque depuis 2000, la balance commerciale n'a jamais été excédentaire dans notre pays. Donc je suggère, je vous suggère de chercher plutôt ensemble des solutions plutôt que d'accabler tous les bancs de cette assemblée, gauche et droite confondues, la réalité c'est que aujourd'hui, l'excédent commercial dont j'ai déjà dit à plusieurs reprises que nous devions faire une des grandes batailles économiques de la prochaine décennie, c'est d'abord dû à l'augmentation de la facture énergétique et à notre dépendance énergétique sur les 16 milliards d'euros de déficit commercial supplémentaire que nous venons d'enregistrer les 2 tiers sont liés à la facture énergétique, je cherche pas, je ne cherche pas des subterfuges, je dis : quelles sont les réalités aujourd'hui des chiffres, la 2ème raison, vous la connaissez aussi bien que moi, je connais votre attachement à ce sujet, c'est la désindustrialisation massive de la France depuis 3 décennies, il n'y aura pas d'excédent de la balance commerciale française 100 réindustrialisation massive rapide volontariste d'autres pays, quelle est la seule majorité qui depuis 20 ans. à recréer des emplois industriels dans notre pays, c'est la nôtre. Quelle est la seule majorité qui peut dire que nous avons ouvert plus d'usine l'année dernière, que nous avons fermé, c'est la nôtre, quelle est la seule majorité qui a eu le courage de baisser les impôts de production de 10 milliards d'euros et qui va à nouveau les baisser pour les années. Qui viennent, c'est la nôtre, donc si vous voulez réduire le déficit de la balance. Thomas à l'extérieur, voter avec nous la nouvelle baisse des impôts de production soutenez l'industrie soutenez la réindustrialisation du pays, et là nous aurons enfin une balance commerciale extérieure positif. car nous venons exactement de vous expliquer ce qu'il fallait faire, écoutez bien la suite des questions du groupe, les républicains tout à l'heure, on vous a expliqué ce que c'était pour le déficit public avec Christine Lavarde sur la réindustrialisation de notre industrie de santé sur la réindustrialisation notre automobile la semaine dernière ou il y a 15 jours plus exactement Laurent Duplomb vous rappelait sur l'agriculture, oui, nous vous faisons des propositions mais vous les entendez pas par dogme, nous proposons d'abord d'énormes et après on dit à notre industrie, vous n'avez plus qu'à vous adapter, hé bien non, on donne des caps, clairs, Monsieur le Ministre on indique ce qu'on veut faire au pays, vous nous dites, faut que ça soit la prochaine décennie, mais vous avez raté la décennie dernière vous avez raté la décennie dernière ce pays n'est aujourd'hui pas souverain et en ce jour anniversaire de la mort du général, la souveraineté aurait mérité d'être vraiment mise à l'honneur, vous l'avez la souveraineté dans les titres, vous ne l'avez pas dans les faits. La parole est maintenant à d'autres collègues, Claude Kern, pour le groupe Union centriste. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, l'installation illicite des gens du voyage est une problématique qui n'est pas nouvelle, loin de là, cela fait 20 ans qu'elle revient régulièrement sur le tapis, sans toutefois constaté de changement effectif la loi Besson n'est ni efficace ni et des situations difficiles en découle pour leur pour nos communes, j'ai encore eu connaissance de plusieurs cas en Alsace et je ne et je sais que mes collègues élus dans d'autres départements sont confrontés aux mêmes problématiques certes certaines intercommunalités encore des difficultés pour développer des aires de grand passage nécessaire au respect de la loi, mais qu'en est-il des territoires qui sont en conformité avec le schéma départemental et qui subissent régulièrement des installations illicites ces communautés, refusant de s'installer sur les aires dédiées, les élus se retrouve alors démuni face à des communautés qui ont une parfaite connaissance des procédures leur permettant de faire échec, un arrêté préfectoral de mise en demeure, en saisissant et médiatiquement, le juge administratif d'un référé suspensif un trou dans la raquette qui leur permet de prolonger leur présence sur le site qu'ils ont investi en toute illégalité, c'est cette suspension qui pose problème : que compte faire le gouvernement pour faire respecter la loi sans pour autant oublier la question de l'après, qui est tout aussi importante, car trop souvent les terrains occupés sont laissés dans un mauvais état avec des dégâts conséquents, monsieur le Ministre, dans quel la délai allez-vous déposer un projet de loi qui mette définitivement un terme à ces installations illicites et protège les élus. La parole est à monsieur. Que Gérald Darmanin Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. je constate que les lois Besson hein hé bé sont de sont difficilement applicables et et en effet je crois que l'autorité républicaine et plusieurs fois bafoué les accueille, mis en place par les élus locaux, souvent ravagée et évidemment pour nos citoyens, des décisions administratives ou d'édition de justice peu compréhensible et qu'à ce titre, je veux évidemment faire le constat avec vous que nous devons améliorer le texte de loi, vous m'accorderez que les préfets de la République applique la loi telle qu'elle est aujourd'hui rédigé, faut-il que ce soit une proposition de loi après tout la haute assemblée, comme l'Assemblée nationale pourrait tout à fait le proposer, faut-il que ce soit un texte du gouvernement peut être un texte ensemble si vous le permettez, monsieur le sénateur pour pouvoir à la fois évidemment accueillir les gens du voyage qui ont évidemment le droit de vivre comme il le souhaite, sur le territoire de la République, bien évidemment en conformité avec la bienséance républicaine et le respect, évidemment des choses publiques ainsi que la propriété privée de nos concitoyens, pour avoir été maire d'une commune qui n'avait pas d'aire d'accueil des gens du voyage, je sais à quel point il est difficile pour la mairie de pouvoir la mettre en place, mais je veux rappeler d'abord que la loi Besson de doit répondre pour l'ensemble des élus de la République aux schémas départementaux et je ne peux malheureusement que constater qu'un certain nombre de conseils départementaux n'ont pas mis en place en place encore leur schéma départemental ou ont pas demandé la révision de celui-ci, monsieur le sénateur, c'est lorsque les personnes s'installent sur des terrains privés ou sur un terrain public ou une partie d'intérêt public ou le détenteur de la propriété ne souhaite pas déposer plainte, soit pour des raisons volontaires, soit parce qu'on ne connaît pas le propriétaire de ce terrain voilà notamment un vide juridique auquel il faudra tous répondre pour que les préfets puissent appliquer la force publique, lorsqu'ils ont soit en flagrance soit par décision de justice, les moyens de le faire et ils le font à chaque fois que vous vous saisissez. Merci monsieur Kern. et d'autant plus qu'elles ont souvent lieu à proximité d'habitations privées, un dernier mot concernant peut être également Lille l'installation illégale de cirque qui s'installe malgré l'interdiction formelle qui leur est notifiée préalablement sur ce point également, les élus locaux sont en attente d'une réponse rapide et efficiente merci. Merci, chers collègues, nous en avons terminé pour aujourd'hui, je vous rappelle que les prochaines questions d'actualité au gouvernement auront lieu le mercredi 16 novembre 2022 je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 16 pour la suite du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, la séance est suspendue.

Chers collègues, la séance est reprise bonjour monsieur le Ministre, monsieur le Ministre, Madame la Ministre, mes chers collègues, je suis particulièrement heureux de saluer la présence dans la tribune d'honneur du Sénat de Monsieur Félix Ouya, vice-président de la République d'El Salvador il est accompagné par notre collègue Nadège avait vice-présidente du groupe d'amitié France-Mexique, pays d'Amérique centrale, en visite de travail à Paris dans le cadre d'une tournée en Europe et en Afrique, il a rencontré cet après-midi, plusieurs sénateurs, membres du groupe d'amitié, la présence de monsieur où il aura au sein de notre assemblée témoigne de l'attachement de son pays à la France et à nos valeurs communes, mes chers collègues, en notre nom à tous, permettez-moi de saluer monsieur ou Doha infructueux séjour et la plus cordiale bienvenue.

bien, cher collègue, la parole est à ma Madame Véronique Guillotin pour des mises au point au sujet d'un vote. Oui, monsieur le président, lors du scrutin numéro 35 sur les amendements identiques 582 rectifié et 1040 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l'article 8 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 Guilaine Pentel souhaitaient voter contre, par ailleurs, lors du scrutin numéro 36 portant sur la 3ème partie du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 Stéphane Artano souhaité s'abstenir et Jean-Pierre Corbisez, souhaité voter contre, merci. Oui, merci Monsieur le Président, je souhaite à mon tour, faire une mise au point suivante sur le scrutin public numéro 29 mes collègues Else Joseph et Jean-Pierre Vogel souhaitaient voter contre. merci, cher collègue, acte et donné de vos mise au point, elles seront publiés au Journal officiel et figurant dans l'analyse politique du scrutin concernés, chers collègues, en application du 5ème alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique et de la loi ordinaire du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a émis lors de sa réunion du mardi 8 novembre 2022, un avis favorable par 20 18 voix pour et 8 voix contre à la nomination de Monsieur Jean Castex, aux fonctions de président directeur général de la Régie autonome des transports parisiens. J'informe également le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi est parvenu à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour. Appelle la suite de la discussion du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, en application de l'article de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour 2023 dans la discussion des articles que nous sommes parvenus à l'article 16. Et nous entamons la discussion de l'article 16 avec. La discussion de 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune le 1er le 674 et présenté par Madame Gruny. Oui, merci Monsieur le Président, cet amendement supprime la prolongation jusqu'au 31 décembre 2023 du dispositif d'indemnisation dérogatoire des arrêts de travail pour certains publics dans le cadre de la crise sanitaire si le dispositif d'indemnisation dérogatoire des arrêts de travail pour certains publics s'est avéré légitime et nécessaire lors des temps forts de l'épidémie sa prolongation paraît injustifiée d'autant plus que l'acceptabilité du dispositif à la fois pour les chefs d'entreprises et pour les salariés non concernés s'érode le présent amendement propose donc de limiter ce dispositif au 31 décembre 2022. Merci madame la présidente, et puis le 2ème amendement le 286 présenté par Monsieur Milhaud. Oui, mais merci monsieur le président, les examens de biologie médicale délocalisé sur des examens de biologie médicale dans la phase analytique et réalisé à proximité du patient en dehors des locaux du laboratoire de biologie médicale : le médecin est responsable de la lecture du résultat, le biologiste demeure évidemment, responsable de la validation a posteriori de celui-ci, la crise Covid 19 a mis en lumière l'utilité et la nécessité d'un développement de la biologie délocaliser l'ouverture de la pratique des tests antigéniques Covid 19 au pharmacien a permis de massifier le dépistage et faire reculer épidémie dans le même esprit que l'article 16 cet amendement donc vise à étendre cette politique de dépistage, la médecine de ville, pour simplifier, et encore davantage le dépistage de la Covid 19. Merci, avis de la commission madame la rapporteure. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, donc, avec certains articles 16 nos attaquants là la 4ème partie du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale donc sa partie dépenses et notamment la partie prévention de ce texte alors sur l'amendement 674 Madame Bruni et et de nos collègues, j'entends évidemment les les arguments de de la présidente grenier, surtout au regard du coût de la mesure pour rappel, le coût de la prise en charge du délai de carence est estimé par le gouvernement à plus de 800 millions d'euros sur l'année, je veux bien, je parle bien des consignes sanitaires actuelles, la suppression de cette prise en charge par l'assurance maladie n'est pas souhaitable aujourd'hui une personne contaminée par le Covid 19 doit s'isoler pour une durée de 5 à 10 jours en fonction de son statut vaccinal si elle n'est pas en mesure de travailler à distance ou si son état le justifie, elle doit bénéficier d'un arrêt de travail. Or, la suppression de cette prise en charge ferait courir un risque de perte de revenus pendant la période de carence pour de nombreux salariés jusqu'alors que des personnes en situation précaire soient ainsi incités à ne pas déclarer leur contamination et à aller travailler en état contagieux, c'est donc un risque pour elle et pour les personnes qu'elles côtoient dans le Rhône environnements professionnels, c'est pour cela qu'en l'état des prescriptions d'isolement, l'avis est défavorable, en revanche, j'aurais peut-être à l'occasion de cet amendement de question Monsieur le Ministre, la première alors que beaucoup de gens renoncent à se faire dépister quand ils présentent des symptômes et que le port du masque n'est plus obligatoire, le gouvernement a-t-il encore réellement une politique de freinage de la propagation du virus et une seconde question : la prise en charge de l'arrêt de travail se fait sous réserve que le salarié ne puisse travailler à distance, y a-t-il des contrôles sur ce point, concernant l'amendement numéro 286 de notre collègue Alain Milon, cet amendement, s'attachant croit reconnaître le rôle de la biologie dans les moyens de dépistage, effectivement, vous l'avez rappelé, c'est une bonne chose mais ce pas tellement l'objet de de de l'article sur le fond, cet amendement est satisfait des professionnels de ville peuvent bien déclarer dans DEP, les résultats des tests qu'ils feraient dans leur cabinet, donc à défaut d'un retrait, c'est un avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre, sur ces deux amendements. Monsieur le président, Mesdames et messieurs, madame la rapporteure concernant la la suppression de certains arrêts de travail dérogatoires à la Covid, je tiens bien sûr, a précisé que ces ces arrêts de travail et ces prolongations ne concerne que les personnes positives à la Covid, donc les personnes malades et ne concerne plus, bien sûr, puisqu'il n'a pas été reconduit les cas contacts en ce qui concerne les personnes malades, ça s'inscrit bien sûr dans un objectif de protection individuelle mais surtout dans un objectif de protection de santé publique en protégeant les travailleurs, je dois avoir rappeler ici que, encore aujourd'hui, il y a un mort toutes les 10 minutes, lié à la l'infection par COVID. Par rapport à la date qui est proposé, je tiens à rappeler également que l'article 16 donne la possibilité d'interrompre la prise en charge de ces arrêts de travail dérogatoires par simple décret avant le 31 décembre 2 trois ce qui nous permet de nous adapter à l'évolution de cette épidémie épidémie pour laquelle les scientifiques nous indique quand même un rebond et une nouvelle vague cet hiver, l'avis est donc défavorable pour répondre aux questions de de la rapporteure, en ce qui concerne la politique de freinage oui bien sûr madame la rapporteure, nous avons une politique de freinage qui se base sur la vaccination et sur les gestes barrières le rappel des gestes barrières et pour ma part, quotidien, même si force est de constater qu'ils sont assez peu respectées, en particulier dans les transports en commun, c'est dommage parce que ces gestes barrières protège non seulement de la Covid, mais également de la grippe également nos enfants des infections par VRS, donc il y a lieu de vraiment insister quant à la vaccination, je reconnais que la campagne d'Automne démarre doucement, puisque seuls 10 personnes des pièces de des personnes cibles sont actuellement vaccinés, il y a lieu de réactiver cette campagne, même avec les les moyens de communication que nous avons actuellement, qui sont les mêmes que les autres campagnes, on voit qu'ils sont moins efficaces, donc nous sommes en train de changer un petit peu ses ses modes de de communication le travail distance il y a des contrôles, pas plus que les contrôles habituels malheureusement concernant les arrêts de travail. Monsieur le sénateur Millon en ce qui concerne la participation de la médecine de ville au dépistage de la Covid, les arrêts de travail sont conditionnés à la réalisation d'un examen de dépistage qui est enregistré dans si DEP les médecins comme les biologistes comme les pharmaciens peuvent enregistrer enregistre déjà des tests dans si DEP, dès lors, je considère que votre amendement est est satisfait donc propose un rejet. Bien les amendements sont maintenus ou retiré Madame Gruny. Je je vais le le retirer mais en revanche, je voudrais quand même relevé une une certaine incohérence parce qu'il me semble que dans le projet de loi de financement, vous avez mis peu de moyens finalement pour une éventuelle reprise de de la Covid, je suppose que vous pensez que nous allons pas avoir beaucoup en fait de malades de la Covid et donc je trouvais tout à fait judicieux d'enlever cette mesure. Merci monsieur Milon, on a un petit bruit là on sait pas trop vous le retirer, OK, OK, on va monsieur le Ministre allez-y, allez-y. de côté pour un milliard porteront un milliard d'euros, a été mis de côté en prévision pour pour 2023, s'il y a bien une chose que nous avons tous appris depuis le début de cette crise, c'est d'être prudent et et de ne pas savoir du tout comment elle va évoluer, on on se permet comme je disais je disais dans cet article, d'interrompre par décret, mais on garde cette possibilité, on verra au fur et à mesure de suivi de l'épidémie et je reste bien sûr à la disposition du Sénat pour vous apporter le suivi régulier de cette épidémie Covid. donc les amendements étant retirés, nous allons passer au vote de l'article 16 qui est pour l'article 16. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté. Ensuite, l'amendement 780. Madame Gréaume. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, alors que l'assurance maladie, l'Unocam et les syndicats de médecins libéraux démarre aujourd'hui les négociations sur la convention médicale notre amendement vise à pointer les échecs de la présence d'un précédent provençaux de 2016 en matière de régulation des dépassements d'honoraires, l'objectif était de doubler le nombre de médecins qui s'engagent à nous limiter les dépassements d'honoraires, mais l'objectif n'a pas été atteint le nombre de spécialistes qui facturent des dépassements d'honoraires est passé de 45 % en 2016 à cinquante fin 2020 en 2021, nouveau record a été battu, avec près de 3 milliards sacs d'euro de dépassement d'honoraires, la prochaine convention médicale pour la période 2023 2028 devra prendre de véritables mesures d'encadrement et de plus des 2 plafonnement pardon de ses déplacements, ceci dans une période de difficultés d'accès aux soins, entraînant une augmentation du reste à charge subit principalement par nos concitoyens les plus précaires et occasionne par la même occasion pour certains ah renoncement aux soins, les jeunes professionnels ne sanctionne quasiment pas les médecins qui pratiquent ces dépassements d'honoraires excessifs face à cette impunité qui renforce les inégalités sociales de santé, nous proposons de rétablir une amende pour les professionnels qui réalisent des dépassements d'honoraires excessifs merci. Merci madame la rapporteure. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avons ce débat chaque année, la position de la commission n'a, n'a pas changé sur ce point l'avis sera défavorable, je rappellerai simplement 3 points d'une part, le respect du tact et de la mesure, la grande majorité des médecins même en secteur du long bien à l'esprit, d'autre part, ce n'est pas parce qu'il y a pas d'amende prévue dans le code de la santé publique, sur ce point que le respect du tact et de la mesure ne sont pas inscrits au sein du code de déontologie des médecins et donc bien suivie par le Conseil de l'Ordre des médecins, enfin, au delà des moyens coercitifs auprès du Conseil de l'Ordre je crois aux effets de l'action de l'assurance maladie qui joue notamment sur des leviers incitatifs, c'est l'objet par exemple des contrats Optam visant à maîtriser les dépassements d'honoraires et assurer un accès aux soins qui ne soit pas freiné pour des motifs économiques voilà donc c'est un avis défavorable sur cet amendement. Monsieur le Ministre. Monsieur le président, messieurs les sénateurs Madame la sénateur Cohen : avis défavorable également, je tiens à rappeler 2 choses sur ce sujet important, tout d'abord que les les assurés les plus fragiles bénéficient de la complémentaire santé solidaire qui les prémunit d'ores et déjà de tout reste à charge sur les consultations médicales parce que les professionnels de santé ne peuvent leur reposer dépassement d'honoraires, hormis dans des cas d'exigences particulières de leur part, visite injustifiée par exemple, d'autre part, les dispositifs de sanctions financières existent déjà pour ces professionnels qui ont des des pratiques tarifs hier qu'on pourrait qualifier d'excessives, ils encourent déjà soit une pénalité financière soit une interdiction temporaire du droit de pratiquer les dépassements, la CNAM à ce titre, a lancé fin 2021, une nouvelle campagne de régulation de ces pratiques tarifaires incluant environ 200 médecins donc défavorable comme j'ai. Il y a un double avis défavorable madame Groux. Et intervenir sur le sujet, parce qu'on parle toujours des plus précaires et ce qu'ils ont les moyens de de payer les dépassements, il y a quand même tous ces smicards aujourd'hui qui ne se soignent plus, parce que ses déplacements, ils savent pas ils savent pas les payer, donc je vous le rappelle, quand même, il faut quand même prendre en considération qu'aujourd'hui les hôpitaux publics ne peuvent plus répondre et les salariés sont obligés aussi d'aller dans le privé parce qu'ils sont orientés par les hôpitaux publics aujourd'hui et ça c'est une réalité, donc je rappelle quand même que les smicards aujourd'hui hé ben il y en a beaucoup qui renoncent à se soigner et c'est dommageable.

il y a effectivement des notions de tact et de mesures qu'il faut bien évidemment garder et on voilà, tout n'est pas possible pour autant moi j'aimerais juste rajouter quelque chose, je veux dire on est aujourd'hui sur un paiement ou l'acte intellectuel en matière de santé n'est pas rémunéré quand on a une consultation d'ophtalmo d'ORL, voilà c'est certains praticiens sont contraints, je dirais comme ça pour d'avoir un exercice en secteur 2 pour pouvoir, hein, un une rémunération correcte ou alors ils sont aussi contraints à faire des actes physiques des échos, enfin des actes des gestes chirurgicaux, des gestes, des gestes micro-invasif pour pouvoir augmenter effectivement les rémunérations alors je crois qu'on est dans un problème beaucoup plus globale, je crois, de de majoration de Dax et de à leur juste mesure des actes dits intellectuels pour les médecines de consultation. Monsieur Jomier. Merci monsieur le président, je crois qu'il faut qu'on accepte quand même le constat que c'est effectivement un échec, la régulation des dépassements d'honoraires,

mais c'est maintenant généraliser c'est-à-dire que les gens quand ils se font opérer maintenant il y a le dépassement du chirurgien et c'est plus pour des opérations standard 100 ou 200 euros en plus c'est plutôt 500000 euros la moyenne et puis il y a l'anesthésiste aussi maintenant, ça c'est nouveau, les les dépassements d'honoraires se cumulent les uns et les autres et des patients qui ont une couverture, y compris avec une complémentaire maintenant que quand ils doivent avoir une intervention chirurgicale sur la hanche et cetera, et cetera et bah ça leur coûte mille euros c'est ça la réalité actuelle des dépassements d'honoraires, et moi j'invite vraiment Monsieur le ministre, à ce que dans la négociation, la nouvelle convention vos instructions en la matière soit très clair : la convention de 2016 est un échec, à cet égard la prochaine doit adopter des mesures réelles parce que c'est un problème d'accès aux soins pour nos compatriotes. Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le le président moi je voudrais monsieur le Ministre, attirer votre attention, il vient d'y avoir une publication de la de la carte de l'UFC que choisir, le 8 novembre 2022, je vais reprendre un certain nombre de chiffre qu'il donne, il souligne, comme l'a dit ma collègue Michelle Gréaume que la la fracture n'est pas seulement géographique pour avoir accès à un médecin, mais qu'elle est aussi financière cette association alerte sur les dépassements de leur d'honoraires pour la plupart des spécialistes, il devient de plus en plus difficile de trouver des médecins qui respectent les tarifs de la Sécurité sociale ainsi près de 7 patiente sur 10 réside en désert médical en termes d'accès au gynécologue en secteur 1, c'est-à-dire sans dépassements d'honoraires, à moins de 45 minutes de chez elle et près d'un enfant sur 2 résidents désert médical pour ce qui est de l'accès au pédiatre au tarif de la Sécurité sociale, on est toujours sur le secteur, hein, une situation d'autant plus alarmante, lorsque l'on sait que le frein financier représente 29 % du renoncement aux soins des patientes et des patients, si je prends par exemple un département comme le Val-de-Marne, Val de Marne Île-de-France Île-de-France le 1er désert médical, hein, donc voilà, et bien sûr un département comme comme

qui n'ont pas d'ophtalmo qui sont en secteur hein, donc vous voyez, je veux dire que effectivement vous nous donner des éléments, mais nous, dans ce débat du PLFSS depuis lundi, nous donnons des arguments qui montre que ça ne fonctionne pas et vous vous entêtez en disant mais si, mais si ça va marcher, je suis volontaire, j'arrive, et essayer un peu de bouger ce PLFSS qui est insuffisant et qui ne va pas dans le bon sens. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, donc moi je ne voterai pas cet amendement mais je peux quand même confirmer que effectivement parfois notamment rurales pour des gens qui ont des petites retraites, alors je ne critique pas du tout les médecins qui font dépassement d'honoraires, quelques fois, comme l'a dit Véronique bah c'est obligé, notamment pour les ophtalmos qui doivent installer des appareils extrêmement cher mais il est évident que certaines personnes ont des difficultés lorsqu'ils se rendent chez certains médecins, on leur dit : bon, ben il faut payer un dépassement d'honoraire et ils ont des difficultés, donc c'est pas du tout, c'est assez fréquent, donc je voulais le confirmer.

on a mis sur pied des contrats solidaires et des contrats qui limité pour certains, la prise en charge de tous ces dépassements d'honoraires et et la conséquence, c'est que, effectivement, maintenant, ça saute aux yeux qu'il a des déplacements qui sont particulièrement importants et ça traduit quoi, ben c'est encore la gestion de la pénurie, Monsieur le Ministre, comme il y a pas suffisamment effectivement le médecin en secteur 1, ben il a sur un secteur de et puis derrière, ben il y a une telle fille de table ronde que effectivement, voilà, il y a une sélection après qui s'opère par les jeux du pouvoir d'achat des des des patients en conséquence plus que jamais, ça traduit bien Monsieur le Ministre, qu'il faut revoir entièrement le dispositif : une loi de santé qui correspond aux préoccupations de nos concitoyens et au financement qu'on veut bien y met en face. Monsieur le Ministre. monsieur le président, Mesdames et messieurs des des sénateurs quelques quelques éléments je je retiens bien sûr la sous-évaluation de la tu intellectuel qui est au au centre des au centre des préoccupations et et des discussions au sein des discussions conventionnelles qui démarre tout comme la problématique des dépassements excessifs, dans ma feuille de route et dans mes engagements, il y a la lutte quand toutes les inégalités d'accès à la santé, dont les inégalités financières également, cependant, pour être vraiment complet dans la discussion et si parlait de de cas particuliers qui sont toujours bien entendu dramatique ramené quelques quelques chiffres, le reste à charge globale des patients n'a pas évolué en France depuis 5 ans, alors certes, il n'a pas diminué mais il n'a pas augmenté, il se situe à 7 % en moyenne et correspond au plus bas reste à charge pour les patients de toute l'Europe, on peut même constater que sur la médecine de ville, ce reste à charge a diminué entre 2000 19 et 2020, c'est certainement insuffisant, mais en tout cas c'est ce sont des éléments importants par ailleurs 97 % de nos concitoyens, grâce à la simplification de de l'obtention de la complémentaire santé solidaire et puis l'ensemble des complémentaires ont maintenant une complémentaire santé compenser, malheureusement ce ce ce dépassement d'honoraire, même si cela pose encore des questions et je vous rejoins sur la nécessité de regarder ce sujet de très près, dans le cadre de la convention. Bien, merci, donc nous allons passer au vote sur cet amendement avec nos avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté. Amendement suivant le 827 Madame Cohen. et qui avait suscité beaucoup de colère, une forte mobilisation des psychologues si nous partageons le constat d'une augmentation des troubles anxieux et dépressifs, notamment depuis la crise sanitaire, nous ne partagions pas et nous ne partageons toujours pas la réponse apportée par cet article, d'où notre demande de suppression de cet article, ce que nous avions d'ailleurs été les seuls à demander l'année dernière, non désaccord portait et porte toujours sur 3 points qui nous sommes majeurs : premièrement, le nom de prévu de séance dans ce forfait psy en l'occurrence, 8 séances maximum qui peut penser qu'un nombre prédéterminé de consultation, lorsque l'on parle de troubles anxiogène dépressif et autres serait le même pour chaque patient est une bonne idée, comment ignorer que la fixation d'un nombre préalables de séance est totalement inopérante et contraire à l'esprit d'une psychothérapie qui doit être individualisée en fonction du patient, deuxièmement, le tarif des consultations quarante euros la première et 30 euros pour les 7 suivante, ce qui est totalement insuffisant, troisièmement, et sans doute le point le plus grave, l'accès à ces séances est conditionné à une prescription médicale, alors que les psychologues ne sont pas des paramédicaux et que, jusqu'à l'an dernier, aucun assujettissement à un médecin ne leur a jamais été demandée pour nous, il s'agit d'un recul et d'une dévalorisation de cette profession qui est déjà très mal considéré, au regard du nombre d'années d'études, tout ceci est grave et s'inscrit, qui plus est dans une certaine offensive pour que la santé mentale soit davantage formaté et uniforme, comme si elle de elle devenait elle devait devenir une science exacte, niant la relation soignant soignant niant la complexité du psychisme humain où tout devrait rentrer dans des dispositifs standardisé, sous couvert de se préoccuper de la santé mentale de nos concitoyens et concitoyennes, cette disposition va produire à terme des effets pervers et mettre à mal la spécificité d'une profession, il est encore temps de revenir dessus en adoptant notre amendement de d'abrogation, je vous remercie. j'ai lu l'objet avec attention, ma chère collègue de de votre amendement ou le forfait psy serait considérée comme étant inadéquate inadaptée méprisant et et maltraitant je trouve les mots forts et je souhaiterais qu'on qu'on garde un petit peu de de mesures sur ce sur et de tact et de tact et en gardant toujours le sourire, je pense que ce dispositif, même s'il n'est pas parfait c'est un complément utile à l'offre de soins en santé mentale, soyons honnêtes, la prise en charge de la santé mentale n'est pas bonne et nous le savons tous le recours est insuffisant pour une série de raisons notamment parfois une autocensure des patients alors que les problèmes de santé mentale sont souvent stigmatisés parallèlement l'offre disponible en psychiatrie est très insuffisante, cela est établie par de nombreux rapports et encore plus préoccupant en pédopsychiatrie, en outre, les chiffres concernant la consommation de psychotropes ne cesse de progresser, signe d'un problème de santé publique, la commission a validé ce dispositif l'an dernier que le rapport de nos collègues Jean Jean-Sol et victoire Jasmin encourageait également avec ce dispositif, il ne s'agit pas de remplacer la psychiatrie : il ne s'agit pas d'une offre au rabais, il est faux de suggérer cela, il s'agit d'un dispositif d'accompagnement qui a vocation à apporter un soutien pour des patients ne ne il s'entend pas nécessairement de prise en charge psychiatrique mais aussi à servir de 1er recours pour d'autres, et ainsi à s'insérer dans une prise en charge, j'insiste sur ce dernier point, puisque le dispositif préserve un adressage médical et un lien entre médecins et psychologues, ce qui était un dénoncé dans votre intervention, mais néanmoins ce qui est la contrepartie du conventionnement avec l'assurance maladie et donc la prise en charge du prix de ces consultations, ce dispositif répond donc à un besoin, nous avions demandé à l'été, des chiffres à la CNAM, qui nous avait indiqué que 3300 patients avaient été pris en charge les 8 premières semaines le gouvernement a sans doute des chiffres actualisés sur le recours pour toutes ces raisons, vous l'avez compris l'avis est défavorable. Monsieur le Ministre. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs Madame la la sénatrice Cohen. Effectivement, la santé mentale est un enjeu majeur de santé publique une priorité pour le gouvernement, comme en témoignent les assises de la psychiatrie et de la santé mentale de l'année dernière, qui ont donné lieu à la création

pour lesquels nous nous aurons sûrement l'occasion de revenir les maisons des adolescents qui se développe de plus en plus et qui apporte vraiment une réponse adaptée à à ces problèmes des enfants. Le dispositif tels que vous le décrivez est accessible à toute la population à partir de trois ans la prise en charge la mise en oeuvre ont été définis après un travail de concertation avec l'ensemble des acteurs normalement, normalement essentiellement pardon les représentants des psychologues cliniciens comme ça l'a été dit par la rapporteure, il répond un fort besoin de la population des chiffres récents, plus de 39000 patients ont pu bénéficier d'une prise en charge de psychologique, médicale depuis le lancement de ce dispositif, 39000 patients. Ce dispositif fera l'objet, et cela est prévu, d'une évaluation d'ici 2025, dans l'optique de poursuivre l'intégration des psychologues cliniciens dans le parcours de santé mentale, il semble donc pertinent et judicieux d'attente des résultats de cette évaluation et d'envisager à ce moment-là, soit une prolongation soit une modification du dispositif pour toutes ces raisons je suis défavorable à votre amendement. Il y a un double avis défavorable monsieur Bueno. Oui, merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre, moi je ne voterai pas cet amendement, je sens bien parfois que ce dispositif, qui relève de l'innovation est imparfait, mais souvent, lorsqu'un dispositif à Paris, il est imparfait, mais en même temps, comment ne pas voir qu'il répond à une demande et que, au lendemain du Covid, hein, d'ailleurs, de la crise du Covid l'état mental d'un certain nombre de personnes étaient et qu'il fallait cette innovation bien évidemment après l'évaluation, je pense qu'il faudra faire un pas supplémentaire, mais jeter le bébé avec l'eau du bain, alors même que ça permet à un certain nombre de personnes hé bien de, de, de trouver des des réponses qu'elle n'aurait pas le moyen de de trouver sans ce dispositif, me paraît tout à fait excessif, raison pour laquelle je ne voterai pas cet amendement, je vous remercie. Madame Cohen. Je suis pas surprise de l'intervention de mon collègue qui va pas voter notre amendement, ni d'ailleurs de de de l'explication de notre rapporteur, moi je suis toujours extrêmement étonné compte on apporte des éléments que ces éléments reposent sur des revendications extrêmement fortes de l'ensemble de la profession, pas de quelques-uns ou de quelques-unes et qu'on nous dise : mais non, mais vous allez voir, il faut attendre. je, je, j'avoue que je ne comprends pas, je ne comprends pas, alors évidemment, Monsieur le Ministre, vous nous dites : on va faire une évaluation. Bon. C'est toujours bien de moi, j'aimerais bien que le gouvernement évalue tout ce qu'il met en place, ce serait déjà pas mal, ce qui ne fait pas mais en attendant. Quand on va dans les services hospitaliers quand on va dans les CMP ou dans les CMPP comme c'est mon cas, et comme c'est le cas de l'ensemble de mes collègues du groupe CRCE et sans doute de beaucoup de mes collègues des autres formations politiques qu'est-ce qu'on remarque, on remarque qu'il y a un manque terrible de psychologues, mais contrairement aux autres professions de santé, c'est pas parce que on manque du nombre de psychologues formés, c'est parce que les postes ne sont pas ouverts et ça Monsieur le Ministre, c'est de votre responsabilité d'ouvrir des postes de revaloriser la la la profession au niveau du salaire et aussi de reconnaître leur formation, donc il y a encore du boulot. Monsieur le ministre, nous vous vous nous avez dit il y a quelques instants que dans 2025 je crois, vous feriez l'évaluation parce que en fait ce que vous dites, c'est que l'avenir c'est celui de l'intégration des psychologues dans le parcours de santé mentale bien sûr. Il y a un tel déficit aujourd'hui en terme de psychiatres hospitaliers, un peu plus en libéral mais on hospitalier un tel déficit avec un tel manque d'appétence aussi pour la psychiatrie hospitalière qui interroge sur le fonctionnement et les moyens qui sont donnés, service de psychiatrie qu'on voit bien la tendance qui effectivement consistera à s'appuyer sur les psychologues cliniciens en santé mentale, mais sans pour autant leur donner le statut qui va avec, alors aller jusqu'au bout, réfléchissons et travaillons ensemble sur les passerelles, par exemple, à quel moment un psychologue clinicien expérimenté ayant travaillé en hôpital peut bénéficier d'une passerelle pour devenir psychiatre ouvre la la la la la la, qu'est ce que j'ai pas dit là, Monsieur le Ministre, et je vous ai vu réagir et je m'attendais à cette réaction et pourtant, et pourtant vous y viendrez d'une façon ou d'une autre, mais sans le faire vraiment, c'est-à-dire que vous utiliserez les psychologues cliniciens, pour suppléer dans les services de psychiatrie à l'absence de psychiatres, mais vous ne leur donnerait pas le statuer la reconnaissance qui auxquels il pourrait prétendre avec des compléments d'étude et au regard d'une expérience professionnelle, je vous invite à y réfléchir parce que c'est probablement la seule voie dignes et honorables et pour la santé mentale et pour les cliniciens. Oui, madame la sénatrice, je me suis permis de de réagir, peut-être de façon excessive, mais je m'en explique, comme vous le savez fort bien les psychologues aujourd'hui ne sont pas une profession de santé, une formation qui n'a pas grand chose à voir avec la santé et en aucun cas je ne peux trait de les comparer à des psychiatres qui ont une formation non seulement médicale de base, mais en plus, une spécialité pour rapport à à la psychiatrie, toutefois, bien entendu, des psychologues cliniciens ont leur. Place à avoir dans les parcours de santé mentale, une place qu'il convient de bien préciser, je vous rappelle aussi que, par la mise en place des infirmières de pratique avancée en particulier des infernal pratique avancée en psychiatrie, qui ont un niveau d'étude de master 5 ans d'études, nous avons là aussi une nouvelle profession qui commence à arriver et qui prend sa place dans ces parcours de santé mentale, nous travaillons avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour voir sous quelle forme, adapter la formation des psychologues cliniciens, pour qu'il puisse venir vers une profession de santé et ainsi trouver toute leur place dans le cadre du parcours de de santé mentale place qui je suis vraiment désolé de le dire ici, il ne sera pas à la place des psychiatres mais sera à côté des psychiatres. Merci, donc nous allons voter sur cet amendement avec un double avis défavorable, donc il est pour cet amendement. C'est contre qui s'abstient, il n'est pas adopté, nous passons à l'amendement suivant présenté par Madame Ferret. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, cet amendement propose la remise d'un rapport concernant l'indemnisation des arrêts de travail pour les maladies chroniques, à leur insertion professionnelle, certaines maladies chroniques entraînent des soins itératif, tels que la chimiothérapie ou la radiothérapie sur une durée plus ou moins longue susceptible d'interrompre partiellement une activité professionnelle face à cette situation dans lesquelles les personnes malades ne se trouve pas en incapacité de travail en dehors du temps de soins les mesures actuelles ne favorisent pas le maintien durable dans l'emploi au-delà du temps partiel thérapeutique plus ou moins limitées dans le temps en fonction des caisses d'assurance-maladie et des trois ans maximum d'arrêt maladie prévue par la réglementation, elle se voit le plus souvent contraintes d'opter pour des dispositifs d'invalidité qui sont coûteux et précipite leur exclusion du monde du travail toutefois un arrêté de 1995 prévoit que la Caisse primaire accorde une indemnité compensatrice de perte de salaire, dès lors que les demandeurs en remplissent certaines conditions mais qui sont trop limitative cet arrêté restent malgré tout encore méconnu à la fois des personnes malades, mais également de nombreuses caisses primaires et ne mentionne que la dialyse à domicile, limitant sa portée et excluant d'emblée toute autre situation qui pourrait justifier cette indemnité, donc voilà pourquoi nous demandons un rapport pour que ce dispositif puisse être plus connu améliorer ainsi les conditions d'application pour favoriser le maintien dans l'emploi de ces personnes atteintes du maladie chroniques qui nécessitent malgré tout des soins réguliers. Madame la rapporteure. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, bon, demande de rappeurs permet effectivement de prendre une prise de parole sur un sujet important, évidemment, j'espère que le gouvernement s'en saisira pour autant c'était un rapport donc ça n'a vidé favorable au sein de ce texte, je vous remercie. Monsieur le ministre. C'est le président et dans les LCD, les sénateurs, madame la sénatrice Ferret vous souhaitez donc faire entrer dans le droit commun le dispose de l'indemnité compensatrice de perte de salaire permettant aujourd'hui aux personnes dialysé de s'absenter sur leur temps de travail pour leur dialyse en percevant une compensation financière de ces absences, à ce titre, vous réclamez la rédaction d'un rapport qui concerne l'indemnisation de ces arrêts de travail, des maladies chroniques et leur insertion professionnelle, les assurés dans la situation médicale nécessite des soins itératif peuvent d'ores et déjà bénéficier de prestations en espèces servies par l'assurance-maladie. Les indemnités journalières maladie classique des indemnités journalières au titre de l'affection de longue durée pendant 3 ans, ou des indemnités journalières, dans le cas d'un temps partiel thérapeutique dans ce dernier cas, le temps de travail à leur aménager et l'assurance maladie couvre la perte de gain, la Syrie peut bénéficier d'une pension d'invalidité s'il exerce une activité professionnelle, ces possibilités de cumul entre revenus d'activité et pension d'invalidité, seront d'ailleurs plus arguments assouplie par dispositions prévues à l'article 55 du PLFSS enfin l'assurer nécessitant une dialyse peut bénéficier d'une indemnité compensatrice pour perte de salaire, je rappelle donc que le dispositif des des indemnités compensatrices pour perte de salaire constitue une aide sociale extra-légale qui n'est ouverte qu'aux personnes dialysés à domicile, enfin, de nombreux rapports ont déjà été publiés ces dernières années concernant la prévention et la désinsertion professionnelle pour les publics vulnérables, dont les personnes atteintes de maladies chroniques, pour ces raisons je suis défavorable à cet amendement. le problème que vient de soulever ma collègue est particulièrement important, les pathologies de type cancer deviennent aujourd'hui des pathologies chroniques et bon nombres de patients veulent reprendre le travail à la suite de de leur traitement ou tout en continuant leur traitement et vous venez de parler du du problème du cumul invalidité avec donc le travail, la reprise du travail un décret de ce printemps, je ne sais plus la date exacte de de 2022, a mis en place la possibilité de cumuler donc à la fois son temps partiel et une pension d'invalidité, sauf qu'il y a un plafond qui est celui de la sécurité sociale qui est à 41136 euros, si je me souviens bien, et qui fait que des patients qui auront repris leur activité à 80 % pour peu qu'ils soient cadres voile leur pension d'invalidité diminuer et ce de façon importante, j'ai eu quelques cas sur sur mon département qui sont venus interpeller pour des pertes de 300 à 500 euros par mois, et donc en fait, plutôt que de reprendre à 80 % leur activité, ils seraient pour eux plus simple de reprendre à cinquante ou à 60 % et de toucher le complément pour arriver au plafond et inutile de se fatiguer en faisant les 4 jours par semaine, comme ils le font actuellement, donc c'est un problème d'ailleurs, j'avais l'intention de nous faire un courrier en ce sens, donc j'en profite, mais c'est un problème important parce que les pathologies chroniques aujourd'hui deviennent de plus en plus permettent de plus en plus de reprendre une activité partielle au niveau du travail. Bien, merci, donc double avis défavorable sous mais l'amendement voix qui est pour. Qui est contre.

merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement rédactionnel précise que les prestations en espèces maladie versées au micro-entrepreneurs exerçant une profession libérale, sont concernés par le mode de calcul dérogatoire sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes dès lors qu'elles le sont en pratique.

Qui est contre qui s'abstient, il est adopté, je soumets aux voix, l'article 16 bis qui est pour. Qui est contre, s'abstient-il être adopté. Sur l'article 17 j'de demandes de prise de parole la première Madame la rapporteure. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues permettez-moi un mot général d'introduction à l'article 17 qui anticipe aussi sur la présentation des 2 premiers amendements que la commission adoptée sur ma proposition et fera gagner un petit peu de temps dans la discussion commune l'article 17 mettent en oeuvre à la mesure phare du gouvernement en matière de prévention, la création d'une forme de parcours composé de 3 rendez-vous de prévention tout au long de la vie adulte et pris en charge par l'assurance maladie, c'est une idée intéressante et utile, compte tenu de la prévalence des comportements à risque et de leurs conséquences dans notre pays, mais que sait-on de ce qu'il faudrait faire en la matière, les bilans de santé en population générale ne sont pas très efficaces pour améliorer les indicateurs de santé publique, il touche peu les personnes éloignées des soins qui sont celles qui en ont le plus besoin, ils peuvent même conduire à du sur-traitement voilà ce que disent les analystes, passe au crible par la revue Prescrire, le mois dernier, c'est aussi ce que disait le Haut Conseil de la santé publique en 2009 et ce que semble dire l'expérience du bilan de santé en milieu de vie, conduite par nos voisins anglais depuis 2008, un autre exemple étranger, parfois en la matière et celui du programme du comté de Waechter Botton dans ces petits villages du nord de la Suède, si les consultations à caractère général portent leurs fruits depuis des décennies, c'est semble-t-il parce que dans ces communautés rurales à forte cohésion sociale la continuité du suivi médical est grande et l'éloignement des soins est faible, d'une manière générale, mais surtout à défaut d'une parfaite couverture de la population en médecin traitant la prévention gagne à être efficacement ciblé, soit sur la recherche de pathologies précises, c'est l'objet des programmes spécifiques, tels ceux du dépistage organisé du cancer colorectal du cancer du sein, du col de l'utérus, soit sur des populations à risque, par exemple les personnes éloignées des soins ou traversant un moment de fragilité tels que celui du chômage ou de la retraite, c'est pourquoi la Commission a accueilli le dispositif gouvernemental avec bienveillance dans les grandes lignes, mais à la condition de préciser de catégories de choses d'abord la nature du service proposé aux assurés sur ce point, l'article 17 est flou et la meilleure preuve qu'il est flou, c'est la longueur mais, chers collègues de la discussion commune que nous allons avoir, car si son contenu était net vous ne seriez pas si nombreux, mes chers collègues, à vouloir le préciser en effet pour trois rendez-vous promis, nous n'avons qu'une consultation effectivement nouvelle à 20 25 ans un rendez vous à 40 45 ans, qui pourra donner lieu à une consultation mais pas nécessairement et un examen à 60 65 ans, qui est déjà en cours de déploiement depuis le quinquennat précédent. On ne sait pas très bien par ailleurs ce que seront ses rendez-vous ou ces séances de prévention, la Commission proposant de préciser le dispositif d'abord en assurant la sincérité de la promesse faite aux assurés qui commande d'appeler consultation le service qui leur serait rendue, lequel ne pourrait se tenir à distance, car si l'on prétend faire un bilan personnalisé de santé servant notamment par exemple à mettre à jour des vaccinations, mieux vaut que le patient soit physiquement présent 2ème catégorie d'ambiguïté à lever l'objet de ces consultations en cette matière, en cette matière aussi le mieux est l'ennemi de bien mieux longs précise à quoi serviront les rendez-vous plus on les fait ressembler à des bilans globaux en population générale, lesquels sont peu efficaces et peu efficient, c'est pourquoi j'émettrai un avis défavorable aux amendements qui précise l'objet des rendez-vous car soit ils s'écartent Alexey écarte à l'excès les mailles du filet préventif, soit ils prétendent dire aux professionnels du soin, ce qu'il doit faire dans l'exercice de son métier, alors qu'ils sont alors, et alors ils sont satisfaits par l'appellation de consultation, la Commission ne prétend pas savoir mieux que la littérature scientifique, ce qu'il faut faire à ces occasions et comment cibler les assurés auxquels ses rendez-vous bénéficieront le plus son amendement propose simplement d'objectiver un minimum la chose en disposant que les occurrences des consultations soient fixées par voie réglementaire, après avis du Haut Conseil de la santé publique les occurrences pourrait d'ailleurs très bien être des bornes d'âge mais sur lesquels tous les scientifiques ne s'accordent pas forcément autant que des situations de fragilité, tels que le bénéfice de l'allocation chômage ou l'absence de médecins traitants déclaré depuis une certaine durée, quoi qu'il en soit, le succès des examens de prévention dépendra étroitement des efforts faits en matière d'aller vers les populations qui auront le plus besoin de ses examens, c'est pourquoi je vous proposerai un 3ème amendement visant à améliorer la capacité de la CNAM d'informer utilement les assurés, si nous voulons que notre pays prenne enfin le virage préventif, l'important, mes chers collègues, ne sera pas de détailler dans la loi l'objet des rendez-vous et de s'assurer que les personnes dont la situation les conduit à laisser se dégrader leur état de santé se retrouvant au moment adéquate face à un professionnel du soin qui leur accordera la considération qu'il mérite, la commission ne pouvait guère promettre davantage article 40 oblige les elle tient à ce que l'article 17 attire autant que possible la confiance des Français, je vous remercie. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, l'annonce de faire un ministère de la Santé, de la prévention était a priori une très bonne intention, c'est en effet un effet d'annonce, en réalité, cela s'apparente à du vent, j'ai fait des propositions concernant la prévention pour les jeunes de 12 à 17 ans, pour lesquels il y a un angle mort pour la prévention du suicide, prévention des risques addictif prévention pour les pathologies mentales, la vraie prévention des malheureusement pas au rendez-vous et c'est vraiment dommage, il n'y a pas de pédopsychiatres sur certains territoires comme le mien en Guadeloupe, par exemple dans les mer à obtenir un rendez-vous dans l'Hexagone, déjà c'est entre 6 et 12 mois voire plus, c'est inquiétant, c'est la santé des femmes également et Unicancer nous lien et nous alerte sur l'ensemble du territoire national et en particulier en outre-mer, il y aura et il y a déjà de très grandes disparités Monsieur le Ministre, les intentions ne valent pas toujours les actions. Monsieur le Ministre votre thème virage, la prévention, voilà une promesse gouvernementale pour ce PLFSS bien que certaines mesures nous apparaissent intéressante, nous sommes tout de même bien loin du virage, a lancé le texte ne parle que de prévention médicale qui s'apparente selon moi plus à du dépistage, cas de la prévention, aucun article ne traite de la prévention primaire, la qualité de l'air, l'alimentation, les effets de la solidarité de la sédentarité des conditions de travail et si à l'origine, notre système de sécurité sociale a été pensée dans une option curative et c'était normal et qui accapare 97 % des dépenses santé face à la montée préoccupante du Mali chronique de pour 100 par an à l'apparition aussi d'une nouvelle pandémie à l'accroissement des inégalités sociales dans le domaine de la santé, il est aujourd'hui indispensable de repenser notre modèle de santé et de prévention, son objectif ne doit plus simplement être l'augmentation des aussi 42 vie mais l'augmentation de l'espérance de se dit en bonne santé à titre d'exemple en France, 46 % des Français depuis 65 ans, sont en bonne santé, ce taux est de 77 % en Suède, si nous voulons un modèle basé sur la santé et non sur le soin, il faut agir, non seulement sur les maladies, mais sur les déterminants de la santé, ce qu'on appelle en général d'exposants, il s'agit là d'un véritable changement de paradigme, c'est-à-dire d'une approche décloisonnée de santé dans les professionnels encore aujourd'hui beaucoup trop en et et il faut prendre en considération la santé environnementale dans l'ensemble des politiques publiques, telle que développé par le concept que nous connaissons tous de santé intégrés ou à neuf, des travaux ont été menés dans cette assemblée sur cette question de la prévention de la santé environnementale, que ce soit par mon collègue Bernard Jomier ou par le groupe gestes avec Mélanie Vogel dans la mission d'information, de protéger et accompagner les individus en construisant la sécurité sociale, écologique du XXIe siècle, à laquelle j'ai participé, je ne peux que déplorer que les moeurs conclusion pourtant éclairante et constructive, n'ait pas été davantage prise en compte dans ce PLFSS. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, je je me permet de rebondir, peut-être pour gagner du temps, ensuite dans la discussion sur les les différents amendements je me réjouis de l'ensemble des amendements qui ont été faits sur ce texte sur la prévention et et je me réjouis du fait que le Sénat s'est emparée de ce sujet de la prévention, c'est la première fois, vous l'avez dit, que nous avons un ministère de la Santé et de la prévention est certes, si l'on peut peut-être déplorer que cela ne va pas aujourd'hui assez loin, c'est un 1er pas et pas loin d'être négligeables qui en plus est suivi d'un certain nombre de mesures complémentaires qui n'apparaissent pas forcément dans ce dans je suis globalement en accord avec ce qu'a dit la la rapporteure, même si sur certains points, nous aurons quelques petits différents, je voudrais préciser que l'intérêt de ces rendez-vous de prévention ce n'est effectivement pas. De toucher les publics qui vont tous les mois, à voir leur médecin et qui ont un suivi parfaitement réguliers, mais c'est bien d'aller chercher les publics qui sont les plus loin actuellement du soin et de la santé, c'est tout un des enjeux que nous avons avec les CNR territoriaux et j'ai pu constater à à Marseille dans les quartiers nord, l'intérêt des médiations et des médiateurs de santé justement dans le cadre de cette prévention, ce sera l'objet de de discussion que nous pourrons avoir une autre fois, concernant l'intérêt non seulement aller vers ceux qui sont du soin mais aussi avoir la possibilité de proposer des parcours de santé, à l'issue de ces rendez-vous prévention ce n'pas si je peux m'exprimer un One shot mais c'est bien le début d'une prise en charge beaucoup plus globale, certes, des dépistages organisés existe. Structurellement, malheureusement, force est de constater qu'ils n'ont pas toujours l'efficacité attendue, seuls 50 % des femmes qui devraient en bénéficier ont un dépistage du cancer du sein et 30 des hommes qui devraient bénéficier d'un dépistage du cancer du cancer colorectal long réellement, d'où l'importance de ces rendez-vous et l'importance surtout de ne pas entrer dans trop de détails dans ses rendez-vous prévention fais quand même confiance aux professionnels de santé pour adapter à chaque individu le contenu de ces rendez-vous de prévention, le terme consultation peut prêter à confusion, c'est pour ça qu'on ne nous avons préféré le thème rendez-vous puisque consultation pas systématiquement un médecin. Alors, je suis persuadé, et nous verrons l'avis du Haut Conseil de santé publique que d'autres professionnels de santé doivent pouvoir participer à cet effort et à cette politique de prévention concernant les jeunes de 12 à 17 ans, bien entendu, c'est une signe qu'il faut atteindre dans le cas de la prévention, c'est déjà le cas, par rapport à des examens obligatoires chez les jeunes, mais c'est aussi un des sujets, j'en parlais tout à l'heure des assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant pour repréciser également dans les éléments complémentaires, je dois vous informer du lancement la semaine dernière. D'une mission Sport santé justement dans le cas de la prévention primaire, secondaire et tertiaire cette mission Sport santé a pour objet de le compléter d'autres propositions, comme les 30 minutes d'activité sportive à l'école, les 2 heures d'activités sportives également activité physique, excusez-moi, à l'école et activité sportive au collège et au lycée, elle a pour objet de faire le point sur les maisons sport santé également plus de 500 maisons sport santé, conformément à l'engagement du président dans le plan ma santé 2000 22 et également le point sur les prescriptions de sport prescription adaptée de sport, les résultats de cette mission sont attendues pour le début, fin du 1er trimestre printemps 2020 3 et si vous le souhaitez, j'aurais bien sûr l'occasion de venir présenter les résultats de cette mission, qui est une mission pour l'instant conjointe avec la ministre des Sports et à laquelle participaient également le ministre de l'autonomie et du handicap, donc nous aurons l'occasion de venir vous présenter ses premiers résultats, si vous le souhaitez, à la commission des affaires sociales, début 2023.

C'est un amendement de la commission, merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement précise la nature des rendez vous de prévention prévues à cet article, en les renommant consultation et en proscrivant le recours à le recours à la télémédecine, afin que le service rendu à l'assuré, ressemble bien à un examen de santé, alors j'ai entendu votre remarque, monsieur le ministre, hein, mais là n'exclut pas l'autre, sauf erreur de ma part il existe des consultations sexuels réalisés par des infirmières, voilà donc le mot de consultation nez et peut-être plus plus large, mais en tout cas, me paraît plus opportun que le mot rendez-vous cette amende montage par ailleurs d'objectiver le séquençage du parcours de prévention en sollicitant le Haut Conseil de la santé publique, pour déterminer les éléments déclencheurs de ces examens, je vous remercie. Merci donc le 319 madame la Sarah. Merci monsieur le Président, la population de patients ayant été atteints de cancer et de plus en plus importante, qu'il s'agisse de patients qui n'ont plus de traitement après cancer ou de patients qui ne sont plus que par hormonothérapie hormonothérapie phase de rétablissement, en effet, si le taux d'incidence du cancer reste relativement stable chez l'homme et augmente chez la femme depuis 90, les taux de mortalité diminue dans les 2 sexes, moins 2 pour 100 pour les hommes et moins 0 7 % pour les femmes entre 2010 et 2018 selon la Ligue contre le cancer il y a quand même 3 millions huit de Français qui vivent avec le cancer et 160000 qui en décèdent chaque année, il est donc nécessaire d'adapter ses rendez-vous aux besoins spécifiques de cette population nombreuse en matière de prévention inclure un objectif de bilan aux consultations de prévention permet de prendre en compte les besoins spécifiques des populations concernées, le terme de bilan permet par ailleurs de couvrir plus largement les besoins de l'ensemble de la population au moment de ces consultations, qui pour permettre de proposer des mesures de prévention efficaces doivent proposer dans un 1er temps un bilan sur les pratiques et mesures de prévention, déjà mis en place par chaque personne concernée. Oui, merci Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord dire que effectivement ça va, ça peut paraître semblait se. Tous ces amendements une liste à la Prévert, mais moi je pense que sans être prescriptif, il est bon, tout comme dans les examens obligatoires d'ailleurs en PMI, qui est une liste un peu, dit M tout simplement sans sans pour cela, que ce soit trop prescriptif vers le médecin parce que ce dispositif, quand même, il est en l'état, relativement général. de sorte qu'il risque vraiment d'être insuffisant quant à son contenu, donc cet amendement comme bien d'autres, vise à préciser, renforcer le dispositif effectivement en l'orientant éventuellement sur un certain nombre de risques les plus courants actuellement, la Ligue, enfin d'abord seuls aurait dit contre l'obésité en 2022 17 % des Français sont en situation d'obésité, selon Santé publique France, le nombre de nouveaux cas de cancers entre 1990 et 2018 a augmenté de 68 % chez l'homme et de 93 % chez les femmes et les troubles dépressifs ont augmenté de près de 2 points entre 2010 et 2017 alors qu'ils avaient été stable entre 2005 et 2010 il touche majoritairement les femmes, les étudiants et les chômeurs enfin, selon l'Insee, en 2000 54 millions de seniors seront en situation de perte d'autonomie, donc surpoids addiction cancer disque professionnels, perte d'autonomie, tous ces facteurs, j'insiste touche selon l'adresse en majorité les classes populaires et les habitants des outre-mer, donc il s'agit bien monsieur le ministre, de s'attaquer aux déterminants sociaux de santé et donc il faut lister ces risques qui, de plus sont très inégal et également porté donc cet amendement se propose de renforcer ses rendez-vous et d'en faire un dispositif de prévention globale en mesure d'apporter un soutien efficace à la lutte contre ses principaux risques de santé et les inégalités de santé. Merci madame c'est mon jeu le suivant est un amendement de repli si je comprends bien. Au mois un autre point, un autre point, c'est pour ça que je dis que c'est une liste à la Prévert, mais bon, je redis que dans les PMI, c'est bien comme ça que que ça se passe pour les examens de santé alors là c'était plutôt seul selon Santé publique France : les troubles musculo-squelettiques et représente la première cause de maladie professionnelle en France avait près de 44500 cas recensés en 2019 ce direction n'avait pas attaqué la santé au travail et réduit enfin et et et réduit et les médecins de facto aujourd'hui qu'on recrute pas, on aurait peut-être pas besoin de le mettre dans un dispositif général selon l'étude, Some Summer rendu à Santé publique France en octobre 2022 quatre-vingt-six % des maladies professionnelles reconnues dans le BTP sont des TMS et 64 % des artisans du bé BTP déclare des douleurs musculaires et articulaires, de manière générale, selon la Darès en 2016 87 % des maladies professionnelles reconnues sont des TMS, un phénomène en hausse continue de 7 % par an depuis 2005, pas tout le monde pareil ces ouvriers qui représentait en 2012 selon la Darès la quasi-totalité des salariés du régime général, victimes de maladies professionnelles, même au delà de des thèmes et les employés sont aussi les principales victimes de cette épidémie qui a trait à la dégradation continue des conditions de travail, ce chiffre de d'Arese confirmé par l'enquête de 2020, commandé par l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail montre alors là encore des publics particuliers, les femmes, les travailleurs migrants, les personnes LGBT qui sont susceptibles d'occuper des emplois et de travailler dans des secteurs caractérisés par une Exposition accrue aux risques pour la santé et au risque notamment de TMS y compris les risques psychosociaux et les risques organisationnels comme d'autres, on vise à compléter les dispositions bienvenue de l'article 17 en renforçant les rendez-vous de prévention afin de donner la possibilité enfin d'ouvrir à la prévention des risques psycho-sociaux et des troubles musculo-ce que l'éthique.

à des âges clés de la vie qui est essentiel pour améliorer le parcours santé pour sensibiliser conseiller ou encore effectuer des dépistages et même les mises à jour de vaccination toutefois ces rendez-vous seront assurés par des professionnels de soins libéraux de moins en moins représentées, notamment dans les déserts médicaux et les territoires et départements d'outre-mer. Et des déserts médicaux sont également des déserts de prévention et des déserts numériques ou l'information est peu accessible aussi notre collègue Stéphane Artano propose que la consultation de de prévention puisse intégrer la programmation de tiers-lieux de prévention proches des patients les plus isolés pour rendent la santé publique du dernier kilomètre plus inclusive. Merci l'amendement suivant n'est pas présenté puisque le signataire n'est pas là, ensuite le 492 Madame Delmont Koropoulis.

alors Madame Jasmin. Excusez moi, le 800 77. Merci monsieur le président, la population des patients ayant atteint et ont été atteints par un cancer et de plus en plus importante, qu'il s'agisse de patients qui n'ont plus de traitement ou de patients qui ne sont plus traités par des hommes en monothérapie, en effet, si le taux d'incidence du cancer reste relativement stables chez l'homme et augmente chez la femme, il y a fort heureusement plus de décès si la population des patients doit être concerné par les rendez-vous de prévention et est nécessaire d'adapter ses rendez-vous aux besoins spécifiques de cette population en matière de prévention inclure un objectif de bilan aux consultations de prévention permet de prendre en compte les besoins spécifiques des personnes concernées, le terme de bilan permet par ailleurs de couvrir plus largement les besoins de l'ensemble de la population au moment de ces consultations qui permettraient de proposer des mesures de prévention efficace. Alors, il faudrait d'après Unicancer inclure la notion de bilan personnalisé et je crois que ce serait intéressant, monsieur le Ministre que vous y fassiez vraiment ce qu'il a à faire pour que ce soit une réalité parce que Unicancer est quand même une des références et je crois que cette proposition devrait vous permettent de prendre en charge différemment les personnes. Merci le 891 Monsieur Iacovelli. Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous le savons, la santé mentale a longtemps été un tabou trop longtemps aujourd'hui la parole se libère la santé mentale prend enfin la place qu'elle se doit dans notre système de soins parce que souffrir en silence souffrir sans que cela se voit souffrir seul c'est le symptôme d'une prise en charge défaillante quelques faits chers collègue et je me permets de vous les rappeler 64 % des Français ont déjà ressenti un trouble ou une souffrance psychique, les Français sont les plus grands consommateurs au monde de psychotropes et un Français sur 5 est touché, chaque année par un trouble psychique de l'Atlas de la santé mentale, il est indiqué qu'en 2017 plus de 7 millions d'individus ont une prise en charge spécialisée du un trouble psychique diagnostiqué ou un traitement psychotrope mais que, malheureusement, ces chiffres sont ne sont qu'une image partielle de la réalité puisqu'en effet la prévalence des troubles de santé mentale demeure difficile à caractériser à cause du non-recours des soins et de la difficulté de poser un diagnostic, c'est pourquoi nous proposons de faire de ces rendez-vous de prévention a déjà ciblé une occasion de détecter en amont, ces troubles sont tentés de préciser les missions des médecins évidemment c'est plutôt par cet amendement, le souhait de dire aux Français, après tant d'années de tabous que leur santé mentale sera un point central dans leur prise en charge pour l'avenir, je profite également de cette prise de parole pour regretter que notre amendement visant à permettre la mise en oeuvre d'une consultation de santé mentale à l'adolescence est été jugé irrecevable l'établissement d'un diagnostic et d'autant plus difficile chez les mineurs, alors même qu'à l'échelle mondiale, un jeune âgé entre 10 et 19 ans sur 7 souffre d'un trouble mental et santé publique rappelle qu'environ la moitié des troubles mentaux se manifeste à l'âge avant l'âge de 14 ans, des mesures ont déjà été prises dans ce sens par le gouvernement, nous avons que nous avons voté mais il faut continuer nos efforts en commun dans ce sens, c'est dans le but dans ce but que nous avions proposé cet amendement ciblant les adolescents et c'est avec cette même volonté que nous présenterons aujourd'hui cette précision de rendez-vous de prévention de l'âge adulte est prévu dans cet article, merci. Merci le 161 Madame Billon. je souhaite toutefois par cet amendement, vous proposer d'intégrer le dépistage de l'endométriose dans les consultations de prévention prévues à l'article 17 l'endométriose touche en France environ 10 % des femmes en âge de procréer, soit 1 virgule 5 à 2 5 millions de femmes, je cite : Olivier Véran, alors ministre de la de la Santé, lorsque l'on parle d'endométriose, on ne parle pas que d'une maladie marginal qui n'affecterait que quelques française, mais bien d'un phénomène massif le diagnostic intervient souvent tardivement le délais estimés étant en moyenne de 7 ans les patientes atteintes d'endométriose souffrent souvent d'une errance de diagnostic induisant une prise en charge non adapté de leurs symptômes, voir une aggravation de la maladie, par ailleurs, si dans un tiers des cas l'endométriose ne se développe pas stagne, voire régresse grâce aux traitements, on sait aussi que certaines endométriose vont évoluer vers des formes sévères dont la prise en charge est complexe et relève de la multidisciplinarité, c'est là tout l'intérêt d'un diagnostic le plus précoce possible pour éviter une potentielle aggravation des symptômes une détérioration de la qualité de vie, donc c'est l'objet de cet amendement, je voudrais également vous rappeler que la prévention, c'est un sujet important, nous avions avec la délégation aux droits des femmes, mené des travaux sur famille ruralité et nous avions fait lécher un déficit notamment de gynécologie médicale 13 départements sont dépourvus de gynécologie médicale 77 départements non pas un taux de suffisant de gynécologues médicaux pour faire que les femmes accèdent normalement à la prévention, au dépistage, donc oui à inscrire dans la loi ces rendez-vous Monsieur le Ministre, mais donnons-nous aussi les moyens de les réaliser, je vous remercie. Merci Monsieur le Président, cet amendement vise à inclure pleinement les kinésithérapeutes dont les rendez-vous de prévention, les consultations de prévention des séances d'information, d'éducation pour la santé de promotion de la santé de prévention proposées pour les adultes, entre 60 et 65 ans ces rendez-vous pourront donner lieu à des consultations de prévention elles séances d'information, et cetera nos politiques de santé se résume souvent à une approche curative, alors que le renforcement de l'intervention des professionnels de santé manière préventive offrirait des résultats très bénéfique pour la santé publique des politiques plus efficaces de prévention permettront de garantir un maintien en bonne santé tout au long de la vie pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d'impliquer l'ensemble des professionnels de santé aussi les proposer de matraque à contribution les compétences des kinésithérapeutes qui sont des professionnels du mouvement et de la prévention, l'implication des kinésithérapeutes dans les rendez-vous consultations de prévention et séances d'information, d'éducation pour la santé de promotion sur la santé de prévention permettra de mobiliser 100000 professionnels de santé formés et bien répartis sur le territoire, les chutes peuvent entraîner une diminution de la faculté de se déplacer et donc une perte de l'autonomie à part, avec parfois de graves conséquences en termes de dépendance pour les patients les plus âgés, les kinésithérapeutes sont particulièrement indiqué pour réaliser les bilans sur l'activité physique pratiquée et recommandé aux patients une activité physique besoins à ses besoins pour cette tranche d'âge. tient défendu bien. Le 554 Madame Bonfanti Dossat. Oui, l'amendement proposé a pour objet de préciser à l'article 17 du projet de loi les rendez-vous de prévention sont effectués par les médecins ou les infirmières qui oriente le cas échéant, vers les professionnels médicaux ou paramédicaux adapté, en effet, au moyen de grille d'évaluation, l'infirmier peut effectuer des bilans à tous les âges de la vie, et ainsi éviter de nombreuses maladies chroniques et des complications, cet amendement a donc pour objet de reconnaître la prévention comme faisant partie intégrante des missions des infirmières et infirmiers en lien étroit avec les autres intervenants à domicile, présent sur l'ensemble du territoire 365 jours par an, je ne parlerai pas des nuits et du du Mans, formés à la prévention, cette nouvelle reconnaissance ne peut que profiter aux plus 2 millions et demi de patients qu'ils accompagnent chaque jour.

Lay 11 millions datent dents estimait en France, assure un rôle crucial dans l'accompagnement et le soutien des personnes handicapées, âgées ou malades en perte d'autonomie, ils sont une ressource essentielle sur lesquels reposent et politique du maintien à domicile cependant et des régulièrement un proche a des conséquences sur la santé de ces aidants et présente également un coût pour la société, le système de santé littérature abondante met en évidence un état de santé physique dégradé chez les aidants, voilà l'analyse de la littérature internationale réalisée par l'Observatoire régional de santé d'Île-de-France, en octobre 2020 ses rendez-vous de prévention sont donc particulièrement important pour eux puisque le risque de conséquences sur la santé et on le sait tous ici, et d'oubli de leur propre santé et plus fréquent parmi cette population, cet amendement vise ainsi à repérer les aidants familiaux lors de ses rendez-vous et à prévenir les conséquences de la situation des dents sur leur état de santé, je vous remercie. Merci monsieur le président, donc l'amendement 955 il vise à ajouter à ses rendez-vous là le repérage. Des mutilations sexuelles et l'orientation des victimes qui le souhaitent, vous savez en France il y a des enfants, des adolescents et puis des adultes qui ont, qui sont, qui ont été victimes de mutilations sexuelles, on pense évidemment à à l'excision, qui qu'est-ce qui nous vient en tête, souvent en 1er mais il y a aussi de nombreux enfants de pour 100 des naissances en France, je le rappelle, qui sont des enfants qui naissent intersexes et qui sont victimes de mutilations parce que tout simplement on considère lorsque ces enfants viennent au monde que leurs corps ne correspondent pas à la vision que l'on se fait de la société et que bien souvent, au lieu de choisir de changer notre vision de la société ont choisi de changer le corps de ses enfants, la France a été en 2016 condamné 3 fois par l'Organisation des Nations-Unies, par le comité contre la torture pour ses mutilations et je sais bien sûr que cet amendement ne ne concerne que les rendez vous qui ont lieu après 18 ans, c'est effectivement la limite de cet amendement, bien sûr qu'il faut détecter ces ces cas plus tôt mais il vaut mieux tard que jamais, et je rappelle que, en France, pour les personnes intersexes il n'y a quasiment aucune personnes intersexes en France, qui n'ait pas été qui n'ait pas été concerné par des traitements, que ce soit des chirurgies ou des traitements hormonaux contre sa volonté, alors que je le rappelle, ces traitements, la plupart du temps n'ont aucun intérêt médical, les personnes intersexes vont très bien, elles sont très bien, comme elles sont, elles, peuvent avoir la vie qu'elles veulent avoir on n'a pas besoin de les modifier, et pourtant, contre leur volonté, parce qu'elles sont souvent bien trop jeune pour pouvoir consentir à quoique ce soit on décide de les modifier, avec des risques pour la santé, à la fois physique et psychique très important. Merci, cher collègue, vous avez encore l'amendement suivant et le suivant, vous en avez deux a présenté. Le 956 puis le 957.

donc le 956 et l'ajout de la prise en compte des besoins spécifiques liés au genre. Au sexe, à l'orientation sexuelle dans ses consultations, c'est une recommandation de la Haute autorité de santé dans son rapport, sexe, genre et santé de 2020, qui recommande que les politiques publiques tiennent compte des différences liées au sexe, aux gens et à l'orientation sexuelle et déploie des mesures spécifiques en fonction de, de ces critères, en France, on a 55 % des personnes LGBT qui lui a plu ce qu'ils disent avoir subi des agressions dans leur vie 65 % des personnes transgenres qui déclarent avoir été victimes de discrimination dans leur parcours de de soins ajoutez ceci à cet article, c'est non seulement garantir que ces discriminations pourrait diminuer mais c'est aussi, je crois, envoyer un message au corps médical pour qu'ils se rendent compte que hé bien ces publics-là existe, qu'ils ont des besoins spécifiques et qu'il est bon de l'avoir en tête quand ils reçoivent ces personnes. Et donc il vous en reste, hein, a présenté le 957 allez. Très bien 957 n'a rien à voir, nous sommes maintenant dans la prévention des risques de santé liés à l'environnement, nous avons fait. Il y a quelques mois, une mission d'information sénatoriale sur la création de ce qu'on appelait, de ce que le groupe écologiste appeler la sécurité sociale, écologique au début, beaucoup de groupes au Sénat nous ont répondu c'est quoi, la sécurité sociale, écologique ne comprends pas ce que c'est et puis, au fil de nos auditions et de nos travaux, je crois que nous avons atteint un consensus dans cet hémicycle, puisque le le rapport a été a été largement adopté pas sur toutes les recommandations, mais au moins sur un constat et sur une idée, le constat c'est que la sécurité sociale n'est pas prête pour faire face aux nouveaux risques qui sont liés au changement climat. Chic et une des choses majeures que nous devons faire, c'est de faire passer la sécurité sociale, d'une logique curative, c'est-à-dire d'une logique qui courent après les risques que notre modèle de société produit à une logique préventive qui est de prévenir les risques et ses rendez vous là font partie. Ce c'est pas du tout le le seul moyen, mais c'est une des dimensions que nous pourrions ajouter le fait que dans ses rendez-vous là il y a une attention des médecins, par rapport à à l'Exposition aux risques environnementaux par exemple les risques chimiques, les risques liés au bruit hier et les disques qu'il y a l'alimentation c'est un enjeu de société, c'est un enjeu de un enjeu social puisque les les risques environnementaux sont distribués inégalement dans la population en fonction de en fonction de la catégorie socio-. Et c'est un enjeu de finances publiques majeur, c'est-à-dire que si nous ne passons pas d'une logique de curative à une logique préventive, notre système de protection sociale n'est pas capable d'absorber le risque majeur pour la santé humaine et pour la planète, qui est à venir, c'est-à-dire le risque climatique. Maintenant, l'amendement 1075 présenté par Madame Ferret. Objectif. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, cet amendement concerne la prise en charge de la douleur et des séquelles, en effet, la douleur s'installe parfois durablement malheureusement bien au-delà de la fin des traitements contre le cancer ainsi au terme de la dernière étude qui était menée par la Ligue contre le cancer 78 % des personnes interrogées déclarent toujours vivre avec des conséquences du cancer ou de ces traitements et pour 30 % d'entre eux avaient des douleurs chroniques, même plus de 16 ans après la fin des traitements, or il est important de rappeler que la loi prévoit à la fois que toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur que celle-ci doit être en toutes circonstances, prévenue évaluée prise en compte et traitées et que les professionnels de santé doivent mettre en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort, cette proposition d'amendement a vocation à permettre une meilleure identification et, par conséquent, une meilleure prise en charge de la douleur et des séquelles pour les personnes atteintes ou ayant été atteintes par un cancer.

comme plusieurs amendements précédents et à venir, nous souhaitons donc compléter cet article lié au rendez-vous de prévention un certain âge clé de la vie, certains ajouts ont été adoptés à l'Assemblée nationale Post 49 3 mais d'autres non, ce que nous regrettons, c'est pourquoi nous proposons de reprendre ici un amendement qui avait été adopté en commission des affaires sociales, suite à un avis sur le PLFSS pour la première fois de la délégation aux droits des femmes, ainsi, nous souhaitons qu'au sein de cet article 17 soit précisé que les modalités, le contenu de ces rendez-vous sont adaptés aux besoins et aux facteurs de risque du citoyen et de la citoyenne, notamment les événements de santé spécifique du corps féminin, les cancers spécifiques ménopause ou encore ostéoporose loin de vouloir faire une liste à la Prévert, il s'agit ici de reconnaître que la médecine est centré sur l'homme, le corps des femmes, on le sait, ne fonctionne pas de la même façon que celui des hommes, notamment à l'échelle de la cellule et pourtant notre modèle médical est issu de connaissances recueillies sur des cellules mal, comme le démontre, Allison Grégor, médecin urgentiste, pionnière de la santé féminine aux États-Unis parce que les femmes ont des besoins spécifiques en matière de santé le contenu de ces visites médicales doit être spécifiées et adapté au corps féminin et, notamment, à certains moments de la vie, sans remettre en cause l'appréciation des médecins, je crois qu'il est essentiel de chausser des lunettes plus féministe de la santé, enlevant certains tabous, je pense notamment à l'amendement de notre collègue Annick Billon sur l'endométriose. Notre amendement s'inscrit évidemment dans la même lignée.

part Madame pour nous pensons que les rendez-vous de prévention peuvent jouer effectivement un rôle important et pour ce faire, pour être efficace, il faut délimiter les contours de ces rendez-vous, de telle sorte qu'il soit autant que possible adapter aux particularités de chacun, mais surtout de chacune, il s'agit d'avoir un regard attentif sur les événements de santé propre au corps féminin comme les cancers spécifiques Cathy on a parlé, mais également la ménopause, l'ostéoporose ou également landau mais trieuses qui doivent être sérieusement pris en considération, en étant intégré à ses rendez-vous l'égalité en droit ne peut pas être synonyme d'effacement des différences, en particulier sur le plan médical, bien au contraire ces spécificités doivent être impérativement prise en compte pour que le dispositif soit finement adapté au parcours de santé de manière égale ainsi le contenu des visites doit être impérativement spécifié adapté au corps féminin et communiquer clairement aux professionnels, de manière à ce qu'il réponde de manière la plus adéquate possible aux besoins des hommes comme des femmes, une description indifférencié du contenu des visites risquerait de fragiliser l'efficacité attendue pour les femmes d'une prévention plus que jamais nécessaire

% des 7709 personnes interrogées lors de la dernière étude menée par la Ligue contre le cancer, déclare vivre aujourd'hui encore avec des douleurs résultant du cancer et les traitements bien sûr pour le combattre, 100 d'entre elles subissent d'ailleurs ses douleurs chroniques, plus de 15 ans après la fin du traitement, le législateur doit envoyer à mon sens un message clair et sans ambiguïté : nous sommes là, nous connaissons vos difficultés, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour apporter des solutions concrètes pratiques parce que toute personne finalement le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur, le code de la santé publique prévoit en outre que cette douleur doit être en toutes circonstances, prévenue évaluée prise en compte et traitées, mes chers collègues, donc, cet amendement a vocation à permettre une meilleure identification et, par conséquent, une meilleure prise en charge de la douleur pour les personnes atteintes ou ayant été atteintes de cancer ou d'une pathologie d'une particulière gravité, je vous remercie. quarante-quatre. Alors le suivant, mes chers collègues, il s'agit d'un amendement de repli, donc ça, poursuit la même volonté, c'est-à-dire de permettre une meilleure identification et une meilleure prise en charge de la douleur, mais cet amendement ne concerne cette fois que les personnes atteintes ou ayant été atteintes de Merci le 750 Me Poncet mange. Merci monsieur le président, alors cet amendement vise à prendre en compte la prévention des troupes de la santé mentale dans les rendez-vous de prévention instaurés par ce projet de loi, donc je vais sauter déjà les arguments peut-être qu'a rappelé monsieur ne mon collègue Iacovelli peut-être dire qu'effectivement si il l'a bien pointé que les affections psychiatriques ce débute avant 15 ans pour la moitié, j'ajoute à une autre précision, elle se déclare pour 75 % avant 25 ans, hein, donc un repérage et une prison en charge précoce donc doivent réduire les risques de développement de ici station de ses troupes, à fortiori sur une population jeune, alors il faut rappeler en regard que le suicide est la 2ème cause de mortalité des 15, 24 ans, et que c'est la maladie mentale qui est le 1er, facteur de risque de décès par suicide, donc voilà la prévention santé mentale s'avère donc cruciale : l'Atlas de la santé mentale, précise les informations permettant de caractériser l'état de santé mentale des enfants et adolescents sont lacunaires particulièrement à des échelles géographiques fine en moyenne et c'est-ce cela qui est très important, je crois, de de bien préciser 8 à 10 ans séparent les premiers symptômes de la maladie mentale et le député de dépistage des troubles mentaux, comme c'est le comme celui de de mon collègue suit cette recommandation en prenant en compte la santé mentale dans les rendez-vous de prévention prévues par la loi.

médecin, une activité physique adaptée ces prescriptions reconnaissent le rôle positif d'une activité non non médicale sur le bien-être et la santé des patients cette évolution positive des mentalités peut être étendu à d'autres pratiques que le sport et c'est actuellement sur quoi se penche le Canada avec l'expérimentation prescrit nature qui permet aux médecins de prescrire à certains patients un temps passé dans la nature, pas seulement pour se ressourcer, mais aussi pour en tirer des bénéfices tangibles et vérifiables en matière de santé selon l'une des professeurs responsables de cette expérimentation expérimentation de 20 à 30 minutes en nature réduit cinéphile significativement la prévalence de la dépression abaisse le taux sanguin de cortisol l'hormone du stress, la pression artérielle et la fréquence cardiaque, en plus de stimuler la mémoire et la créativité sans aucun effet indésirable, il nous semble intéressant d'étudier toutes les pistes, concourant à la bonne santé des patients, il s'agit ici, pas de remplacer le médicament mais de le compléter par d'autres pratiques, j'ajoute que l'impact sur les comptes de la Sécurité Sociale serait minime. Merci le 979 Monsieur dessus. Oui, donc les rendez-vous de de prévention prévues par le présent projet de loi aux âges clés de la vie sont une excellente chose, notamment pour la prévention qui doit être développée ces rendez-où doivent aussi l'occasion de sensibiliser les patients sur les causes de développement de certains cancers, mais nous souhaitons aller plus loin : depuis quelques années, la commission scientifiques alertent sur l'augmentation alarmante des cancers dits précoce c'est-à-dire diagnostiqués avant 50 ans ces cancers ont beaucoup à voir avec des causes environnementales et lié au mode de vie ainsi, sur les 14 types de cancer qui sont en augmentation chez les moins de 50 ans, 8 sont liées au système digestif, ce qui doit nous alerter sur nos habitudes alimentaires, mais aussi surtout sur le système de production et de commercialisation de l'agro-industrie si la prévention est un volet fondamental de la détection ne doit pas non plus être négligé, face à cette augmentation inquiétante des cas de cancer chez les jeunes, nous proposons ainsi que les rendez-vous de prévention soit l'occasion de proposer à tous les patients, quelle que soit leur âge, des solutions de dépistage adapté en fonction de leur profil et de leur mode de vie repérer diagnostiquer sont des piliers indispensables à la politique de santé, surtout dans les cas de cancers qui peuvent être qui qui peuvent mettre de nombreuses années à se développer, les rendez-vous de prévention semble le lieu idéal pour porter cette politique nouvelle et détection des cancers précoces telle le but de cet amendement. Merci le 754 Me Poncet Monge.

nous porte notre attention sur les douleurs chroniques, parfois même plus alors moi j'avais 16 ans et on a dit 15 ans bon après la fin des traitements, je vais peut-être rajouter à ce qui a été déjà dit par Madame Ferret et Madame Morchio que, selon une étude des chercheurs villa

je rappelle pas le code de la santé publique qui, qui prévoit donc quand on dit qu'on y fasse bien attention et ce dispositif donc doit s'adapter à l'augmentation. Sensible du nombre de cancers au sein de la population et proposer une prise en charge des douleurs et des séquelles séquelles liées au cancer, donc c'est une prise en charge en fait spécifique de la douleur et de ses séquelles pour les patients atteints ou ayant été atteints du cancer lors des rendez-vous de prévention instaurés par ce cette loi merci. Merci madame la Sarah de le 500.

Le 691 allez-y. Oui, merci Monsieur le président, donc l'amendement de notre collègue Jean Sol a vocation à permettre une meilleure identification et, par conséquent, une meilleure prise en charge de la douleur et des séquelles pour les personnes atteintes, où il a été atteinte de cancer. madame Micouleau, pardon, excusez-moi. que l'information à la prévention de santé visuelle sera hein bien incluse dans les différentes démarches de prévention prévues par le gouvernement lors des rendez-vous de prévention aux âges clés Merci madame Vogel le 958 défendu madame Meunier le 1067. Oui, merci Monsieur le Président, cet amendement propose d'intégrer la prévention de la fertilité. Pardon madame Meunier là hein donc Merci, cher collègue, c'est vrai, j'arrive, cet amendement, donc le 1067 propose d'intégrer la prévention de l'infertilité dans les consultations de prévention, l'infertilité touche près de 3 1000000 300000 de nos concitoyennes, chiffre qui va croissant, à rapport a été rendu au gouvernement en février 2022, il préconise la mise en place d'une véritable stratégie nationale de prévention et de recherche sur l'infertilité, je le cite : la prévention de l'infertilité ne doit pas se concevoir au niveau individuel, uniquement, elle doit aussi aussi comporter un volet collectif, social et politique, le recours à la PMA, on le sait, n'est pas un remède miracle, il n'y a que 20 % de succès environ, ce qui veut dire 80 % d'échec : c'était un parcours de combattante de combattants qui laisse des traces, l'information et la prévention, notamment chez les jeunes, permettrait un dépistage précoce de certains cas d'infertilité et permettrait d'anticiper la prescription de protocoles médicaux : un couple sur 4 France a du mal à avoir un enfant, et nous pouvons diminuer le recours aux PMA par une telle par une meilleure information du public, en permettant une prise en charge précoce l'infertilité est un enjeu de santé publique majeur qui n'a jamais été réellement traités comme il doit l'être par les pouvoirs publics, ça fait des années que nous le préconisons un diagnostic précoce de l'infertilité peut éviter des parcours long et coûteux, nous avons la possibilité de faire changer les choses à heure ne passons pas à côté, cette fois encore, merci. Madame Meunier le suivant le 1072. Le 1072 donc, pour intégrer le dépistage de l'endométriose dans les consultations de prévention

je pense qu'il y a déjà eu des amendements dans ce sens, tout à l'heure en séance, je sais que le gouvernement a constitué un groupe de travail associant l'institution, l'ARS, les conseils nationaux professionnels et les sociétés savantes, les associations de patientes et les personnes qualifiées sur ce sujet, cadre d'orientation nationale pour la structuration des filières endométriose existe sur le territoire et complète la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose avec cet amendement, nous pouvons faire un pas de plus vers vers la prise en charge plus rapide de l'entre-Mitry hausse ce qui aurait des répercussions sur la prise en charge de l'infertilité, par ricochet, merci. Merci ensuite 3 amendements identiques, le 1er présenté par Monsieur monsieur le président je vais le retirer cet amendement, ce que je regrette beaucoup d'avoir participé à cette liste à la Prévert et j'en parlerai après je retire l'amendement et je regrette d'en avoir cosigné quelques-uns. trois cent vingt-six madame la Sarah. Oui je dire quand même un mot pour être plus proche du besoin de population le contenu, les mesures de promotion des consultations doit faire l'objet d'une consultation annuelle des centres de lutte contre le cancer, par les agences régionales de santé.

que celui qui vient d'être défendu, donc je vais en insistant bien sur le nombre d'une nouvelle fracture et le coût total que ça représente sur l'année pour pour la Caisse nationale d'assurance maladie et en n'insistant aussi sur l'évolution démographique de la population française et qui est le dire que le nombre de fractures devrait augmenter de 30 % et des dépenses pourraient atteindre plus de 6 milliards d'euros par an à l'horizon 2025 donc, cet amendement vise à mettre en place des rendez vous de prévention de la fragilité osseuse. non, je vais partir, et monsieur le président merci messieurs, monsieur le Ministre, pardon, c'est effectivement un nouvel amendement concernant la prise en charge de la douleur, nous avons proposé la rédaction d'un alinéa complémentaire après l'alinéa 5 je ne reviens pas sur les arguments concernant cette problématique de la douleur et des séquelles, mais pour bien insister vont nous avons été nombreux à porter ce type d'amendement sur ce sujet : démonstration est ainsi faite que cela n'est pas précisé dans l'article 17, or c'est vraiment un sujet extrêmement important pour toutes celles et ceux qui sont concernés. Bien, merci, donc, la présentation de tous ces amendements en discussion commune est terminé, donc je vais demander à Madame, la rapporteure de donner son avis sur l'ensemble de ces amendements. je vais faire très court : Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues sont c'est un avis favorable sur l'amendement 47 de la commission et un avis défavorable sur l'ensemble des autres amendements. Et. Bien, merci Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, j'ai essayé de très court mais je serai un tout petit peu plus loin, madame la rapporteure, si vous permettez, concernant l'amendement 40 7 suite à la discussion que nous avons eu tout à l'heure je : je maintiens ma position en disant que j'y j'y suis défavorable concernant les les amendements 319 492 877 et globalement les amendements qui suivront, qui part du détail de de ces consultations, ces consultations concernent systématiquement une approche globale de la personne dans un concept extrêmement personnalisé et dans un concept également de de santé globale Gwenaëlle. Comme on en parle, actuellement, le Haut Conseil de santé publique sera amené à préciser les grands éléments de ces, de ces rendez-vous de prévention, j'ai failli dire consultation de ses rendez-vous de prévention et ainsi que les personnes qui seront habilités pour les faire donc défavorable concernant l'amendement 750 défavorable également, tout en souhaitant préciser que les risques psychiques et physiques au travail dépendent aussi et essentiellement de la santé au au travail même remarque pour l'amendement 752 avec un avis défavorable. l'amende, les amendements 616 998 sur la notion de tiers lieux la question peut se poser et d'ailleurs l'objet de discussions dans le cadre des CNR santé territoriaux en l'état, ce serait un avis défavorable. La notion de bilan personnalisé des amendements 319 492 et 877 j'ai déjà répondu, en particulier en ce qui concerne le cancer et cette approche personnalisée donc défavorable concernant l'amendement 891 il est satisfait, donc à moins d'un d'un rejet, ce sera défavorable de la même façon pour l'amendement 61 concernant l'endométriose prise en charge bien sûr déjà dans le le plan endométriose la santé des femmes, vous le savez, atteindre les objectifs principaux, il y a certes, diminution des gynécologue-obstétricien mais il y a aussi les sages-femmes qui ont maintenant la possibilité d'avoir un rôle dans ces parcours de santé et tout l'intérêt de ses examens de prévention sera justement de réorienter les patients vers des filières qui ont déjà été définis précédemment donc défavorable, le 314 c'est également un avis défavorable, quand on parle de d'autoriser les kinésithérapeutes, les compétences des personnels chargés de faire ses rendez-vous de prévention seront définies par le Haut Conseil de santé publique, c'est le même avis pour le 389 donc défavorable concernant les chirurgiens dentistes de la même façon, pour le 554 et pour les mêmes raisons concernant les infirmiers libéraux concernant l'amendement 452 de madame la sénatrice Guinness repérer les aidants familiaux, les proches aidants lors des rendez-vous prévention c'est un avis favorable Stéphane effectivement quelque chose qui n'avait pas été identifiés lors des discussions préalables et je souhaite mettre un avis favorable concernant l'amendement 955 madame Vogel sur les problèmes de mutilations sexuelles, c'est un avis défavorable puisque. Des rendez-vous seront personnalisés, de la même façon, pour le

c'est pour cela de l'avis est défavorable, défavorable également pour le 1075. Défavorable, ce projet pour les 834014 terre quarante-quatre de repli concernant le cancer, la santé mentale 750 défavorable également considérant que ça fait déjà partie du du contexte des rendez- vous de prévention en ce qui concerne le 980 concernant les moments nature défavorable, rien ne s'oppose en effet à ce que l'activité physique adaptée, se déroule dans un milieu naturel et et au contraire. Le 979 défavorable également le 754 qui revient sur les cancers satisfait donc rejet ou des sinon défavorable, le 500 concernant la également défavorable 692 également 370 l'importance certes de la prévention santé visuelle mais défavorable car fait partie du bilan global et personnalisée de la même façon que des addictions sur l'amendement 958 concernant l'amendement 1067 sur l'adaptation des rendez vous de prévention besoins de santé des femmes en intégrant la notion de prévention d'infertilité semble que cette notion est intéressante, a précisé tant les notions d'infertilité sont méconnus cela reporte également à l'article dix-huit les infections sexuellement transmissibles étant une des causes majeures d'infertilité chez la femme, j'aurais donc pour cet amendement, un avis favorable pour le 1072 l'endométriose défavorable, nous en avons déjà parlé, je vous remercie Monsieur Millon d'avoir retiré l'amendement 173 pour les 326 et 448 concernant la fragilité osseuse l'vie est également défavorable pour les mêmes raisons, comme pour le mythe sur la douleur : avis défavorable, je vous remercie. sauf sur le 47 pour Madame la rapporteure et avis défavorable de Monsieur le Ministre, sauf sur le 1067 je précise que l'adoption de l'amendement 47 de la commission qui aurait dit intégralement lésiné à les alinéas 4 et 5 fera tomber tous les amendements de la discussion commune qui apporte des modifications au sein de ces alinéas, les seuls amendements qui ne seront pas concernés par le fait de tomber, c'est les 443 et 444 de Madame font Borchio Fontimp parce que ils rajoute un alinéa qui n'était pas inclus dans c'est trop rédaction de l'amendement 47 donc Monsieur Merci monsieur le président je pense que cette discussion est parti sur de mauvaises bases et on le voit dès l'amendement 47 et l'échange entre le ministre et la rapporteure sur rendez-vous consultation parce que, au fond, le virage de la prévention que vous nous proposez là dans ce dispositif, Monsieur le Ministre, on ne sait pas si ce sont des consultations médicalisée ou pas, c'est ce à quoi tend en fait la rapporteure en disant c'est des consultations mais j'entends là dans la bouche du ministre hypothèse de rendez vous et moi je souscris au fait que la prévention ne doit pas être nécessairement médicalisé et que il y a tout un ensemble de professions qui pourraient contribuer à ces consultations à ses rendez-vous de prévention Agnès Buzyn quand elle était ministre, avait commencé à légiférer sur les conseillers en environnement intérieur et à faire émerger cette profession, je crois que là on a lancé la discussion sur, je vais me faire beaucoup de de pas amis dans l'hémicycle, maintenant tout le monde a porté des thématiques importantes sur le fond. Mais ça n'aura aucun intérêt tous ces amendements excusez-moi chers collègues n'ont aucun intérêt, ils n'ont aucune portée normative et donc tous ces thèmes sont importants, mais il n'y a pas d'intérêt à voter ça, non mais Monsieur le Ministre, parce que vous avez voulu dès ce texte affiché un virage de la prévention, vous, on vous en donne acte, mais que le dispositif n'est pas du tout prêts en fait, hé bien le débat semaine ben des amendements sans intérêt au lieu de discuter de savoir qui doit faire de la prévention dans notre pays, ce sont les médecins, ce sont d'autres professions de santé, ce sont des professions qui ne sont pas catalogué comme profession de santé, ben moi je réponds oui, que ce n'est pas de la prévention uniquement médicalisée et là comme on est parti, la suite logique c'est discuter dans la convention de la valeur des actes, des consultations de prévention et rien d'autre, voilà et donc je trouve que on s'égare, on s'égare et je ne voterai pas, pardon, l'amendement de Madame Imbert, parce qu'il semble refermée du coup vers la prévention médicalisé et je préfère à tout prendre qu'on en reste à la rédaction actuelle mais avec une grande insatisfaction. Merci, je vais donner la parole aux autres qui l'ont demandé juste en précisant une chose, je crois que j'ai fait une petite erreur, c'est-à-dire qu'il y avait également un avis favorable de Monsieur le Ministre, pour l'amendement 452 de Madame 10 Days, donc il y avait 2 2 amendements avec avis favorable Madame Bonfanti Dossat. Oui merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, moi j'ai du mal à comprendre la prévention, c'est l'essence même de la profession des infirmières libérales que dit votre projet de loi, il met l'accent sur une priorité : vieillir à domicile et pour bien vieillir à domicile, on ne peut pas s'affranchir d'une bonne prévention qui garantit un maintien à domicile, en bonne santé, alors Monsieur le Ministre, certes, les intentions sont là les effets d'annonce aussi, mais vous n'avez pas les moyens de votre politique. Monsieur Millon. Oui, mais merci monsieur le président je vais pas revenir sur ce qu'a dit Bernard Jomier je suis d'accord avec lui et je pense madame reporter que nous avons eu tort d'opposer, rendez-vous de prévention et consultation, c'est vrai que si on met consultations médicalisent le rendez-vous et on est peut-être pas obligé de le médicalisé, faire un rendez vous de prévention me semble plus utile directement puisqu'on peut rencontrer différents types de professionnels dans ce cas-là, une consultation, c'est un professionnel médical je voudrais ajouter des choses par rapport à ce qui a été dit, parce que dans la liste qu'une qu'on nous a donné, si nous mettons en place cette liste les rhumatismes inflammatoires n'y seront pas l'optique n'y est pas le VIH n'y est pas le VHC n'y est pas, la surveillance des vaccins n'y est pas, la validation des vaccins n'y est pas, et

donc restons-en au texte du gouvernement qui me semble être, pour l'instant, le meilleur travaillons par la suite pour améliorer les choses aux votants aujourd'hui le texte qui est demandé par Monsieur le Ministre, je crois que c'est plus que nécessaire afin d'éviter évidemment des erreurs qui serait malheureuse pour l'ensemble de nos concitoyens, et en particulier dans le cadre de ses rendez vous. De santé. Madame Vogel. Oui, merci Monsieur le Président, moi je voulais juste exprimé une une frustration vis-à-vis de la manière dont on discute globalement de de cette partie prévention du PLFSS en réalité, on sait que l'enjeu principal des dépenses maladie à venir, c'est l'augmentation des maladies chroniques et des maladies liées à l'Exposition aux risques et plus globalement aux risques environnementaux chimiques climatique et et la manière dont on discute la manière dont on dont dont. Fabriquer notre procédure budgétaire, de mon point de vue nous empêche en tant que parlementaire, vraiment, de faire les propositions qu'il faut faire pour faire que notre sécurité sociale, soit à la fois qu'elle remplisse son rôle, c'est-à-dire de protéger les individus face au risque, mais aussi qu'elle soit financièrement stable, il y a beaucoup de propositions que le groupe écologiste avait formulé qui ont été déclarés recevables Arctique quarante ça aggrave les dépenses c'est c'est tout à fait, c'est une évaluation tout à fait subjectif, moi je crois que c'est même le contraire, un exemple, l'allocation universelle alimentaire qui est une des recommandations de notre rapport de la mission sur la sécurité sociale, écologique, demande de réfléchir à la mise en place d'une telle allocation moi je crois que c'est l'inverse : ça améliorer largement les comptes de la Sécurité sociale si les personnes avaient accès à une meilleure alimentation, manger mieux les personnes seraient moins malades et on aurait moins de dépenses maladie et donc en réalité, la manière dont on réfléchit à nos dépenses à la sécurité sociale en général, la manière dont on construit la procédure budgétaire nous empêche, je pense, de faire des propositions qui sont de notre responsabilité et là en l'occurrence, tous les amendements qui avait vocation à faire ce que je crois, devrait être la sécurité sociale du XXIe siècle, c'est-à-dire une protection sociale qui protège contre le risque majeur qui le risque environnemental tous ces amendements ont été rejetés, et donc en quelque sorte, moi j'ai l'impression que on ne peut pas faire notre travail. Madame Mellow. Merci monsieur le président, monsieur le ministre madame la rapporteure, mes chers collègues, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit par mon collègue Monsieur Millon, ainsi que par Monsieur Jomier je crois qu'il est intéressant de de considérer que la prévention peut être faite par d'autres,

l'amendement 616 parce que c'est un lieu où les les personnes isolées, les personnes qui n'ont, qui n'irait pas dans d'autres structures peuvent aller et où on peut pratiquer vraiment de la prévention, je suis allé à l'inauguration d'un tiers-lieux et j'ai trouvé cela fort intéressant, il y a une multiplicité d'offres que ce soit nutritive ou sportive et on peut y ajouter la prévention médicale, bon, je pensais que cet amendement était intéressant, donc je voulais le souligner et souligner l'importance des tiers-lieux tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Si Madame la rapporteure. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, une petite précision toutefois sur cet amendement 47 l'alinéa. 4 dit tous les adultes de 18 ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comporte notamment, ça c'est le texte du gouvernement, c'est bien d'accord : mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comporte notamment et, effectivement, la commission a remplacé au lieu de dire des rendez vous de prévention, elle a été mis des consultations de prévention. Chez le kiné, c'est une consultation chez l'infirmière, c'est une consultation, vous avez des consultations pour la les provinciaux sexuelle porte cette par des infirmières chez la chasse ça chôme, ce sont des consultations donc le mot consultation va au delà, là, l'article ne dit pas : consultations de prévention par un médecin généraliste ou par un médecin spécialiste, voilà c'est tout ce que je voulais vous allez vous faire remarquer, mes chers collègues. Monsieur Chassang. Monsieur le président, monsieur le Ministre, mes chers collègues, moi je, effectivement je je prendrais l'interprétation de Madame la rapporteure parce que effectivement c'est : c'est bien une consultation alors après, et même si vous voulez pour l'amendement, de Madame est ce qui est un peu particulier mais ça fait partie aussi des consultations et les personnes qui vont recevoir ou qui vont, qui peuvent être effectivement d'autres professionnels de santé que le médecin, mais elles vont pouvoir aiguiller la personne vers d'autres professionnels pour la prendre en charge, mais c'est au départ, ça me paraît bien être une consultation. Madame la la présidente. je, je voulais soutenir ce qu'a dit Corinne Imbert on est on est sur un problème de de santé en effet de alors de consultation pour moi qu'elle soit faite par des sages-femmes par des infirmiers n'fait par et et les médecins ou les professionnels de santé, mais on est bien quand même, sur quelque chose qui touche à la santé, or je pense que si on veut que ce soit efficace, il faut que les personnes qui qui qui fasse ces moments où le patient ou le citoyen va être vu soient soient formés pour le faire, parce que sinon ça reste quelque fois quelque chose de ce qui peut être sympathique, entre guillemets, mais l'objectif c'est quand même d'arriver à détecter chez une personne les fragilités, les vulnérabilités qui méritent, en effet, que que ce soit pris et et je pense que l'amendement de Corinne Imbert il rédigé ainsi, et c'est bien qu'il le soit ainsi après ça n'empêche pas d'avoir un effet des des Liens qui se fasse avec, avec d'autres, si on est-ce qu'on fait un peu dans les contrats locaux de santé ce que l'on fait avec d'autres personnes, mais quand même, lorsqu'on veut prendre un citoyen et et regarder là où sont les méthodes ou les moyens de prévention et sentir là où il a besoin de d'être suivis de rentrer d'un parcours de soins comme l'a dit monsieur le Ministre, il faut, et pour moi, le terme de consultation qui n'est à aucun moment, ça n'a été con mais consultations par un médecin, hein, c'est une consultation, c'est c'est un interrogatoire, c'est ce qui est une consultation un interrogatoire un examen un examen physique éventuelle, je pense que vraiment on peut maintenir ce là sans risque quant à tout ce qui a été dit, bien sûr qu'on partage l'endométriose la santé mentale, la fertilité, les cancers, bien évidemment, partage ce que elle été dit mais justement si c'est fait par un professionnel par quelqu'un qui a cette connaissance de ce qu'est la santé en général, de ce qu'on ait pathologies parce, charge à lui après de, de, de définir justement avec la personne qu'il voit ce qui est le mieux adapté comme parcours de soin comme parcours je partage ce que dit Mélanie Vogel, je pense que dans les difficultés et les problèmes de financement de notre système de santé, on a des moyens en effet peut-être de, de trouver des marges de manoeuvre, on envoie et autres, mais je pense que dans à moyen terme, à court terme, même à court terme, mais à moyen terme, le meilleur moyen de faire baisser les dépenses en santé dans notre pays, c'est la prévention, c'est indéniable, tous les cancers évitables toutes les maladies chroniques, tout ça c'est c'est ça arrive est il faut le prendre en effet dès le plus jeune âge, mais aussi à tous les âges de la vie, j'aurais pu rajouter plein de choses sur le dépistage de l'hypercholestérolémie les familial sur beaucoup de de pathologies où je reçois régulièrement des soit des associations de patients, soit à chaque fois, on sent bien que que le problème il est au niveau du dépistage et du diagnostic d'un traitement précoce et je pense que la prévention et à terme, le meilleur moyen d'arriver à à financer notre protection. Merci donc j'ai encore 3 demandes de prise de parole, je vous propose de les donner, puis ensuite on passera au vote, je pense que Madame Poncet. Donc, Donc, puisqu'on nous invite à prendre du Champ, à prendre de la hauteur, je dirais que si les mutuelles, les organismes complémentaires de santé n'était pas en fin de compte, obligé de venir combler les de remboursement de la Sécurité sociale où les dépassements, on en a parlé tout à l'heure des des spécialistes des médecins qui ont leur justification, mais qui sont quelquefois abusive, ils pourraient faire ce pourquoi ils peuvent être faits, enfin il serait pertinent, à savoir faire de la prévention, ça a été dit par le le groupe CRCE si vous voulez, là on a vraiment les mutuelles, elles ont un Champ entier à côté de la sécurité sociale mais un Champ entier qui devrait être celui-là et non de de pallier le recul le déremboursement de la sécurité sociale, d'ailleurs, les mutuelles se plaignent de ne pas être associés à ces rendez-vous, c'est le rendez-vous de de prévention, elles font remarquer que, elles ont elles-mêmes mis en place des dispositifs de soutien psychologique qui sont beaucoup qui ont touché beaucoup plus de population, j'ai pas les chiffres que les femmes, dispositif que le le groupe communiste voulait annuler donc vraiment elle le montre si vous voulez, et elle sur le fait que, elles ont demandé d'être partenaire de ses rendez vous de santé et que le le gouvernement qui voulait justifier effectivement seront l'ajout de la prévention à côté du ministère de la santé ont refusé alors que je pense que vraiment c'est un acteur essentiel et d'ailleurs, pour ceux qui ont une mutuelle, je terminerai là-dessus quand on part à la retraite et qu'on a une bonne mutuelle, hé bien, on a une demi-journée à une journée de cet âge, paraît-il, critique où on passe à l'inactivité ça pas été critique, pour moi, mais bon voilà et donc ils savent faire, ils le font donc voilà réintégrer les complémentaires santé dans leur vrai vrai rôle la prévention. Merci monsieur Hainaut. Oui merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, je voudrais reprendre au fond en quelque sorte la les arguments de Madame de roche, je pense que cette question de la prévention, une la grande question de notre système de santé pour le XXIe siècle, et surtout dans notre pays où le Docteur Knock et a fait beaucoup de tort sur la question de la prévention, hein, et sur la peur qu'on peut avoir d'aller chez le le médecin c'est donc culturelles

c'est d'abord l'affaire des personnes et puis c'est l'affaire du médicale et je dirais même du médico-social et si je prends l'exemple de, de, de, de, de ce qui concerne le bilan des 4 ans autrefois, c'était la seule affaire des des médecins et puis il est advenu que quelques fois les les médecins du fait de la rareté était remplacé dans cette bilan par les infirmières et je crois que c'est un exemple et c'est comme ça qu'il va falloir et il me semble que cet amendement va dans le sens du renforcement de la prévention en en en ouvrant cette cette possibilité, autant que faire se peut, je vous remercie. Merci Monsieur Savary. Oui, merci, moi je voulais remercier Alain Milon, d'avoir soulevé le problème qui a permis de donner des explications par la rapporteure, parce que c'est vrai entre rendez-vous et consultation, ce qui est important, c'est que il y a un professionnel de santé ou un même avoir une médical ou d'autres personnes, Monsieur le Ministre de la prévention selon les différents territoires et c'est là où je voulais en venir, merci aussi à Madame, la rapporteure d'avoir mis un amendement reprécise en notamment que et la Haute autorité de santé va t terminer hein ça dans un certain nombre de thèmes, c'était pas, me semble-t-il, dans le texte initial, donc on voit bien qu'elle traverse la il y a des avis divergents, mais qui peuvent converger parce qu'il y a tout à faire dans la prévention, mais Monsieur le Ministre, je voulais attirer votre attention, être hein, au plus près du territoire, et faire en sorte que non seulement il y a des consultations très bien, mais que des gens se déplacent pour aller voir celles et ceux qui ne sont pas directement sensibilisé à ces problèmes de prévention et la prévention, c'est à la fois sanitaires ça à la fois sociales sociales et et il peut y avoir également la prévention du handicap mais c'est également professionnel, notamment si on veut faire en sorte que dans cette société il y a une vision différente des seniors, ce rendez-vous sera tout à fait ça permettra véritablement de faire en sorte que la société voit complètement différemment les choses à la fois sur le plan de la santé mais également sur le plan de la branche vieillesse, avec une réforme des retraites qui interpelle déjà nos concitoyens mais qui méritent véritablement d'être approfondie. merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, un un mot rapide, mais encore une fois, pour remercier de de l'ensemble des débats sur cette question de la prévention, bien entendu, nous sommes, nous sommes au début du chemin, il reste pas mal de de choses à faire quelques petits points on, on m'a demandé l'autre jour, ce qu'était la prévention, j'essaie de de trouver un petit peu une formule pour dire ce qui était la prévention finalement celle que j'ai trouvé, c'est la prévention, c'est d'abord prendre soin de soi et je pense que c'est peut-être ça qui est aussi, explique toutes nos discussions de savoir qui fait de la prévention, la prévention, c'est d'abord quelque chose d'individuel et il faut former notre société à à cette politique de prévention, en ce qui concerne les, les différentes discussions je me propose de revenir très clairement auprès de la commission des affaires sociales sur 3 sujets si vous le voulez bien le premier dès lors que nous aurons le le rapport du Haut Conseil de santé publique pour en discuter avec vous des tenants et des aboutissants concernant les contenus de cette prévention, la façon de les mettre en place, j'en parlais tout à l'heure sur le sport santé également, si vous souhaitez en discuter, vous parliez, madame la présidente de gain le sport santé, ça permet d'éviter 4 cancers sur 10, 8 maladies cardiovasculaires sur 10 est un enjeu majeur et et c'est un enjeu qui est rapidement applicables enfin le le 3ème point pour faire le lien avec les tiers-lieux le texte en l'état, n'interdit en rien de faire de la prévention, au niveau des tiers-lieux au contraire simplement évalué et c'est probablement une discussion qui est beaucoup plus locale et et je reviens là-dessus, sur le 3ème point vers lequel je me proposerai de venir à l'issue du du 1er trimestre 2023 vers la commission qui est celui des médiateurs en santé, c'est-à-dire c'est personnel, ces citoyens qui font l'interface entre le système de santé et les personnes qui sont au plus loin dans une logique de de aller vers médiateur en santé, pour lequel j'ai confié une mission à la Docteur Philippe de Normandie pour faire le point là-dessus pour la fin du 1er trimestre 2023 je vous remercie. voter, donc nous allons commencer par voter sur l'amendement 47 proposé par la commission, qui est une réécriture des alinéas 4 et 5 de cet article, donc avec un avis défavorable du gouvernement et un avis favorable de la commission évidemment qui est pour le l'amendement numéro 47. Qui est contre.

donc tous les amendements de la discussion commune tombe puisque, comme l'amendement 47 qui a été adoptée réécrit les alinéas, il ne peut plus y avoir d'amendements sur les alinéas qui préexistait à la à l'adoption de cet amendement, donc même ceux qui ont reçu un avis favorable parce que Madame du gouvernement tombe à cause de l'adoption de l'amendement numéro 47 c'est la procédure, c'est comme ça, donc il reste 2 amendements qui n'étaient pas concernés par cette réécriture, donc l'amendement 443 de Madame beaucoup Fontimp avec un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté 444 même botte j'imagine même vote, donc nous Nous poursuivons avec 4 amendements en discussion commune le 1er présentée par Madame Jacques mais le 700. Merci monsieur le président, Monsieur le ministre, à Madame, la rapporteure le présent amendement propose que les rendez-vous de prévention à certains âges clés de la vie qui participe de la volonté d'un virage préventif dont nous pouvons collectivement nous réjouir puisse donner lieu à une prise en charge par les contrats de complémentaire santé et par la complémentaire santé solidaire pour qu'elle puisse se diffuser et toucher les populations les plus concernées, la dynamique de prévention primaire doit pouvoir s'appuyer sur l'implication conjuguée de tous les acteurs en contact Direct avec les assurés sociaux dans l'exercice de leur droit à la protection sociale, c'est pourquoi l'association des AMC à la définition et au cofinancement de ces nouveaux rendez-vous de prévention et souhaitable, d'une part, le financement par les AMC de ces consultations aidera à définir juste tarif compte tenu de la durée de ces rendez-vous, d'autre part, la définition précise des conditions de réalisation de ces rendez-vous de prévention dans leurs conditions tarifaires devraient faire l'objet d'une négociation avec les médecins, à laquelle les AMC feront partie, mes chers collègues, vous l'aurez compris c'est l'intérêt d'un partage plus équilibré des dépenses dans la prise en charge de ces rendez-vous de prévention instaurée à l'article 17 de ce PLF qui justifie le présent amendement, je vous remercie. Merci un amendements identiques présentés par Madame Jasmin. Le 1056. merci Monsieur le Président, donc c'est identique et l'implication de tous les acteurs est très important pour la prévention, je crois que les complémentaires le font déjà la Mutualité, le français, entre autres, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui pourraient apporter un plus dans la mesure où il est nécessaire et plus que jamais nécessaire que la prévention pour ne pas la présidente de la commission des affaires sociales, a dit la prévention va permettre également de résoudre beaucoup de problèmes pour les finances de la Sécurité sociale. Merci l'amendement 48 présenté par Madame la rapporteure. au de 25 ans les complémentaires pourront ainsi contribuer à l'effort d'aller vers les populations pouvant le plus bénéficier des consultations et ainsi aider à porter le taux de recours à ces consultations au-delà de l'objectif que s'est fixé le gouvernement, à savoir de 15 pour 2023, à titre d'exemple et je vais revenir sur le dispositif MonPsy les complémentaires ont efficacement contribuer à la prévention santé mentale, les dispositifs de prise en charge de séances de psychologue en 2021 ont permis de financer de 3 millions de séance en 2021 bénéficier auprès de 430000 personnes qui ont utilement compléter le dispositif MonPsy qui n'a, lui, permis de remboursé que 130000 séance bénéficiant à 39000 personnes au total, je vous remercie. Merci et un amendement présenté par Madame Filleul. Il est retiré, monsieur le Président, compte-tenu des échanges que nous avons eu près préalablement sur la délimitation des rendez-vous en question. OK merci donc avis de la commission sur les trois amendements en discussion commune enfin sur les 2 autres puisque sur le ventre. Oui, monsieur le président, ce sera évidemment un avis favorable à celui de la commission quant aux amendements 700 et 1000 56 qui supprime la dispense du ticket modérateur pour les consultations de prévention et pour l'ensemble des consultations de de prévention, là que la commission partage en partie l'analyse des auteurs de l'amendement, mais préfère maintenir la dispense du ticket modérateur pour les plus. Pour les plus jeunes, pardon, qui n'ont pas forcément de couverture complémentaire donc la Commission conserve le dispositif du gouvernement pour le 1er rendez-vous 20 25 ans, pris en charge en totalité par l'assurance maladie et propose une participation des complémentaires pour les 2 autres rendez-vous à 40 45 ans, et 60 65, donc c'est une demande de retrait à des fois un avis défavorable pour ces 2 amendements. les sénateurs Madame la rapporteure concernant les les trois amendements, l'un des enjeux majeurs de de la réussite de cette politique de de prévention, c'est essentiellement l'accessibilité financière pour l'ensemble de nos concitoyens à ses rendez-vous de prévention, il est impératif, je le disais en préambule qu'il touche les personnes les plus éloignées du système de santé. C'est pourquoi, et suivant les engagements du président de la République ses rendez-vous de ce prévention seront intégralement pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. Toutefois, les complémentaires ont bien sûr un rôle très important à jouer dans le cas de de la prévention et son particulier particulièrement investi dans le cas de la prévention en en entreprise dans le cadre de contrats d'entreprises et elles auront de toute façon un rôle à jouer, à participer à la promotion et au financement des dispositifs d'aval sur des thématiques qui ne seront pas pris en charge complètement par l'assurance maladie, on peut en citer quelques-unes, la diététique voir l'activité physique, si on n'est pas dans le cadre de la prescription d'une activité physique adaptée, un travail de concertation est en cours avec les organismes complémentaires sur des points financier de ce Plfss, mais également sur le Champ de la prévention pour toutes ces raisons, je vous demanderai de retirer ces trois amendements, à défaut, j'y serai défavorable. Bien, donc sur les deux amendements identiques 700 et 1000 56 ceux qui sont, il y a une double demande de retrait, ils sont maintenus. Vous le retirer. Et Madame Jasmin. Il est maintenu, donc nous votons sur l'amendement 1056 avec un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient n'est pas adopté ensuite amendement de la commission le 48 présenté par Madame la rapporteure avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Il s'abstient-il être adopté suite amendement 49 présenté par Madame la rapporteure au nom de la commission. Merci monsieur le président, président, ce Ministre, mes chers collègues, cet amendement reprend certaines des dispositions qui avaient été proposées lors de l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, qui visait à préciser la faculté pour l'assurance maladie, d'envoyer des informations ciblées aux assurés, ainsi qu'à sécuriser la transmission des données entre professionnels de santé, ces dispositions présentées isolement dans un article additionnel dans le Plfss pour 2022 avait été déclarée irrecevable car en elle même dépourvu d'impact sur les comptes de la Sécurité sociale, mais elle se rattache cette fois-ci très directement au dispositif de l'article 17 c'est l'enjeu essentiel pour assurer le succès du dispositif peut-être Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous préciser les moyens que l'assurance maladie qui seront déployés pour aller vers, je vous remercie.

je tiens à rappeler que l'assurance-maladie communique déjà tout au long de l'année pour favoriser l'accès au au droit et aux soins pour aider à adopter les bons réflexes se prémunir contre certaines maladies ou encore développer le bon usage du système de santé cette communication se fait de manière dématérialisée par le biais de l'espace Amélie parfois par des courriers postaux et surtout depuis le vingt-deux 2022 les assurés disposent d'un espace numérique en santé pour simplifier les parcours et les échanges entre les professionnels et les usagers se d'évolution de mon espace santé qui remplace ce dossier médical partagé permet une messagerie sécurisée pour les échanges et permet aussi de mettre en avant un certain nombre de mesures de prévention et aussi de participer à d'aller vers mon espace santé, il faut le le remarquer, de l'ensemble des assurés sociaux ont été interpellés sur l'ouverture de ce carnet de santé, un petit peu numérique mon espace santé et la France doit s'enorgueillir d'avoir 98 % d'avis favorables, que 2 pour de nos assurés sociaux qui ont refusé de se faire ouvrir mon espace santé ce qui le place dans le meilleur dans les les meilleurs résultats au niveau européen dans le cadre de la rendez-vous de de ces mises en place de rendez vous de prévention, il est évident que mon espace santé sera lui aussi un des éléments pour aller vers, comme je le disais tout à l'heure, les médiateurs en santé dont j'ai rapidement parler le ministère de la Santé, de la prévention de l'assurance maladie mettront tout en oeuvre, comme lors de la crise Covid pour la vaccination pour informer les assurés éligible de l'existence de ces rendez-vous aussi ouverte avec les les fournisseurs de logiciels chez les médecins pour signaler les âges et et prévenir également ses patients des âges de rendez-vous tout ça interface et avec mon espace santé mon espace santé qui ouvrent la porte aussi à des applications tiers qui vont permettre d'entrer là dedans, bref, tous les moyens sont sont mis en oeuvre et pour cette raison, je serais plutôt défavorable à votre amendement. Bien donc amendement de la commission et qu'un avis défavorable du gouvernement nous votons, qui est pour.

OK et Madame Delmont Koropoulis idem il est retiré bien. Donc ils sont retirés, donc je vais mettre aux voix l'article 17 qui est pour l'article 17. Qui est contre. Qui s'abstient. Nous passons aux amendements, il est adopté, pardon, nous passons aux amendements après l'article 17 le 416 madame Pumerole. merci Monsieur le Président, nous avions déposé un amendement concernant le remboursement d'activités physiques adaptées mais compte tenu du problème de de recevabilité, nous avons été retoqué et donc, nous demandons un rapport qui va venir remplacer qui va nous permettre de parler de son nous parlons déjà depuis une heure et demie à peu près sur l'intérêt de la prévention et vous-même, Monsieur le Ministre, vous avez avez noté tout à l'heure, l'intérêt du sport et santé et j'ai bien entendu qu'il y avait une mission ministérielle qui était chargé de faire un rapport là dessus, donc on pourra pas être à en bénéficier, vous avez vous-même évoqué le fait que l'activité physique et sportive qu'on fait une prévention de 4 cancers sur 10 de 8 pathologies cardio-cardiovasculaires sur 10, je crois que l'intérêt de l'activité physique adaptée, non pas en prévention primaire mais par exemple dans les suites d'un cancer, on sait, nous avions une audition de chercheurs de l'INSERM dessus qui montre que on a au moins 24 % de récidive de cancer du sein en moins chez les femmes qui ont dû l'activiste plutôt que celles qui ne font pas de sport, donc si on a besoin d'une promotion de cette activité physique adaptée et pour qu'elle soit bien suivi, il faut qu'elle soit prise en charge au niveau des remboursements de la Sécurité sociale, ce rapport, c'est pour bien mettre en évidence l'intérêt qu'il y aurait à rembourser l'activité physique adaptée dans la prévention, en particulier des récidives de cancer. ma collègue, on connaît la conclusion, néanmoins je vais prendre le temps de de lui répondent, puisque cet amendement demande effectivement un rapport sur l'expérimentation prévue en 2019 par la loi de financement de la Sécurité sociale pour pour 2020, qui créé un parcours de soins post-cancer comprenant notamment de l'activité physique adaptée de sujet mérite c'est vrai d'être approfondie car les connaissances progressent sur les bienfaits de la prescription d'activité physique, mais je crois que le diagnostic, il est, il est fait sur ce sujet, la Haute Autorité de Santé vient d'ailleurs d'adopter en juillet dernier un guide sur la consultation à la prescription médicale d'activité physique, il est vrai par ailleurs que l'évaluation prévue par l'expérimentation là elle n'a pas donné lieu, ou plutôt d'a donné lieu qu'à quelques paragraphes dans le rapport annuel sur les expérimentations article 51 de la des suivante c'est loin d'être un désintérêt du sujet, mais comme on on connaît le le devenir des, des, des demandes de rapport, je propose un avis défavorable. Monsieur le Ministre. Oui, monsieur le président, et ça faisait, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, bon bien entendu vous avez compris mon mon intérêt pour l'activité physique adaptée d'une façon générale juste préciser que à l'heure actuelle, 26 expérimentation article 51 sont en cours, dont les résultats sont programmés, mi-2023 qui nous permettront de faire le point à ce moment-là de façon plus précise également sur le remboursement dans le cas des préventions, secondaire, tertiaire et une interrogation aussi dans le cadre de la prévention primaire je considère donc votre demande est satisfaite et je vous demande de rejeter cet amendement. Alors donc double avis défavorable je soumets l'amour.

Merci président alors cet amendement. Demande un rapport. Allô. Pourtant, sur l'état des lieux de la prise en charge de l'obésité et du surpoids dans les territoires dans les articles 73 et 74 de la Constitution, en effet, qu'on voulait sauver le taux d'obésité dépasse 20 % de la population dans les territoires ultramarins alors qu'il est proche de 15 un hexagone, les chiffres sont flagrants 30 % de la population est en surpoids sur ces territoires, l'étude publiée par l'adresse, l'année dernière, analysant pour la première fois la situation des outre-mer a permis de soulever un enjeu de nouveau la prévalence de l'obésité est encore plus marquée chez les femmes dans les territoires d'outre-mer, Mayotte est le plus touché avec 34 % d'obésité parmi les femmes de 15 et plus, et même plus de 50 % après après 45 ans, le rapport de mes collègues des Affaires sociales a démontré tout l'intérêt d'analyser ce phénomène mais le restera à trouver des pistes de réflexion spécifique, pourrait prendre plus plus précisément sur à cette situation dans les territoires ultramarins, mes chers collègues, il y a donc urgence à mettre en oeuvre une prise en charge adéquate de l'obésité et de surpoids et du surpoids. Un autre maire la remise du rapport qui vous est proposé serait ainsi un 1er pas vers une meilleure prévention et l'amélioration de cette situation, je vous remercie. Madame la rapporteure. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, bon, vous connaissez la conclusion de mon intervention, ça sera un avis défavorable, puisque c'est une demande de rapport sur la prise en charge de surpoids et d'obésité, il est vrai que ce sont des enjeux de de de santé. Public de première importance, comme l'a montré aussi l'excellent rapport qui lui existe sur le le surpoids et d'obésité, de nos collègues, Chantal de scène Brigitte des visas, de visas il est tout récent, puisque ce rapport date de juin dernier, il ne portait certes pas exclusivement sur les outre-mer mais il faisait la synthèse des informations disponibles sur le taux d'obésité dans ces territoires, il évaluer les politiques de prise en charge et listait un certain nombre de propositions pour améliorer la lutte. Contre le surpoids et l'obésité dans l'Hexagone et dans les outre-mer, que vous souhaitez, je pense, et du coup, satisfait, peut-être pas, peut-être pas en totalité, peut-être pas dans le détail, mais je vous invite à le consulter en tout cas je pense que ça ne justifie pas une demande, une nouvelle demande de rapport et je vous propose le retrait ou à des fois un avis défavorable. Monsieur le ministre. C'est le président madame la rapporteure, mesdames et messieurs les sénateurs, même avis que que la rapporteure, une petite précision, le volet outre-mer du PNNS IV publié le le 30 septembre 2 villes 22 montre bien toute la volonté d'agir pour lutter contre la sédentarité, améliorer la la maîtrise, la nutrition dans nos Terres d'outre-mer. C'est, c'est tout l'enjeu du CNR santé CNR santé qui dans au niveau territorial dans ses déclinaisons ah justement le Champ de de la prévention je suis amené à à me rendre à Mayotte, à la fin du mois pour assister là aussi voir les travaux d'un CNR et je ne manquerai pas d'insister sur l'importance de la nutrition et du contrôle de la nutrition dans la dans la prévention santé

Alors on on le soumet aux voix, alors donc il est maintenu, donc, qui, qui, avec un double avis défavorable qui est pour cet amendement. Qui est contre. N'est pas adopté. Nous passons maintenant à l'article dix-huit avec plusieurs demandes de prise de parole Monsieur Chassang. président, monsieur le ministre, mes chers collègues, donc si vous voulez, après l'article 17 je voudrais saluer l'action du gouvernement concernant la prévention puisque l'élargissement du du remboursement des dépistages sans ordonnance des infections sexuellement transmissibles, en plus du VIH et il y avait que le VIH vous savez que ça c'est dû aux bactéries, virus, parasites, un enjeu de santé publique puisque, au niveau donc des femmes s'entraîne stérilité et et des grossesses extra-utérines, mais aussi chez l'homme des complications aigües et chroniques donc cet objectif de remboursement des IST, autre que le VIH sans ordonnance et une prise en charge intégrale si inférieur à 26 ans, donc, que je salue tout cela mais je regrette si vous voulez que ça puisse pas être pris en charge tout le temps et donc j'avais fait effectivement un amendement pour que cela puisse se prolonger après 26 ans, et il a disparu, peut-être dû à l'article quarante mais je le regrette.

ma collègue Annick Billon et moi-même tenons à saluer cet article dans lequel est introduite une mesure importante visant à faciliter l'accès au dépistage des infections sexuellement transmissibles dites IST, rendant ces dépistages accessibles sans ordonnance dans tous les laboratoires de biologie médicale et étendant leur remboursement à 100 % pour les moins de 26 ans, cependant la santé sexuelle concerne toutes les classes d'âge, une infection sexuellement transmissible non dépistés provoque des cas d'infertilité chez de plus en plus de femmes adultes qui découvrent parfois trop tard, une infection pourtant bénigne lorsqu'elle est prise à temps, il apparaît dès lors nécessaire que l'accès à ces dépistages soient au maximum facilité pour les populations adultes également, actuellement, les tests de dépistage du VIH et le seul test à être gratuit sans ordonnance pour toutes et toutes pour tous et toutes sans limite d'âge, et j'insiste sur ce point depuis le 1er janvier 2022, il serait donc souhaitable à terme et cela et le sens de cette prise de parole d'envisager la gratuité à tout âge des dépistage des IST, notre présidente Catherine Deroche ne disait tout à l'heure, le meilleur moyen de faire baisser les dépenses de santé et la prévention et je crois que c'est bien ce que nous vous proposons là, alors Monsieur le Ministre, je livre cette suggestion à votre réflexion, je vous remercie. Vous voyez le numéro. Oui, merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre, j'ai trouvé que cet article 18 pour vous alerter sur un petit problème concernant un un virus important, celui de l'hépatite C, l'élimination du virus de l'hépatite C à horizon 2025 est un objectif de santé publique qui figurent dans le plan Priorité prévention 2018, 2022 pourtant, l'objectif n'est pas atteint et selon Santé publique France en 2019 près de 100000 personnes étaient touchées par une infection VHC, beaucoup ayant été précédemment dépister mais ne sont pas entrer dans un parcours de soins, pourtant, les études épidémiologiques du sur le VHC ont permis d'identifier notamment de familles de patients pouvant être pris en charge d'une part, les personnes ayant été exposées à du sang ou des tissus infectés et, d'autre part des populations en situation de forte précarité est particulièrement exposée au risque de contamination à l'instar, par exemple, des usagers de drogue au regard de ses particularités épidémiologique de la circulation du vieux acheter favoriser le dépistage des patients affectés joue évidemment un rôle majeur dans l'élimination du virus pour les patients déjà dépistés et pour les patients qui ignorent qu'ils sont porteurs du virus, grâce aux nouveaux traitements et l'optimisation des parcours de soins permise notamment avec l'ouverture universelle de la prescription des antiviraux à action directe les à des des patients infectés peuvent être plus efficacement et rapidement prise en charge, on leur évite ainsi de développer des pathologies chroniques graves comme la cirrhose ou le cancer du foie alors je tenais, Monsieur le Ministre, à vous alerter sur le fait de l'absence de résultats suffisants par rapport au plan Priorité Santé et de la nécessité, donc de faire une meilleure information, merci. Merci, cher collègue pour ses interventions, il n'y a pas d'amendement soumis à votre vote sur cet article donc je vais soumettre aux voix. Monsieur le Ministre vous dire un mot. Merci monsieur le Président, rapidement, mesdames et messieurs les sénateurs, pour vous remercier de de vos remarques, je vais intégrer dans la réflexion dans l'évolution ultérieure du texte, effectivement, je rappelle que ces infections sexuellement transmissibles augmentent de façon très importante au cours de ces dernières années chez l'homme comme chez la femme de plus de 50 % en ce qui concerne le chlamydia 30 % en ce qui concerne le gonocoque, et qui a vraiment besoin de d'agir rapidement à ce sens et je vous remercie. merci, je vais soumettre aux voix, l'article 18 qui est pour l'article dix-huit. Qui est contre. Qui s'abstient-il être adopté, nous passons l'article 18 bis, avec une demande de prise de parole de Madame Jasmin. Merci monsieur le président, il est vraiment nécessaire de maintenir cet article la drépanocytose doit nous concerner tous nous devons plus que jamais nous investir dans la prévention de la drépanocytose et je prends la parole ici parce que j'ai contribué très fortement à des travaux concernant la drépanocytose j'ai cosigné plusieurs publications. Avec le professeur Jean Rosa, Frédéric Atheros, le professeur Berchel et beaucoup d'autres et je crois que nous devons faire un travail sérieux et non pas faire n'importe quoi, il est nécessaire de maintenir cet article et de l'Hadopi, la Haute autorité de santé n'a pas encore publié de décrets, les promesses n'engagent que ceux qui les font après le la défection concernant la 5ème branche je ne peux accepter une telle méthodologie l'expérimentation pour la drépanocytaire là de panneaux Cytos est nécessaire, le nombre de drépanocytaire il est là, donc c'est une démarche qui devrait être utile quand le décret sera publié, on pourra toujours Antonio Conte, la prévention et les expérimentations doivent être prises et prise en compte réellement, j'étais co-signataire comme je vous le disais pour concernant plusieurs. Hémoglobine Avec, à l'époque certains que j'ai cité, mais aussi pour la découverte de l'hémoglobine aux auprès tapis l'hémoglobine senti donc je crois qu'il est important que nous puissions donner toute sa place à la drépanocytose et n'a plus laissé seulement les associations, faire ce qu'ils ont à faire : récolter des sous alors qu'il y a beaucoup de maladies qui n'en n'ont pas la même importance je crois que nous devons être sérieux à un moment donné, donc Monsieur le Ministre, vous l'avez dit cet après-midi au cul agir répondant à l'un de nos collègues tous les champs de la santé de l'enfant. Vous ce comté de travailler sur tous les champs, vous l'avez dit, alors, il est aujourd'hui question de cela, la drépanocytose soutenu de plus en plus par les associations, les ben bénévoles, l'État doit aujourd'hui ainsi que vous-même les collègues vous en en Paris, je vous remercie. Merci madame Jasmin, donc nous passons à l'examen du premier amendement présenté par Madame la rapporteure. merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet article 18 bis propose en effet à titre expérimental, pour une durée de 3 ans, la réalisation d'un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire et c'est vrai, j'ai proposé à la commission un amant se un amendement de suppression parce que la Haute autorité de santé qui, en 2014 avait émis un avis défavorable à ce dépistage ensuite en 2018 je crois, oui, c'est le défenseur des droits, qui avait souhaité que ce dépistage et lieu et la maman de, de, de travail sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, nous avons une information que la Haute autorité de santé était sur le point d'émettre un avis. contraire à celui enfin qui avait évolué depuis 2014, à savoir un avis favorable systématique et obligatoire du dépistage de la Dream drépanocytose et l'amendement de suppression était simplement pour dire : ben l'expérimentation n'a plus de sens si derrière la vida HS c'est pour un dépistage systématique et obligatoire, c'était en ce sens que j'avais pensé cet amendement de suppression, maintenant je vais je vais interroger Monsieur le Ministre, pour savoir s'il a plus de nouvelles sur cet avis, je regrette que cet avis ne soit pas publié au moment où nous étudions ce texte mais si toutefois les informer. Sont donnés par le ministre nous sont favorables, tout cas vont dans le bon sens, je retirerai, un amendement de suppression. Monsieur le Ministre. Monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les députés, nous, nous on ne reviendrait pas sur les sénateurs pardon. Après. Fatigue un peu cette. Je recommence, monsieur le président, madame la rapporteure mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. Je ne reviendrai pas sur, sur la gravité de de la drépanocytose et les perturbations que ça entraîne au cours de la vie pour pris en charge à plusieurs reprises des crises veino occlusive aiguë, c'est particulièrement compliqué, je tiens à remercier le député Thomas Mesnier d'avoir déposé cet amendement à la commission des affaires sociales qui nous a permis d'éclairer de façon plus nette la problématique de de la drépanocytose, alors je vous rejoins l'avis de la HAS est attendue dans les jours, dans les semaines qui viennent, probablement favorables à cette à ce dépistage pour autant pour autant nous avons besoin d'un peu de temps pour évaluer cette faisabilité, les moyens de la mettre en place et le coût que représentera un tel dépistage qui serait généralisé, c'est pour cela je serais plutôt favorable parce que vous retiriez cet amendement, faut de quoi je serais défavorable mais en tout cas, n'ayez aucun doute contrat mon engagement et l'engagement du ministère à à développer ce dépistage de la drépanocytose. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, bon vous l'avez bien compris, j'étais pas contre ce dépistage, c'était juste me dire l'expérimentation n'avait pas de sens si d'un autre côté, la Haute autorité de santé dit oui c'est important. Attends, il faut le rendre obligatoire systématique voilà c'est dans ce sens-là, j'entends que l'avis de la Haute autorité de santé ne va pas tarder, j'entends qu'il faut un petit peu de temps au gouvernement, voilà, je reste très favorables à ce dépistage parce que je pense que la Haute autorité de santé, a un avis important pertinent et que ça va aller dans ce sens-là dont je retire si mes collègues en sont d'accord, cet amendement de suppression. Bien, donc, l'amendement est retiré, donc maintenant nous allons examiner l'amendement 1079 de Madame Jasmin. Merci madame la rapporteure, merci Monsieur le Ministre, merci à vous tous, alors il s'agit par cet amendement de reprendre une proposition du colloque drépanocytose en France ouvrant les yeux sur une maladie invisible qui a eu lieu en juin 2021. La drépanocytose et la première maladie génétique en France et aujourd'hui plus que jamais avec les brassages de population parce qu'on a trop souvent dit qu'il s'agissait d'une maladie pour les noirs, c'est une maladie génétique, mais maintenant, beaucoup de personnes sont était hétérozygote et on a de plus en plus de naissances d'homozygote ici, alors il faudrait prendre une décision, est ce qu'on veut vraiment maîtriser les coûts avec la sécurité sociale ou est-ce qu'on veut faire quelque chose, donc moi je dis que là n'est pas n'aussitôt étant cette première maladie génétique en France et dans le monde parle, parce qu'en France dans le monde, pourtant, elle reste très largement inconnue du grand public et ne bénéficient pas de visibilité médiatique et politique à la hauteur de l'enjeu de santé publique qu'elle représente, aujourd'hui, il est proposé de généraliser ce dépistage, on en a parlé, et de faire en sorte qu'il y ait

nous devons faire de cet effort là c'est important de faire cet effort là et ça va vous faire gagner de l'argent, si c'est ça que vous craignez, Monsieur le Ministre, donc aujourd'hui nous devons prendre la mesure de ce que cela représente pour l'ensemble de la population, et pas uniquement pour les noix. merci à vide la de Madame la rapporteure sur cet amendement. du dépistage des hétérozygote je ne suis pas certaine l'opportunité d'intelligent élargissement mais c'est pas à moi de le dire, alors que la Haute autorité de santé est censée rendre et on on vient de le dire public son avis sur la question dans les prochains jours, l'un des enjeux principaux de son avis concerne les enjeux éthiques associées au dépistage de l'hétérozygote que dira-t-on une personne dépistée pour l'une des maladies génétiques rechercher mais ch'laquelle on trouvera aussi une mutation que le associé à un risque élevé d'un cancer par exemple, voilà, je n'ai pas forcément la réponse et c'est plutôt vous proposer de retirer l'amendement et d'attendre aussi la position de la HAS à défaut sera un avis défavorable. Monsieur le Ministre. Monsieur le président, madame la rapporteure mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, effectivement le le hétérozygote il n'a, n'a pas de retentissement pour la personne concernée et ne nécessite aucune prise en charge particulière les enfants hétérozygote ne nécessite ni surveillance particulière ni traitement la question effectivement qui pourra se poser sur la base de l'avis de la HAS ce que nous attendons tous, c'est la modalité d'information des parents en cas de de découverte, une Ray Ozzie Gotti, à l'occasion du dépistage, celles-ci n'ont pas d'impact pour la santé, donc c'est un sujet qui soulève des questions éthiques qui font bien sûr l'objet d'une attention particulière

Les hétérozygote, c'est vrai, ne ils transmettent, ils ne sont pas forcément malade mais ils transmettent et 2 hétérozygote peuvent donner un SS, donc un homozygote et la maladie en plus un hétérozygote pu rencontrer effectivement quelqu'un qui a une thalassémie et on a justement tout le pourtour méditerranéen, beaucoup de personnes qui ont dû thalassémie, donc il faut à un moment donné, prendre au sérieux ces problématiques là d'autant plus que, à la naissance, évidemment, il y a beaucoup, qui ont encore de l'hémoglobine foetale qui se portent plus ou moins bien, mais quand le diagnostic est fait avant, et un diagnostic anti-natal et fait avant les parents savent à quoi s'attendre les médecins et également, mais la et les biopsies de troupeaux Blast, on peut les faire à l'époque, ça se faisait couramment, en outre, mais on le fait plus ou moins, il y a un centre caribéen, qui est devenu un service hospitalier aujourd'hui en Guadeloupe et qui s'occupe justement pour toute la Caraïbe ici aujourd'hui dans l'Hexagone, il y a à faire quelque chose, donc, la HAS n'a rien fait, peut-être qu'il le fera, mais en attendant, je voudrais qu'on vote ceci, ça sera peut-être comme beaucoup d'amendements parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de de questions également écrit au gouvernement qui ne répond jamais juste, ils deviennent caduques alors en ce moment, nous sommes sur un Champ qui est précieux, qui est important, je crois que nous devons voter cet amendement et si la HAS fait effectivement son travail et prouve que, effectivement, qu'il avait une cohérence entre ce que vous êtes en train de dire et ce qui devrait devrait être fait, hé bien il n'y aura pas de problème, on ne va plus tenu compte de l'amendement, parce que la HAS pour le moment on n'en est pas là, alors soyons sérieux. Non, mais par rapport à ce timing quoi moi je voulais savoir, Monsieur le Ministre, si l'HAS rend un avis favorable, vous avez dit qu'il fallait un délai, mais ce qu'on peut, ce que vous pouvez vous engager à ce qu'on le trouve dans le PLFSS de l'année prochaine la généralisation parce que il ne faudrait pas que l'expérimentation dure trop longtemps, après un avis favorable quand même de la la AS voilà c'était ma question. Monsieur le Ministre. Oui, monsieur le président, Mesdames et messieurs, je je prendrai effectivement dans mes éléments de réflexion, l'avis de la HAS, bien entendu, n'ayant pas encore cet avis : je ne peux pas m'engager en quoi que ce soit pour l'instant, mais effectivement le temps que nous avons entre la discussion ici et la nouvelle discussion à l'Assemblée, permettra de compléter la réflexion.

Qui est contre qui s'abstient, il est adopté, nous attaquons l'article 19 avec plusieurs demandes de prise de parole Madame Laurence Cohen. Merci Monsieur le Président, juste quelques mots pour soutenir l'une des rares mesures positives de ce Plfss 2023 en effet, cet article propose d'antan, d'étendre aux majeurs, la délivrance gratuite de la contraception d'urgence en pharmacie sans prescription médicale, l'objectif est bien évidemment d'éviter des grossesses non désirées et limiter ainsi le recours à l'IVG pour rappel : il existe 2 types de pilule dite du lendemain qui ont un coût : entre 4 et 20 euros, ce qui peut constituer un frein financier pour les plus précaires, d'ailleurs il est effectivement plus opportun de parler de contraception d'urgence, plutôt que de pilules du lendemain qui peut induire en erreur car, en réalité, le délai d'efficacité va de 72 heures à 120 heures après le rapport sexuel non protégé, selon la Haute autorité de santé la contraception d'urgence est bien connu des jeunes en particulier, des très jeunes, plus de 95 % des moins de 30 ans et 97 % des 15 19 ans, mais on constate que plus l'âge augmente, moins les modalités de délivrance sont clairement identifiés beaucoup ignorent qu'elle peut être délivré sans ordonnance, d'où la nécessité de mieux informer, nous n'avons pas donc d'opposition à l'amendement de la rapporteure Carole Corinne pardon Imbert pourtant sur le domaine réglementaire de cette information, l'essentiel étant que cette information se fasse bel et bien, et ce de façon régulière, en attendant, nous voterons cet article, je vous remercie. Monsieur Chassang. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, donc je suis allé tout à fait dans le même sens que Laurence Cohen, c'est une prise en charge, élargi aux majeur de la contraception d'urgence en pharmacie sans prescription médicale, c'est ça qui est important, si vous voulez actuellement 90 % ou plus des contraceptions d'urgence ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, parce que pour avoir une prescription médicale, il faudrait avoir un rendez vous chez le médecin et les dames bien sûr sont obligés d'aller à la pharmacie, le plus rapidement possible donc a actuellement donc la prise en charge est à 100 % pour les mineurs sans prescription médicale mais sur prescription médicale pour les personnes qui sont elle serait remboursée à 100 % si elles ont pas 26 ans, 65 %, plus de 26 ans, peu importe, c'est une proposition qui me paraît très important qu'il faut saluer donc gratuité de la délivrance sans prescription médicale, de la construction d'urgence à toutes les femmes, c'est une avancée, merci. Madame Rossignol. Monsieur le Ministre je, je vais me greffer sur cet article 19 parce que c'est lui qui m'a semblé plus proche du sujet dont je voulais vous parler, et en fait je voulais vous parler de la la loi du de de la loi du 3 mars 2022, et en particulier de la liste que vous avez publié cette semaine des établissements autorisés à pratiquer, être centre expérimentateurs de l'IVG instrumentale, la liste que vous avez publiés se limitent à 18 Centre, dont la moitié en Île-de-France et ça crée un certain émoi chez les professionnels et formateurs, enfin tous les les gens qui ça, qui sont les sages-femmes, bien entendu, tous les gens qui soutiennent cette expérimentation et qui sont investis, puisque des dossiers aussi sérieux le CHU de Nantes, CHU de Tours CHU d'Amiens, hôpital de la Croix-Rousse, Centre hospitalier d'Annecy d'bonasse de Blois de Vierzon, ces établissements n'ont pas été retenus alors il y a 2 options : soit une liste complémentaire est en cours de préparation dans vos services et ce serait une excellente nouvelle, si vous nous le disiez ce soir au Sénat, soit vous avez une approche malthusienne de ces centres d'expérimentation et des critères qui sont pas pas connus et pas compréhensible mais j'espère qu'il y a une liste complémentaire que vous allez nous annoncer. merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs concernant l'IVG instrumentale et ses centres j'avoue là, ne pas avoir une réponse à vous apporter immédiatement mais je vous la porterez ce soir en ayant récupéré des des informations entre temps. donc nous nous passons aux amendements, le premier amendement : c'est l'amendement 51 madame la rapporteure. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, applicable aux mineurs, et en ce qui concerne la dispensation de la contraception d'urgence dans les eaux. Piscine, sachez qu'il y a le comité d'éducation sanitaire et sociale de la pharmacie, le 16 femmes qui met à disposition des professionnels de santé. Des brochures, des cartes d'information que le professionnel de santé peut bien sûr remettre et qui doit remettre pour la bonne information à à la femme qui vient chercher la pilule du lendemain, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle dans le langage courant, donc, même si la contraception d'urgence ne concerne pas que les 2 formes de de pilules voilà donc sachez que cette information est disponible pour les professionnels de santé et qu'ils se doivent de la remettre aux patientes ouais. Merci, monsieur le Ministre sur cet amendement. Merci monsieur le président, Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, effectivement, vous proposez de supprimer cette précision qui a été ajoutée par les députés, et il est vraiment essentiel d'informer pleinement les femmes non seulement de des circonstances de la contraception d'urgence, mais aussi du retour vers une contraception normal ou d'une aller vers une contraception plus normal, la HAS a émis en 2019 des recommandations qui rappelle aux pharmaciens, l'importance de souligner ce caractère exceptionnel de de la contraception d'urgence et d'orienter vers une contraception régulière, la HAS recommande mais ne fait que recommander la délivrance d'un dépliant d'information contraception d'urgence qui rappelle aussi la gratuité de la contraception régulière pour les moins de 26 ans, je pense qu'il est important d'insister et et de mettre dans ce cadre législatif cette obligation d'information, c'est pourquoi dans ce cas dans la, je serais plutôt défavorable à votre amendement.

Qui est contre. Qui s'abstient. Donc, l'amendement est adopté, l'amendement 960 madame Vogel. Merci monsieur le président, tout d'abord : je voulais évidemment m'associer aux prises de parole précédente sur sur le fait que cet article est bienvenu et vous présenter ici un amendement qui est, j'en suis désolé, une demande de rapport sur le l'extension de la gratuité à la contraception, ils comprennent la contraction d'urgence, on a permis la gratuité de la contraception pour les femmes jusqu'à 26 ans, c'est très bien, c'est une très bonne mesure, bon elle a quelques quelques limites puisque elle n'est appliquée qu'à la première prescription et uniquement pour certaines pilules, beaucoup de femmes qui ont même qui ont moins de 26 ans, non, ne peuvent pas en bénéficier ou en bénéficier pour des pilules qu'elle ne souhaite pas prendre au-delà de de ce problème, nous souhaitons demander un rapport sur 3 choses : tout d'abord l'extension de l'âge de 26 à 30 ans, et ensuite l'extension du public cible à la fois pour pour les hommes cisgenre genre et pour les hommes, transe, alors pour les hommes six Jean pour une raison assez simple parce que nous pensons qu'il serait temps, ça fait environ 2 millénaire que les femmes ont entièrement la charge mentale de la contraception et ce serait pas mal qu'on la partage un petit peu et la 2ème chose c'est les hommes, transe, tout simplement parce que les hommes transe peuvent avoir besoin d'accès à la contraception, on comprend pas bien pourquoi une personne qui serait une femme à l'état civil pourrait avoir accès gratuitement à la contraception et puis quand elle changerait son état civil. Cette personne n'y aurait plus accès, on nous a répondu que c'était il recevable parce que Arctique quarante mais je voulais juste vous juste une chose, en fait, ces personnes, ce sont les mêmes personnes, d'accord, ça n'aggrave pas les les charges, ce sont les mêmes personnes, elles y avaient droit soudainement, elle change, état civil, elles ont plus droit, mais en fait c'est c'est les mêmes gens, c'est les mêmes être s'humains, donc on comprend pas bien pourquoi soudainement ont retiré l'accès à un droit qui est un droit fondamental parce qu'on aurait eu accès à un autre droit qui est de faire changer son état civil. merci, avis de la commission. à toutes les femmes de moins de 26 ans, ainsi que sur l'opportunité d'élargir la prise en charge de la contraception des hommes si genre et des hommes transgenre jusqu'à 30 ans, voilà donc c'est c'est une demande de rapport, je vous propose le retrait des fois un avis défavorable. Monsieur le Ministre. C'est le président, mesdames les sénatrices messieurs sénateurs même avis que que la commission, sachant que de nombreux rapports sont déjà produits par Santé publique France par l'adresse par l'Insee sur la contraception, rapport supplémentaire ne semble pas nécessaire, je partage votre préoccupation sur la la contraception masculine, la charge de la contraception pesant trop sur sur les femmes, mais il faut toutefois que la HAS puisse se prononcer sur les méthodes de contraception masculine, qu'elle soit validée scientifiquement qu'elle soit disponible je comme je l'ai dit retrait ou avis défavorable. Alors donc un double avis défavorable sur l'amendement je le soumets aux voix qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient n'est pas adopté chou mais voit l'article 19 qui est pour. Qui c'est qui s'abstient, il est adopté, après l'article 19 l'amendement 963. Madame Bougel, mais elle vient de s'absenter. Madame Vogel. L'amendement 963. Vous savez moi, excusez-moi, excusez-moi, merci, alors récemment on a eu des débats très intéressant dans cet hémicycle sur l'introduction à la constitution du droit à l'IVG un des arguments qui a développé la droite de l'hémicycle pour s'opposer. Ah, cette PPL, c'était de dire ce qui est vraiment important c'est pas tellement le droit, c'est l'accès au droit, c'est ça qui est important, quelle ne fut pas notre surprise de découvrir qu'il avait pas tellement d'amendements. Ah ce PLFSS pour améliorer l'accès à l'IVG qui visiblement a été la grande préoccupation, ce dont je me félicite donc cet amendement, il a vocation à répondre à un des freins de l'accès à l'IVG en France qui est les surcoûts. Que ce soit l'éloignement géographique, parce que vous devez faire des kilomètres pour aller faire une consultation puis avoir accès à l'intervention puis parfois refaire de nouveaux tests souvent, enfin, c'est en France et ces coûts ne sont pas pris en charge, il y a des pays où c'est pris en charge en Angleterre, vous ferez de transport sont pris en charge qu'on vous avez accès à l'interruption volontaire de grossesse, c'est un coût qui est important, surtout quand on vit dans des zones où les soins sont éloignés de chez soi. Il y a parfois de nouveaux tests à faire qui ne sont pas nécessairement pris en charge et évaluer ces coûts, c'est une demande de rapport sur sur ces coûts évalués, ces coûts, ça permet de les mesurer et en les mesurant ça permettrait de les couvrir et en les couvrant, hé bien on ne ferait avancer en France l'accès effectif au droit à l'IVG et comme je sais que dans cet hémicycle, il s'est développé une forme de passion pour l'accès à l'IVG, je ne doute pas que cet amendement sera adopté avec enthousiasme.

je ne doute pas que ce il y avait pas eu l'article 40, vous auriez proposé un élargissement pour moins de reste à charge pour moi c'est un avis défavorable. C'est le président madame dessinatrice, messieurs les sénateurs, avis défavorable également en précisant que la loi du du 2 mars 2022, qui vise à renforcer le droit à l'avortement prévoit déjà la remise d'un rapport sur l'évaluation de l'accès des femmes à l'IVG et je pense que vous trouverez ces informations dans ce rapport.

monsieur lévrier. Et sa prise en charge par la Sécurité sociale : le Sénat refuse les rapports généralement mais pas systématiquement, bien par cet amendement, notre groupe souhaite mettre en lumière les disparités entre femmes et hommes en ce qui concerne les moyens de contraception en effet de nombreuses études montrent que les femmes sont davantage responsabilisés sur les moyens de contraception que les hommes avec la charge mentale que cela peut entraîner, il existerait donc des disparités en matière de connaissances liées aux moyens de contraception entre femmes et hommes, il apparaît fondamental de rétablir une meilleure répartition de la responsabilité de la vie sexuelle, cet amendement vise donc à réaffirmer notre attachement à l'égalité entre femmes et hommes en matière de responsabilité de la vie sexuelle, je vous remercie. Madame la rapporteure

c'est l'effet Suède ça donc notre collègue Martin lévrier a demandé. Très habilement remise d'un rapport relatif à l'information de la population sur la contraception et sa prise en charge par la Sécurité sociale avec un un sujet qui n'est pas sans importance, mais que je trouverai plus sage qu'on reporte dans que notre demande c'est une demande de retrait des fois un avis défavorable. je partage, monsieur le sénateur Iacovelli, votre objectif bien entendu d'information plus large de la de la population plus qu'un rapport, s'il vous plaît, vraiment utile de poursuivre les efforts d'information et de communication autour de de ces mesures, c'est le rôle de l'assurance maladie de santé publique France à travers entre autres son site son site question sexualité c'est aussi le rôle des professionnels de terrain, des professionnels de santé, des associations, même avis que la rapporteure retrait sinon avis défavorable. Pour retirer l'amendement monsieur lévriers bien ah on passe au débat sur l'article 20 avec de demandes de prise de parole Madame Cohen. Merci monsieur le président, je profite de cet article 20 qui vise à autoriser les femmes, les pharmaciens, sages-femmes et infirmiers à prescrire des vaccins pour intervenir sur un sujet d'actualité particulièrement grave pour le seul mois d'octobre, notre pays a détruit 4 millions de doses de vaccin Moderna utilisé contre la Covid 19 cette gabegie faite en toute discrétion, représente un montant de près de 80 millions d'euros, comme le révèle aujourd'hui le journal L'Humanité en mai dernier, ce sont plus de 3 millions de vaccins AstraZeneca qui ont subi le même sort, il est très probable que d'autres ont également été jetés à la poubelle, dans les mois précédents et que les mois à venir verront ce scénario se répéter au delà de la nécessité d'avoir la garantie d'un stock suffisant de vaccins de la question des dates de péremption et du fait que ces vaccins première génération ne soit pas très adapté au nouveau variant, nous sommes face à un véritable scandale sanitaire et financier dès l'arrivée des premiers vaccins nous avons dénoncé l'accaparement par les pays riches, des stocks de vaccins au détriment des pays pauvres, nous sommes en train de détruire des doses faute de les avoir utilisées quand de donc, quand de nombreux pays, n'y ont pas eu accès dès le début, nous avons dénoncé le manque de transparence dans les négociations avec les laboratoires et l'opacité des contrats sur les volumes, le calendrier de livraison, les prix au nom du secret des affaires, je vous invite à lire combien coûtent nos vies, enquête sur les politiques du médicament de Pauline non et Jérôme Martin, cofondateur de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, vous avez refusé de lever les brevets et par votre politique, vous avez permis à l'industrie pharmaceutique, de faire des profits des super profits, pour reprendre une expression très en très en vogue, le tout sur le dos de la pandémie 26 milliards pour Pfizer en 2022 12 milliards pour Moderna on voit le résultat aujourd'hui, alors Monsieur le mini, je vais vous faire un cadeau, je vais vous donner en main propre le rapport que j'ai fait sur la création d'un pôle public du médicament ainsi que la proposition de loi que nous avons fait au niveau du groupe communiste communiste républicain et citoyen, il y a beaucoup d'informations extrêmement intéressantes. Merci madame Cohen Monsieur Chassang. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais à nouveau moi salué la proposition du du gouvernement, de permettre aux pharmaciens, infirmiers, sages-femmes de prescrire des vaccins, je voudrais dire que les pharmaciens ont fait un très très gros travail au niveau de vaccination du du Covid donc actuellement les sages-femmes peuvent prescrire en plus des médecins, des vaccins, mais uniquement pour les femmes 1, rubéole étais n'était polio rougeole, oreillons papi papillomavirus et uniquement les BCG pour les nourrissons, les pharmaciens peuvent faire les vaccins que je viens de citer plus la grippe bien sûr, puisque la la grippe, il y a pas de de prescription alors les infirmiers peuvent administrer mais sur prescription médicale, l'ensemble des vaccins que je viens de citer également donc en 2022, monsieur le Ministre, la HAS et vous-même avez souhaité élargir les compétences aux pharmaciens, infirmières et sages-femmes pour prescrire et administrer donc la compétence de prescription administrations maintenant pour les pharmaciens, infirmiers, ça je sais pas pour les vaccins de tous les calendriers de bas de vaccination, sauf certains vaccins pour les personnes immuno-déprimées pour les mineurs, peu de à 16 ans, et donc je salue ses nouvelles compétences pour ces professionnels de santé après formation de certifier en vaccinologie, cela devrait permettre de simplifier beaucoup de parcours vaccinal de tous les assurés et avec le Mans que de médecins, permettre une facilité et améliorer le taux de vaccination merci. Merci Monsieur Chassaing, donc maintenant on examine trois amendements identiques, le 1er est présenté par Madame Gruny le 2 Merci monsieur le président, le présent amendement vise à exclure les mineurs de moins de 16 ans des dispositions de cet article afin de ne pas morceler le suivi vaccinal des enfants, considérant que la vaccination fait partie intégrante du suivi médical des nourrissons car incluse dans la ville, les visites obligatoires l'articulation des consultations obligatoires avec le calendrier vaccinal est un élément majeur dans les stratégies de prévention des pathologies de l'enfant en matière de dépistage et de diagnostic précoce, cet amendement ne s'oppose toutefois pas ne oui toutefois pas à l'habite mutation des infirmiers purée culteurs à pratiquer des actes de vaccination nourrissons dans le cadre strict d'une délégation de tâches dans le cas de cabinets médicaux ou de maisons pédiatrique par les infirmiers puériculture cette délégation de tâches doit être précédée d'une formation qui ne doit pas se résumer à l'apprentissage des techniques d'injection déjà plus compliqué chez l'enfant, mais aussi à des connaissances minimales sur les vaccins leur indication leur contre indication leurs précautions d'emploi, l'objectif est d'assurer un accompagnement spécifique des familles face à un geste anxiogène pour certains la phobie des piqûres et des vaccins contribue à des couverture vaccinale

et le vaccin doit se faire dans l'acte de consultation, il suit la consultation ouvrir la vaccination du nourrisson, à tous les paramédicaux, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus besoin de consultation, donc la crainte, c'est que certains parents face le vaccin uniquement le vaccin et n'est pas de de suivi classique du nourrisson avec un examen médical complet, c'est pour ça que je j'étais également favorable à à cette exclusion pour les moins de 16 ans du de la généralisation des vaccinateurs. Et Monsieur Hénault oui merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre, j'en profite pour saluer l'effort des pharmaciens en faveur de de la vaccination, mais pour ce qui concerne l'amendement s'est défendu. Merci madame la rapporteure. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement propose effectivement que l'article 20 ne s'applique pas aux mineurs de moins de de ses enfin de ne pas, je cite, ne pas morceler le suivi vaccinal des enfants, on comprend bien l'intention des auteurs, mais l'article n'impose aucunement que le suivi vacciner les enfants soit fait par des professionnels de santé différent, il ne vise qu'à pérenniser ce qui a été expérimentée avec succès lors de la campagne de vaccination récente, à savoir l'élargissement des compétences de l'administration et de prescription des vaccins à d'autres professionnels de santé. je voudrais juste dire que que ce soit pour les sages-femmes, les infirmiers et les pharmaciens, c'est une possibilité et que, et peut-être que Monsieur le Ministre, nous apportera des précisant mais que la prescription de certains vaccins pour chacune de ces pour pour chacun de ces professionnels de santé sera possible à partir d'une liste, y compris, que ce soit pour les vaccins ou pour les personnes susceptibles de bénéficier qui seront déterminées par un arrêté justement du ministre chargé de la santé et de la prévention, pris après avis de la Haute autorité de santé de l'Agence nationale de sécurité. Du médicament et des produits de santé, c'est-à-dire à à l'heure où on se parle, rien n'exclut, effectivement, que les les jeunes de moins de 16 ans ne puissent pas être vacciné mais rien ne le dit, non plus, donc peut-être que le ministre va nous éclairer en tout cas c'est une demande de retrait des fois un avis défavorable. Monsieur le ministre. Mon objectif dans cet article, c'est d'augmenter au maximum la couverture vaccinale de toute la population c'est de simplifier les parcours vaccinaux du du citoyen et et dans ce cadre-là, les recommandations de la Haute autorité de santé de juin 2022 sont particulièrement claires et et préconise d'étendre ses compétences à ces 3 professions y compris pour les enfants à partir de 2 ans pour donc pharmaciens, infirmiers et sages-femmes, bien entendu, l'extension de ses compétences liées à une formation préalable, en particulier pour la prescription des vaccins et et fera l'objet d'un décret concernant le type de vaccin et les conditions dans lesquelles ils peuvent être prescrits et réalisé pour toutes ces raisons, je suis l'avis de la rapporteure retrait sinon défavorable. Merci Madame Gruny. merci monsieur le le président, Monsieur le Ministre, l'inquiétude en fait, c'est que des enfants ne suis si Monsieur le Ministre, que des enfants ne soient mais voilà ne généraliste ou un pédiatre et sincèrement, moi dans mon département, on a une très grande précarité dans les familles il y a des enfants qui passe sous les radars ont fait milieu médical, donc moi je j'entends bien, en fait, votre sujet sur élargir la vaccination ça, moi je suis d'accord, mais en revanche, les enfants, ils doivent être vus par des médecins, donc si la prescription, elle est faite par d'autres professionnels de santé que qu'un médecin, moi je trouve que, on passe à côté à côté pour pour des familles, merci.

un vaccin comme le BCG peut être dangereux chez un n'en font immuno-déprimés, qui vous dit que que le le l'enfant qui va aller se faire vacciner chez une sage-femme, par exemple, qui n'a, qui n'a pas de formation au-delà du premier mois de l'enfant de la des 28 premiers jours qui vous dit que ces ces ses contre-indications seront respectés et par ailleurs, moi, je suis allée me faire vacciner contre la grippe chez mon pharmacien qui m'a qui m'a dit qu'il n'avait aucune envie de participer à la vaccination des nourrissons vacciner un nourrisson si c'est pas fait correctement, ça veut dire qu'il y aura un refus des vaccins ultérieur, y compris à l'âge adulte parce qu'il y aura une phobie de la piqûre, donc je pense quand même qu'il faut, il faut rester réaliste et considérer que que le Monsieur le Ministre, vous avez, vous parlez des assises de la pédiatrie, soit on considère que ce sont des métiers inutiles et qu'après tout, les pédiatres peuvent peuvent bien disparaître, soit on reconnaît vraiment l'expertise de ce métier, et en particulier l'approche des enfants avant de les vacciner. Monsieur Jomier. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre dans j'ai bien entendu votre vos propos sur l'avis de la HAS du mois de juin, mais dans son avis du mois de janvier 2022 sur l'extension des des pratiques vaccinales, la HAS recommande hé bien que ce soit limité aux enfants de plus de 16 ans donc que la HAS 32 avis opposé en six mois d'écart souligne simplement que le sujet mérite notre attention, et moi je trouve que nos collègues Gruny là Sarah No ont raison dans les arguments qu'ils avancent et qu'un principe de prudence, certes, on sait ce qui vous guide dans l'élargissement dans le la gestion de la pénurie actuelle de soignants, mais attention, attention à ne pas mettre en cause quand même une prudence sanitaire, les enfants de les moins de 16 ans et particulièrement les nourrissons sont exposés à des difficultés dans leur prise en charge si on élargit par trop les professions qui peuvent prescrire et ou administrer les vaccins, donc, pour notre part, nous voterons ces amendements. Monsieur le président, monsieur mise, mes chers collègues, je voudrais dire à mes collègues que les infirmiers actuellement sur prescription médicale, font des vaccins, ils font des vaccins aux nourrissons, je voulais également dire que il me semble bien avoir lu dans le projet de loi que ce n'est les les pharmaciens qui auront une formation les infirmiers ont qui l'ont et les sages-femmes ne feront les vaccins qu'après les, pour les enfants de 2 ans et plus, merci. Oui, simplement, sur prescription, c'est quand même différent, ça veut dire que l'enfant avait un médecin qui a prescrit donc c'est ça qui est important, moi on on ne peut pas cantonner exercé comme certains le le la médecine, on voit bien, vous Découvrez l'enfant quand il est malade, c'est-à-dire quand il a trente-huit ou quarante le soir ou à la période où on faisait bien sûr les permanences de soins ou le week-end, et cetera, vous Découvrez l'enfant, hein, si vous l'avez pas suivi régulièrement et notamment à travers les visites obligatoires et la vaccination,

il y avait des manifestement des comportements qui est, qui n'était pas ce qu'on voyait parce qu'on en avait quand même en vacciner quand même un certain nombre et donc on voyait bien la différence de moi j'attire l'attention

donc véritablement, j'aurais tendance à à voter cet cet amendement dans un 1er temps, quitte après à en faire le bilan et puis revenir et effectivement progressivement, quand on aura appris mais soyons quand même attentif à cela, Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, moi c'est pas en tant que médecin que j'ai réagi, mais plutôt en tant que père de famille en quelque sorte, hein, c'est-à-dire que moi, je suis très favorable, je l'ai dit d'ailleurs à tout mettre en oeuvre pour faciliter la vaccination mais, en revanche, il m'a semblé que pour les, les, les enfants et les plus petits enfants, il fallait faire preuve d'une plus grande précaution et c'est une forme de pragmatisme qui vaut cet amendement, je vous remercie. Madame la rapporteure. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la la position de la était au regard de la rédaction. Parce que, effectivement, ce n'était pas très clair puisque ça renvoie à un décret ou un arrêté un arrêté du ministre donc je je vous laisserai il travaillait Monsieur le Ministre, évidemment, à titre personnel, je partage ce qui a été dit. Je comprends, je partage il y a un sujet sur le plan la politique sanitaire, c'est la vaccination contre le papillomavirus à partir de, de 11 ans où nous sommes en retard, il faut le reconnaître dans notre pays, je crois qu'il y a à peu près un tiers des jeunes filles qui sont vaccinés et c'est peut-être 10 % des garçons malgré, là aussi, une campagne d'information et de promotion de la vaccination de la part des autorités sanitaires et de la caisse et des caisses primaires d'assurance maladie, voilà donc le ministre, moi je, je, je vais dire sagesse a-t-il personnel ou en tout cas voilà. Je j'ai bien compris je comprends aux attitudes a-t-il persuadé, encore une fois, je vous les partage, je partage vos questionnements et je fais aussi confiance parce que ce que dit le texte ces peuvent peuvent je fais aussi confiance aux professionnels de santé sur ce sujet là, mais votre votre arrêter Monsieur sera très important évidemment. Monsieur le Ministre, un mot avant qu'on vote. je peux au moins vous rassurer sur un point, c'est que les virus vivant atténué chez les immunodéprimés ne font pas partie de cette, de cette extension et son sont exclus toutefois je je pense et et je rejoins là aussi d'rapporteur de l'importance des retards qu'on a rattrapé certes sur le papillomavirus arrivent également demain le vaccin qui nous permettra de lutter contre la bronchiolite le VRS on aura pour l'hiver prochain, malheureusement on n'a pas, on n'a pas assez vite, il y aura une nécessité de vaccination extrêmement large et puis moi aussi je fais confiance aux professionnels, on est dans le cadre d'un exercice qui reste coordonnées qui est coordonné autour du médecin traitant dans une équipe de soins avec je vous en parlais tout à l'heure, mon espace santé ce carnet de santé numérique cette messagerie sécurisée pour échanger entre les professionnels de santé, je pense sincèrement qu'il faut là aussi faire confiance au au professionnel les travaux et et l'aboutissement des travaux au sein du Clio inter-ordres a justement ouvert la porte vers ce partage de compétences, je pense qu'il ne faut pas ici la refermer et et je maintiens donc un avis défavorable.

on va passer au vote, si, si vous voulez bien, donc, donc on a un avis défavorable du gouvernement et un avis de la commission qui est passé d'autres défavorables, un avis de sagesse voilà donc qui est pour ces amendements. Qui est contre. Qui s'abstient ils sont adoptés, on va passer au vote sur l'article 20 qui est pour l'article 20.

la loi de financement de sécurité sociale de 2000 pour 2021 a autorisé l'expérimentation d'un parcours d'accompagnement, ce parcours devait comprendre un bilan d'activité physique, ainsi qu'un bilan de consultation de suivi nutritionnel et psychologique pour les personnes pour lesquelles une complication du diabète de type 2 a été où avait été découverte les effets positifs de l'activité physique adaptée sur le traitement de cette affection sont clairement reconnu et de manière incontesté par toute la littérature médicale et scientifique, il permet ainsi de diminuer le coût de prise en charge, notamment par la baisse de consommation des médicaments or malheureusement

pour la publication du décret d'application à ce qui permettra aux patients atteints de de diabète de type 2, souffrant d'une complication de bénéficier de manière effective d'une, de cette avancée dans la prise en charge de leur pathologie. Merci à vie de Madame la rapporteure. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, découverte, alors en effet il ne semble pas que le décret d'application était pris, donc ça serait un avis favorable. Monsieur le ministre. Monsieur le président, madame la rapporteure mesdames les sénatrices messieurs des des sénateurs. Le travail préalable concernant, c'est la mise en place d'un tel parcours étant lieu étant en train d'être fait, pardon, avec les différents acteurs, il a rejoint le cas d'une expérimentation d'article 51 pour pouvoir justement faire cette co-construction avec les différents acteurs et les ARS dans la définition de l'organisation territoriale du parcours adaptés, il reste des questions sur le portage locales sur les systèmes d'information, qui sont là aussi fondamental, même si je je partage et je comprends votre volonté de d'avancer le plus rapidement possible la date butoir du 31 décembre 2023 semble un peu prématuré pour le, c'est pourquoi je suis défavorable.

sincèrement je trouve quand même incroyable, on a l'Assemblée nationale, on a le Sénat, on est là pour pour créer les lois pour les appliquer les suivre et en fin de compte, il y a des lois qui sont votées et les décrets sont pas appliquées, alors moi je veux bien, mais je suis tout à fait d'accord avec mon collègue, il y a pas besoin de plusieurs années pour pour faire un décret d'application, donc je pense que moi j'appelle à votre attention, un décret d'application, dire que il faut encore un an avant de le mettre en place, c'est quand même fort de café, voilà donc je vous laisse à la réflexion et je suis tout à fait d'accord avec mon collègue.

Merci monsieur le président, dans bon nombre d'établissements de santé, en particulier au sein des centres de lutte contre le cancer, les infirmiers exerçant en pratique avancée exercent des missions indispensables permettant une amélioration des prises en charge, complexe, ainsi qu'une optimisation générale de l'organisation des soins les IPA permettent d'améliorer le suivi des patients d'optimiser le temps médical de renforcer l'accès aux soins, pourtant le déploiement des IPA se heurte à des problématiques de financement d'opacité des rôles de rigidité des normes, il est nécessaire de réunir largement les acteurs du système de santé afin de tirer un bilan et d'élaborer des propositions concrètes pour améliorer leur déploiement.

Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement crée une conférence des parties prenantes, chargé de faire un bilan de la. Création d'auxiliaires médicaux en en pratique avancée des auxiliaires médicaux en pratique avancée sont désormais un rouage fondamental de notre système de santé, il est vrai que l'organisation générale n'est pas stabilisée, il y a des spécialités dans lesquelles nous aurions besoin d'en créer, nous avons par exemple proposé de faire en soins palliatifs dans le rapport, c'est au nom de la commission avec Michel Meunier Christine Bonfanti Dossat je ne suis toutefois pas certaine que la création d'une conférence des parties prenantes s'impose pour faire un bilan d'ailleurs le Champ de compétences et le recrutement des IPA font déjà partie des sujets abordés au sein du Conseil national, c'est une demande de retrait, à défaut, un avis défavorable. Monsieur le président, madame la rapporteure mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, même avis que la rapporteur en en précisant qu'il y a déjà une inspection IGAS et j'ai pendant le printemps et l'été 2000 22 et et les conclusions de ce rapport, permettront de traiter justement ces sujets donc, il ne semble pas utile. De convoquer une nouvelle conférence donc retrait sinon défavorable.

Merci monsieur le président, alors le présent amendement c'est un rapport, c'est donc un amendement d'appel relatif, un sujet de santé publique qui touche à de nombreuses femmes, le cancer du col de l'utérus pour lutter contre ce cancer, une solution a fait ses preuves, la vaccination contre les infections liées au peuple papillomavirus humains dit vaccin HPV aujourd'hui ce vaccin fait l'objet d'un remboursement à hauteur de 65 % par la Sécurité sociale, mais seulement pour les jeunes jusqu'à 19 ans et ils suivent suivant en cela les recommandations effectivement de la Haute autorité de santé toutefois, on a vu tout à l'heure qu'il y a très peu de vaccination que la France est nettement en retard et donc même si on connaît bon la raison de d'une vaccination, jeune, il nous semble que cette limite aujourd'hui est un peu trop basse à mesure que la société de mieux en mieux informés sur cette vaccination de nombreuses femmes voir de d'hommes souhaitent se faire vacciner, passé cet âge, aussi nous proposons que le gouvernement réfléchisse à lever cette limite de 19 ans pour améliorer notre politique de vaccination, je connais les réticences du Sénat vis-à-vis d'Aeroports mais puisque la politique vaccinale relève du décret c'était malheureusement le seul outil à notre disposition, je vous remercie. Merci madame la rapporteure. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues oui donc une demande de rapport sur la pertinence de l'extension du remboursement par la Sécurité sociale, la vaccination contre les infections liées au papillomavirus après consultation de la Haute autorité de santé et de la CNAM, un tel rapport sera en effet plutôt de la compétence de la Haute autorité de santé de la CNAM et s'il y a lieu de se prononcer sur politiquement sur l'extension des temps de cette couverture pour des motifs de de santé publique, je pense que déjà, il faudrait qu'on améliore, je ne dis pas que c'est pas un sujet mais je dis qu'il faudrait déjà qu'on améliore la couverture vaccinale chez les jeunes filles et chez les jeunes garçons, voilà au moins on aura parlé de ce vaccin, ce soir, dans cet hémicycle. Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, madame la rapporteure mesdames, une sénatrice, messieurs les sénateurs, l'heure est tardive, mais le le sujet est essentiel sur la vaccination du papillomavirus c'est un un sujet de santé publique majeur qui m'interpelle, de façon extrêmement importante. La vaccination contre le papillomavirus une une méta-analyse comme on dit récente sur 14 pays qui l'ont développé, mais essentiellement chez les filles, montres que ça diminue des 2 tiers, les cancers du col de l'utérus et de 50 % les lésions précancéreuses si on regarde ce qui est fait en Australie où il y a une vaccination large des garçons et des filles, les Australiens envisagent la disparition du cancer du col de l'utérus à échéance 10 ans et également une diminution drastique des cancers ORL mais également des concerts à recto donc cette vaccination est essentielle. Je me permets là de de faire une remarque et de regretter un peu votre décision concernant l'amendement précédent parce que cette vaccination doit avoir lieu avant les premières relations sexuelles donc plutôt à l'âge de 11 ans et ils nous auront tout intérêt à laisser d'autres professionnels là réalisé en particulier, les pharmaciens, c'était une remarque, je me devais de faire concernant la demande de ce rapport, l'extension et pris en charge par la Sécurité sociale aux garçons et aux filles date de 6 mois, il me semble vraiment prématuré de demander un rapport mais en tout cas c'est un enjeu majeur de santé publique, je le redis, ça fait partie des réflexions que j'ai demandé à la Haute autorité de santé aussi dans le cas des obligations vaccinales, donc nous aurons bien entendu l'occasion de d'en reparler, je suis donc défavorable, vous l'avez compris à cet amendement. Un double avis défavorable, je le soumets aux voix qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté, nous allons arrêter la l'examen des amendements pour cette séance, je vais donner la parole à monsieur Serge mais Riou pour une mise au point au sujet d'un vote. Oui, donc il s'agit d'un correctif sur le scrutin public numéro 34 portant sur l'amendement 1039 rectifié pour le groupe socialiste, écologiste et républicain, monsieur le président, donc le groupe socialiste écologique et républicain souhaite procéder aux correctifs suivants concernant le scrutin public numéro 34 Hervé et Joël Bigot Sabine Van Gogh Yannick Vaugrenard souhaité voter contre cet amendement énorme voté pour Gilbert Luc devina souhaité s'abstenir sur cet amendement et n'ont voté pour, je vous en remercie. je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 21 heures 30 pour la suite de l'examen de ce texte, la séance est suspendue.